la séance est reprise, l'ordre du jour appelle l'examen des crédits de la mission Agriculture alimentation forêt et affaires rurales et les Arctic 41 c'est Et la discussion du compte spécial développement agricole et rural du projet de loi de finances pour 2023. La parole dans cette discussion est à monsieur Patrice Joly, rapporteur spécial de la commission des finances. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur général, madame la présidente, mon cher, mes chers collègues, chers collègues corapporteur la mission Agriculture alimentation forêt et affaires rurales s'inscrit en 2023 dans la mise en oeuvre de la nouvelle politique agricole commune pour la période 2023 2027 qu'il représente pour la France sur l'ensemble de la période, une enveloppe de 45 2 milliards d'euros, les crédits de cette mission s'élève en 2023, quant à eux à 3 8 milliards d'euros, soit un peu moins de 30 % d'augmentation par rapport à 2022, à périmètre constant, cela ne représente plus que 15 % et en tenant compte de l'inflation, cela représente une hausse de 8 pour des sujets majeurs concernant en particulier l'alimentation et la forêt, il ne s'agit rien de moins que de répondre également aux défis climatiques, économiques, géopolitiques et le plus important de tous, le défi humain qui menace nos agriculteurs rempart de notre souveraineté alimentaire ce budget prend en compte un certain nombre de ces défis tout d'abord la réforme de l'assurance-récolte qui entrera en vigueur le 1er janvier prochain et qui crée un dispositif universel de couverture des risques partagés entre les agriculteurs, les assureurs, et l'État, le montant total de l'enveloppe, publique, et de 560 millions d'euros en 2023 pour cette réforme nécessaire, on peut craindre que le soutien public soit insuffisante 600 millions d'euros avaient en effet été annoncé une autre réforme concernant la nouvelle répartition des aides non surface entre l'État et les régions sera mis en oeuvre, celle-ci relevait jusqu'à présent de l'État, elles sont transférées aux régions, désormais, il s'agit notamment du soutien aux investissements des aides à l'installation des jeunes agriculteurs et des aides au développement local, une exception toutefois : Mayotte, les aides non surface il demeure quant à elle, sous l'autorité de l'État, cette nouvelle répartition se traduit par la budgétisation de 100 millions d'euros, s'agissant du dispositif d'exonération de cotisations patronales de Sécurité sociale, dit TODE, il sera intégralement financé en 2023 sur les crédits budgétaires de la mission cette exonération tend à faciliter l'emploi de la main d'oeuvre nécessaire à la réalisation des travaux agricoles saisonniers, ces exonérations ne seront plus compensées par une fraction de TVA, comme l'an dernier, ce qui constitue un élément de fragilité pour la pérennité nécessaire de ce dispositif dans le domaine de la sécurité alimentaire, on peut saluer la création d'une police unique dont la dotation s'élève à plus de 654 millions d'euros, soit une augmentation d'à peu près 7 % par rapport à 2022, la nouvelle politique unique chargé de la sécurité alimentaire tend à répondre à des besoins de lisibilité réactivité et efficience des contrôles, la direction générale de l'alimentation deviendra l'organisme de contrôle officiel en matière de sécurité alimentaire des aliments à total de 150 ETP lui sera affecté par transfert pour 60 ETP de la direction générale de la on se c'est pour une paye par une création de quatre-vingt-dix ETP, la question de la localisation des agents sera déterminant sur l'efficacité de cette nouvelle organisation, l'enjeu n'est pas mince si l'on a en tête les affaires parfois d'armes dramatiques des plus anciennes avec du cheval dans les raviolis ou dans des plats cuisinés au plus récentes avec des steaks hachés et des pizzas contaminées par la bactérie E-coli en dépit des réformes et de l'augmentation de certaines dotations plusieurs constats demeure alarmant : tout d'abord s'agissant de l'agriculture biologique, je tiens à rappeler que la Commission européenne a demandé en avril à France de revoir son plan stratégique, critiquant le faible niveau d'ambition environnementale et climatique, avec notamment un soutien insuffisant du bio. Le gouvernement a présenté sa nouvelle version, début juillet, avec de nouveaux arbitrages proposant de rehausser les aides des éco-régime pour les exploitations en bio et de renforcer les exigences en matière d'eau de biodiversité de réduction des pesticides du Label haute valeur environnementale, objet de nombreuses critiques des défenseurs de l'agro-biologie la filière est aujourd'hui en difficulté, sans que l'on sache, il s'agit d'une situation conjoncturelle ou structurelle, la croissance du marché du bio, c'est en effet interrompu en 2021, avec une baisse de 3,1 % des ventes par rapport à 2020, cette baisse de consommation est inquiétante, tout autant que celle des produits agricoles en général aussi, je veux, je ne peux que déplorer vivement la promesse que la promesse de campagne présidentielle d'un chèque alimentaire n'ait pas été tenues à ce jour 2ème alarme concernant l'état de nos forêts tout d'abord permettez-moi, Monsieur le Ministre, de regretter que la dénomination de votre portefeuille nos mentionne plus la forêt alors même que celle-ci est confrontée à de nombreux défis l'an dernier nous observions déjà que la filière était confronté à des difficultés économiques, tandis que l'Office national des forêts traversait de grandes difficultés, le Conseil sont aujourd'hui certes une amélioration de l'office mais très conjoncturelle, en tout cas très liés au marché et du bois, or l'office électeurs essentiel de la préservation de nos forêts, celles-ci sont aujourd'hui plus que jamais atteintes par la sécheresse et les incendies, il n'a qu'à voir ce qui s'est passé au cours de l'été dernier les forêts sont menacés de dépérissement à horizon 2050 et environ 230 E 30 % d'entre elles risquent de basculer en situation d'inconfort climatique, il appartiendra à l'ONF de procéder à des renouvellements d'espèces à un rythme double de celui que l'on constate ordinairement 70000 hectares contre 40000 ne peut relever qu'on ne peut relever que par la réduction constante des employes constaté au cours de ces 3 dernières années, alors on peut avoir des doutes sur le caractère surprise suffisant des crédits qui sont dédiés à la forêt et qui, aujourd'hui, conduisent à une perte de 20 équivalents temps plein dans les effectifs de l'ONF dernier constat concerne notre souveraineté alimentaire et celui du danger qui pèse sur le renouvellement des générations d'agriculteurs sur le renvoie à la question de leurs revenus de la transmission des exploitations et de l'installation des jeunes, les chiffres sont évocateurs : la population agricole et celle qui est plus touchés par la pauvreté et 10 % des agriculteurs les plus modestes ont revenu qui ne dépasse pas 9800 euros, il est temps de répondre à ces éleveurs et maraîchers et autres producteurs qui travaillent sans revenu décent quant à la transmission c'est constitue l'angle mort des la politique publique en matière agricole, avec une perte de 260000 exploitants depuis 2000 depuis 2000. En août 43 % des Fatton 55 ans ou plus, c'est pourquoi un soutien plus actif aux entrons comme au sortant s'impose.

du développement rural, il ne pourra être adopté que si l'ensemble des crédits qui sont affectées sont utilisés pour la recherche appliquée dans le monde agricole, je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur, et la parole est maintenant à Vincent Séguin, rapporteur spécial de la commission des finances.

Monsieur le président, Monsieur le Ministre, madame la présidente, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le 28 septembre dernier la commission des affaires économiques rendait son rapport sur la ferme France un rapport alarmant sur la perte de compétitivité mesurée sur les 20 dernières années, je cite, alors que le commerce international de produits agroalimentaires n'a jamais été aussi dynamique, la France est l'un des seuls grands pays agricoles dont les parts de marché recule. Les exportations sont uniquement porté par les vins et les spiritueux et Doren amant plus de la moitié des denrées consommées sont importées, ces pertes de marché sont dues à la perte de compétitivité de la ferme France qui je le rappelle, est due à un coût de travail élevé à la surtransposition de règles environnementales à l'interdiction de construction de retenues d'eau, ou plus généralement à la prévention des aléas climatiques, qui entraîne des pertes de rendement et de volume et surtout à la stratégie de montée en gamme des produits agricoles et agroalimentaires menée depuis 2017 sans un raisonnement adapté par filière. On aurait pu croire que dans le pays où l'industrie du luxe et bénéficiaire, la stratégie de la montée en gamme soit opportune, mais c'est ignorer le besoin de consommation et de pouvoir d'achat des Français et je pense que nous faisons fausse route à titre d'exemple, on critique la production de volaille en batterie par rapport au bien-être animal, mais en même temps on apporte des poulets issus de ces élevages pour la consommation quotidienne des Français, la restauration hors domicile. On interdit le diméthoate pour la culture de la cerise, on risque de perdre des producteurs français, faute de récolte en même temps on importe de la cerises de Turquie sans vérifier s'il reste des résidus de diméthoate sur les fruits. On laisse détruire des réserves d'eau pourtant autorisée administrativement pour faire face au réchauffement climatique, pourtant nous sommes conscients qu'il va tomber toujours autant d'eau mais différemment avec des mois d'hyper sécheresse et des mois d'hyper plus. La quantité d'eau prélevée au moment où nous en auront le plus besoin va diminuer, il faut donc repenser à notre stratégie de réserve de combien d'autres exemples existent la balance commerciale de moins en moins excédentaire et les alertes que nous lançons pour l'agriculture depuis ces dernières années, rappellent celles qui ont été faites au moment des choix de désindustrialisation de la France nous compte, nous connaissons les conséquences et faisons seulement machine arrière, je tiens à le répéter. Pourtant, à la lecture du budget de la mission Agriculture alimentation et forêts, nous observons une augmentation du budget de 29,88 %, comme vous l'a rappelé mon collègue Patrice Joly, à l'instant. Si tout se résumer au budget, nous pourrions penser que tout ira mieux, mais encore une fois, je suis persuadé que nous ne réglerons pas tous les maux par de l'argent public est de plus en plus j'ai le sentiment que les ministères font la course aux dotations supplémentaires plutôt qu'à la maîtrise et à l'efficience de l'utilisation de ces dotations. Rappelons cependant que l'augmentation du budget est en partie due à la mise en place de l'assurance-récolte qui définit dorénavant le rôle de chacun entre l'agriculteur, l'assureur et l'État, cette ligne budgétaire et donc plus sincère et évitera sûrement des PLFR mais nous regrettons que le budget de 600 millions ne soit pas inscrit dans sa totalité 560 millions pour subventionner 70 pour 100 des cotisations de l'assurance et pour intervenir au-delà de 50 % de perte sauf en arboriculture et en prairie où on interviendra à partir de 30 %. C 560 millions sont financés à hauteur de 120 millions par le fond FN Gerra contribution des agriculteurs 185 millions par le Feader issu de la PAC et le reste par le budget de l'agriculture, cette assurance était attendue, puisque je vous le rappelle, ne récolte sur 5 était perdu et que cela démotive les jeunes à la reprise, la ferme France perd de la compétitivité à cause d'un coup de travail élevée, c'est pour cette raison qu'il a été mis en place le Théo de qui vise à exonérer ses charges sociales sur les emplois saisonniers reconduit pour 3 ans par les députés, nous souhaitons qu'il devienne pérenne pour l'installation des jeunes qui emploient de la main-d'oeuvre afin qu'ils fassent un prévisionnel stable et rentable sur le temps long. Bien sûr, cet amendement n'a pas été repris dans le 49 3 du PLFSS et nous regrettons encore de ne pas avoir été entendue et suivie. Perte de compétitivité parce que nous nous imposons à nos agriculteurs, des normes supplémentaire sur l'emploi des produits et sur les installations qui n'apporte pas de rentabilité complémentaires, ces normes françaises que nous imposons ne sont pas revalorisées dans les prix de vente parce que l'ensemble des Français n'a pas le pouvoir d'achat extensible la filière bio a eu le mérite de mettre une qualité sur un prix, mais cela restera un marché de niche, nous le voyons avec la hausse de l'inflation, tout le monde a envie de manger mieux, mais le portefeuille des Français fixe les limites. Bilan nous important sans contrôler aux frontières, la qualité des des produits par rapport aux normes françaises, pire, nous renforçons les effectifs pour contrôler les fermes françaises au risque de continuer à les décourager, il est temps que l'administration accompagne l'économie plutôt que la contrôler et la sanctionner enfin les agriculteurs finance chaque année, le Canada, hauteur de 140 millions ce fonds est fléchée vers la recherche pour trouver de nouvelles variétés face aux aléas ou des vaccins, le budget plafonne à 126 millions d'euros et n'est pas utilisé dans sa totalité, faute de projet, comment le ministère de l'agriculture peut-il se satisfaire de cette situation depuis tant d'années pour conclure le ministère doit fixer des objectifs en matière de politique agricole pour rétablir la situation économique actuelle et retrouver à la fois notre compétitivité, mais aussi et surtout notre souveraineté alimentaire, nous attendons donc des réponses sur Laurent, renforcement des contrôles aux importations avec l'application des clauses miroirs le développement de la recherche pour adapter nos productions végétales changement climatique et des vaccins face aux maladies, nous attendons l'application d'une politique de l'eau qui satisfasse l'environnement de et l'agriculture, avec une autorité de l'État face aux perturbateurs, nous attendons, enfin la suppression des sur-transpositions aux règles qui affaiblissent notre compétitivité compétitivité face à ces attentes, et contrairement à l'esprit du Sénat qui est habitué au consensus et qui cherche toujours le compromis. La commission des finances, a décidé de rejeter le budget de la mission Agriculture pour être en cohérence avec ce rejet le demanderont le retrait des amendements à nos collègues, même si nous nous empêchons pas de donner un avis. J'espère cependant Monsieur le Ministre, que vous prendrez le temps de répondre à ces questions et surtout que vous retiendrez dans le 49 3 les plus importants pour faire face, je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur spécial, et maintenant la parole est à Laurent Duplomb, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. C'est le président monsieur le 1er ministre, mes chers collègues. Monsieur le Ministre de l'Agriculture, excusez-moi, mes chers collègues. au vu d'un budget qui paraît aussi séduisant, il est vrai qu'on aurait pu penser pouvoir parler, peut être 1er ministre ce budget étant séduisant, certes, mais malheureusement tranports avoir ce budget a augmenté de plus de 900 millions d'euros et atteindre presque 4 milliards d'euros, nous pourrions-nous dire tout simplement, enfin ils ont compris, hé bien non, ceci est trompeur parce que, en fait, ces 900 millions se résume en 3 lignes qui elles ne sont malheureusement pas très séduisante c'est la ligne de 400 millions d'euros correspondant à une mesure de périmètre qui consiste à basculer le budget du TO-DE sur le budget de l'agriculture, avec une petite particularité, c'est que le président de la République nous dit au Salon de l'agriculture nous allons pérenniser le TO-DE et dès que nous vous proposons de le faire par le 49 3, vous nous dites : ben non, on va le repousser que jusqu'en 2026. Transports aussi les 200 millions d'euros, qui a vu à l'inflation sont rajoutés au budget qui est aussi une mesure de périmètre si on le prend sous cet angle-là, correspondant à la réalité de l'actualité de l'de l'inflation, 5 pour 100 enfants 200 millions malheureusement à 7 % nous serions un peu traite à 280 millions et puis enfin 255 millions qui consiste, qui constitue avec l'aide européenne et la participation à hauteur de 120 millions des agriculteurs au budget de l'assurance-récolte là aussi c'est un peu trompeur puisqu'après toutes les annonces qui ont été faites, le principe d'avoir accepté, comme l'a dit mon collègue Vincent les 4 qui ont été écrit dans la loi à la sortie de la, de l'examen au Sénat, hé bien, c'est pas 560 millions d'euros que vous auriez dû écrire : Monsieur le Ministre, mais 680 au-delà de cette problématique, mathématiques, il reste quand même sur l'assurance-récolte des points précis à examiner et à finir de régler dans un espace très court puisque je vous le rappelle, il faudrait que tout cela soit réglé définitivement pour le 1er janvier de l'année prochaine, nous avons encore et toujours la problématique de la moyenne olympique encore et toujours, même s'il semblerait que ça avance, la problématique de l'évaluation indiciel lié au satellite pour les prairies et puis enfin une petite nouvelle que je dont je me suis aperçu cette semaine pour avoir moi-même essayer de faire calculer le coût de mon assurance récolte c'est l'actualisation des grilles des barèmes d'un désir simplement pour que vous compreniez bien quand vous indemniser une tonne de maïs en matière sèche à 111 euros la tonne, hé bien tout simplement, vous êtes pas du tout sur le montant d'une tonne de maïs que vous auriez été obligé d'acheter puisque, par définition, c'est 3 fois plus important alors Monsieur le Ministre, un budget que nous aurions que pu adopter peut être voté aurait été un budget qui crée la confiance, le TO-DE ne la créent pas l'assurance ne récolte non plus au vu du montant que vous y mettez là sur le, sur le budget que nous aurions pu voter, c'est un budget qui prend en compte les enjeux, les enjeux de souveraineté les enjeux dans les agriculteurs vous font par tous les jours où ils vous disent très clairement, nous, nous en avons marre des contraintes et d'énormes et, malheureusement, hé bien ce budget comme tous les autres ils laisse planer la possibilité de continuer d'en rajouter sans cesse et de se dire que dans le même temps nous ouvrant les portes aux importations. parole, la parole est maintenant Madame Françoise Férat, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Merci monsieur le président, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission, chers collègues, le débat sur les crédits, agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales a été écourtée à l'Assemblée nationale par l'activation de l'article 49 49 alinéa 3 de la Constitution, en plein milieu de l'examen de la mission, ce qui a pu engendrer une certaine frustration, je suis heureuse que ce débat puisse avoir lieu au Sénat Jacques dans les temps très limité, qui sont les nôtres, je partage ce que vient de dire notre co-rapporteur Laurent Duplomb ce budget est insuffisant, d'un point de vue économique, il est aussi d'un point de vue social dans ses conséquences pour le métier vécue au quotidien par les agriculteurs. J'en veux pour preuve les crédits là en application de la feuille de route pour la prise en charge du mal-être agricole tout nous déplorons au passage la dispersion et du coup, le manque de lisibilité, le rythme de décaissement de l'aide à la relance des exploitations agricoles la Aria laisse à désirer, alors qu'elle est vitale pour les agriculteurs en détresse si sous-consommation il y a, elle, n'est pas à mettre sur le compte d'un manque de besoin mais plutôt du non-recours la pression psychologique et normative subis par les agriculteurs, compliquant leur accès à des aides auxquelles ils ont droit, autre élément de soutien en milieu rural, on devrait profiter des économies réalisées sur les stages tutoré vétérinaire qui donne d'excellents résultats avec 80 % de maintien dans la zone concernée pour en créer de nouveaux, ce n'est pas le cas s'agissant de la santé animale, il manque six petits millions d'euros pour la mise à jour des bases d'identification animale, portée notamment par les chambres d'agriculture dans le contexte de crise sanitaire que l'on connaît, il s'agit pourtant d'un outil essentiel de traçabilité et de surveillance dans une logique préventive toujours dans cette même logique, non pas tant face à l'influenza aviaire comme anticipation des autres crises qui ne manqueront pas malheureusement d'éclater, nous proposons une multiplication par 10 des crédits dédiés à la recherche de vaccination en santé animale comparé aux milliards d'euros d'indemnisation depuis l'an dernier ce te hausse ne paraît pas exagéré et surtout, elle est en phase avec notre conviction que les solutions pour l'agriculture de demain sous doit trouver dans la recherche et la science comme vous le constatez, Monsieur le Ministre, notre opposition et constructive malgré nos différences alerte ce budget n'est pas à la hauteur de l'ambition que nous souhaitons porter pour notre agriculture, monsieur le Ministre, croyait que je le regrette infiniment, je ne pourrai pas voter ce budget. la parole est maintenant à Jean-Claude Tissot, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Monsieur Monsieur le président, Monsieur le Ministre, madame la présidente de la commission des affaires économiques, messieurs les rapporteurs spéciaux, chers collègues, Laurent Duplomb a insisté sur la faiblesse économique de ce budget, Françoise Férat, à l'instant sur sa faiblesse social et sociétal et je compléterai notre travail d'équipe en insistant sur sa dimension environnementale qui ne me semble pas non plus à la hauteur pour adapter notre modèle agricole au changement climatique, il est essentiel d'investir dans l'expérimentation de nouvelles plaques pratiques culturales et de maintenir une recherche et innovation agricole au niveau de ce fait, un mot sur le casse d'art dont année après année les recettes continuent d'être plafonné et on ne voit pas bien la logique budgétaire, Monsieur le Ministre de cette sous-estimation, en effet, vous nous aviez dit en audition que vous vous engagiez à récupérer de l'argent, enfin l'excédent de cette collecte de 17 millions d'euros en 2022 donc pour 2023, les recettes sont et sont estimés à 126 millions d'euros, comme cette année, alors qu'avec l'inflation, les recettes continueront de grimper les programmes de recherche appliquée des instituts techniques nécessitent pourtant de la visibilité, pour cette raison, nous appelons au rejet des crédits du CASDAR nous appelant en outre à accélérer l'effort d'un temps d'identification des crédits mobilisables sur le sol de comptable du CASDAR pour prendre de l'avance sur la programmation 2022 2022 2027 du PND, l'adaptation au changement climatique n'attend pas sur la forêt, les feux de cet été ont souligné la nécessité de plus de surveillance dans les massifs et de plus de gestion durable, c'est pourquoi nous appelons à renforcer les crédits et les effectifs de l'ONF et du CNPF, car il ne faut pas oublier que la forêt privée représentent trois quarts des surfaces et 90 % des surfaces qui ont brûlé cet été sur l'ONF, le gouvernement n'a pas contribué à la clarté des débats, bien au contraire, en supprimant dans le budget initial, puis un rétablissement de l'Assemblée nationale 80 postes rétablissant d'ailleurs rétablissement pardon d'ailleurs partiel puisque seuls 60 postes sont vraiment financé par l'État, l'ONF devant prendre en charge des 20 postes restants en parallèle, nous appelons augmenter d'autant les effectifs du CNPF pour dynamiser la gestion et créer des postes de référent incendie conjointement avec les membres de la mission de contrôle sur la prévention des feux de forêt, des, des, des amendements qui qu'on qu'on nous défendrons tout à l'heure je tiens également à souligner que les 5 amendements proposé par la commission des affaires économiques ne coûte pas plus de 30 millions d'euros mis Boutabout, soit à peine 1 des crédits de la mission ils sert souvent à financer le dernier kilomètre d'une politique publique, inachevé, de ce fait, nous espérons que le gouvernement reprendra certaines de nos propositions Monsieur le Ministre. Peu coûteuse et inutile. Merci Merci donc dans la suite de notre discussion, je vous rappelle que le temps de parole attribués à chaque groupe pour chaque unité discussion qu'on prend le temps d'intervention général et celui de l'explication de vote par ailleurs le gouvernement dispose au total de quinze minutes pour intervenir, donc la parole dans la discussion générale, Bernard buis pour le groupe RDPI. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, madame la présidente de la commission des affaires économiques, messieurs les rapporteurs spéciaux, Madame et messieurs les rapporteurs pour avis, mes chers collègues, autant éviter tout suspense inutile d'autres groupes politiques ne s'associera pas au concert de critiques et de commentaires plus ou moins acerbes que l'on entend ici ou là, nous voterons les crédits de cette mission, car ils sont à la hauteur des enjeux, le décor est planté, nous le savons, notre modèle agricole ne vit pas un long fleuve tranquille enjeux climatiques géopolitiques, socio-sanitaires et technologiques, l'agriculture française vit actuellement de profondes mutations, d'abord avec le défi conjoncturel lié à la guerre en Ukraine, la montée des prix de l'énergie la hausse record des prix des engrais qui pousse les agriculteurs à retarder leurs décisions d'achat d'engrais et donc de plantations risquant d'affecter la récolte en 2023, ensuite avec les défis structurels, comme les conséquences du dérèglement climatique, le renouvellement des générations et les attentes grandissantes en matière d'alimentation durable que Seine enfin au bout du chemin, il y a la souveraineté alimentaire qui est la priorité de ce quinquennat mis en musique par le plan France 2030 face à ces nombreux enjeux le ministère compétent et plus globalement ce gouvernement sont au rendez-vous, en augmentant les moyens financiers, on peut débattre indéfiniment du niveau de la hausse prévue par cette mission mais selon nous, ce qui compte réellement, c'est de savoir si les investissements prévus par l'ensemble des programmes répondent aux attentes de nos agriculteurs et des défis de notre modèle agricole, mes chers collègues, j'aurai la faiblesse de penser que oui, arrêtons-nous quelques instants sur les points saillants de cette hausse budgétaire le programme 149 programme au moteur de la mission était en baisse l'année dernière il progresse désormais de 21 %. Une hausse qui s'explique principalement par la mise en oeuvre de la forme de l'assurance-récolte vous savez comme moi que, face aux sécheresses à répétition face aux gelées tardives ou aux fortes pluies, cette réforme était très attendu par la profession, les agriculteurs drômois particulièrement impacté ces 2 dernières années par les épisodes de gel et de grêle on parle régulièrement quelques mois seulement après son adoption au Parlement la réforme est en ordre de marche, la majorité sénatoriale a d'ailleurs pleinement participé à l'élaboration de cette loi. Que dit ce budget 680 millions d'euros sont visés pour le triennal, sachant que 560 millions d'euros sont déjà mis sur la table 256 millions inscrit noir sur blanc, qui s'ajoutent aux 185 millions d'euros de crédits européens et aux 120 millions d'euros de taxe affectée que demander de vous, de plus, mes chers collègues, j'évoquerai également l'action numéro 26 et la gestion durable de la forêt, le dérèglement climatique, a des conséquences dramatiques sur notre biodiversité qui plus est sur nos forêts en 2022 pas moins de 65000 hectares de forêts sont partis en fumée, nous nous sommes rapprochés des records de 1976 et 2003 devant pareil drame écologique je salue l'engagement de ce gouvernement visant renouveler 10 % la forêt française, de 10 mais pour parer à l'urgence, je salue surtout les 20 millions d'euros supplémentaires dirigée vers l'ONF qui permettront de mettre fin, enfin un terme aux suppressions d'emplois, l'occasion également de souligner le renforcement des crédits dédiés aux besoins des patrouilles de surveillance et de contrôle réalisé par l'ONF, la prévention et la gestion face aux crises sanitaires sont également des priorités de cette mission, nous vivons dans un contexte d'atteinte citoyenne forte et justifiée en l'occurrence la réduction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques la prise en compte du bien-être amical animal ou encore l'objectif de 50 % de produits de qualité dont 20 % de produits bio dans nos cantines en progression globale de 7 % nous saluons la mise en place de la police unique en charge de la sécurité alimentaire des aliments qui devrait à terme être plus lisible, plus réactive et plus efficience, mais aussi plus coercitives, par ailleurs, réjouissons-nous que la couverture géographique des projets alimentaires territoriaux, cher à notre collègue Frédéric Marchand est fortement augmenté en 2021 passant de 65 % à 97 % sous le double effet de la simplification de la procédure de reconnaissance et d'un renforcement du soutien à l'émergence de ces projets en fait si l'on ajoute à ce budget, le plan France 2030, qui apporte de 9 milliards d'euros à l'agriculture, en apportant son soutien à l'innovation et au développement des entreprises agricoles à travers des financements de projets, on peut considérer que ce budget se donne les moyens de financer tant les besoins impératifs de nos agriculteurs, que des nouvelles fondations basée sur l'innovation et l'agroécologie pour le renouvellement des générations, à ce propos, je salue également les crédits consacrés à l'enseignement agricole qui atteignent un total de près de 2 milliards d'euros, c'est donc un budget ambitieux et visionnaire que notre groupe s'apprête à voter, il est donc étonnant que la majorité souhaiterait trattoria le souhaite le rejeter un choix d'autant plus étonnant que vous avez approuvé l'année dernière, ce budget en commission des finances, pourtant en stagnation, mais il est encore plus étonnant, refusé de voter les crédits en commission, tout en proposant de multiples amant demain, permettez-moi de m'interroger sur la cohérence d'une telle méthode, vous l'aurez compris pour notre groupe, il n'y a aucune raison objective de rejeter cette mission et j'invite les groupes politiques qui partagent cet avis à faire preuve de responsabilité, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est maintenant à Franck Montaugé pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Monsieur Monsieur le président, monsieur le ministre et chers collègues, en considération des mesures budgétaires agricole de l'État et de la sécurité sociale, ainsi que de la nouvelle PAC, la France va consacrer 23 virgule 3 milliards d'euros à son agriculture en 2023 corrigé des mesures de transfert TODE à notre sécurité sociale et état le TO-DE, qui au passage existe toujours grâce à la volonté politique constante et unanime du Sénat les crédits augmentent de 460 millions d'euros à 5 % d'inflation, hypothèse basse pour 2023, il aurait fallu, à périmètre constant, 700 millions d'euros supplémentaires dans ce budget global pour retrouver le niveau de soutien de 2000 22 et de 140 millions si on met de côté la PAC, le budget que vous nous présentez ne va donc pas dans le sens d'un renforcement des moyens consacrés à la souveraineté alimentaire, à la différence de ce que le récent rapport de la commission des affaires économiques du Sénat sur la souvent été économique jugent indispensable de faire les dispositifs de soutien que vous déployez sont insuffisants, c'est ce que nous disent aux nombres d'exploitants, le gouvernement est attendu là dessus de manière plus ciblée sur quelques dispositifs à fort enjeu, je constate en matière d'assurance, la difficulté de budgéter les sommes nécessaires, l'épisode de gel de 2021 a coûté un milliard d'euros à l'État, le dispositif prévu pour 2023 toutes lignes confondues, dont celle du Feader nous amènera au mieux à 560 millions d'euros, on voit ici la fragilité du dispositif, côté recettes par rapport aux besoins et on s'interroge toujours sur les effets délétères qu'aura la moyenne olympique sur les remboursements de payer aux assurés, il y va de l'acceptabilité de l'assurance par les aveugles pour les agriculteurs eux-mêmes comment Monsieur le le ministre, envisagez-vous de contourner cette règle de l'OMC dans les USA s'affranchissent avec toujours moins de scrupules, nous attendons beaucoup du président de la République à ce sujet des mesures fortes dans l'intérêt 1er de nos filières agro-agroalimentaires notamment un bail européenne acte est indispensable, je note positivement le milliard d'euros prévus pour la grippe aviaire mais cela me paraît insuffisant pour couvrir la valeur ajoutée, perdu à chaque étape de la chaîne des producteurs aux consommateurs, je vous exprime aussi de nouveau la nécessité de mettre en oeuvre des dispositifs de gestion de crise adaptés aux différents types d'élevage, sauf à vouloir les faire disparaître, ce qui n'est pas ce qui n'est dans l'intérêt de personne, les élevages extensifs autarcique, ce qui autarcique, souvent à l'agroforesterie et sur des débouchés de circuits courts ne peuvent être réglementairement traité comme les élevages à forte densité, aucune étude scientifique n'a démontré à ce jour que ces élevages sont générateur ou vecteur de l'influenza aviaire il y va aussi de l'image de nos territoires, comme c'est le cas dans le Gers et je ne veux pas que là aussi des drames sociaux face la chronique des faits divers, je n'ai que trop rencontrer Monsieur le Ministre, des éleveurs et des éleveurs et des éleveuse au bord des larmes et je n'exagère pas, parce que le Varenne, de l'eau est restée inaboutie sur la question de la ressource et de ses usages certains un appel à un plan Marshall de l'eau pour l'agriculture, la question, on le sait, se pose pour tous les usages, et dans un cadre de dérèglement climatique qui complexifie la gestion, cette question n'avancera que dans le cas de d'un partage, et d'une co-construction démocratique à échelle territoriale adéquate envisagez-vous, Monsieur le Ministre, de généraliser sur la base des recommandations j'ai récente du Conseil général à à l'agriculture, les péter GE combien dans ce budget 2023, comptez-vous consacré au soutien des investissements nécessaires aux opérations de curage des retenues existantes dans la restauration, de capacité de stockage initial permettrait de régler de nombreux problèmes d'irrigation envisagez-vous des simplifications réglementaires ou un acte législatif spécifique pour avancer sans attendre pour ce qui est de la nouvelle PAC dont les crédits sont eux aussi en baisse à euros constants, comment la mise en oeuvre du PSN va-t-elle permettre et territoires éparpillés, territoire de compenser cette perte financière financière hélas à se répéter au-delà de 2023 le développement plus avant de l'agro-écologie devrait être au coeur de la loi d'orientation agricole annoncé Les Échos Chem du PSN devrait permettre de payer aux agriculteurs, notamment les externalités positives de leur travail, il y a-t-il dans ce budget au, delà de système très spécifiques à certaines pratiques ou milieu une volonté de mise en oeuvre de PSE et enfin quel dispositif envisagez-vous pour soutenir avant qu'elle ne disparaisse, je le crains, l'agriculture de polyculture élevage seule possible sur des terroirs difficiles, défavorisés, la dernière révision de la carte des ICHN je suis bien placé dans le Gers pour le dire, nous laisse très dubitatif à cet égard et la notion de zone intermédiaire reste à définir, réglementairement et géographiquement le modèle de la montagne a fait ses preuves pour le pastoralisme, d'autres régions difficiles méritent une égale attention je vous remercie. merci, cher collègue, la parole est maintenant à notre collègue Fabien Gay pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. C'est

crise de l'approvisionnement en entrant pour les agriculteurs et agricultrices, la peine est triple : de la production à la distribution en passant par le stockage, c'est tout un secteur clé de l'économie française qui est pris en étau, avec une hausse des coûts de production de plus de 26 % en un an, la filière agroalimentaire française est aujourd'hui au pied du mur sans autre perspective que celle d'un dépôt de bilan pour de nombreux agriculteurs ou d'une répercussion des coûts sur les consommateurs. Je dis bien pour seule perspective parce qu'aucune exploitation ne pas absorber des factures d'énergie à plus 400 % quand dans le même temps, les volumes de ventes sont en baisse pour les communes et les départements, l'inflation subie par nos agriculteurs se répercute directement sur la commande publique cantines scolaires CCAS Epad : la hausse des prix des denrées alimentaires, est aussi un poids pour les finances locales, pourtant déjà contrainte ensuite pour les consommateurs, les consommatrices pour qui le pouvoir d'achat s'effondre sans que les salaires augmentent l'inflation alimentaire plus 12 % un an ne laisse pas d'autre choix pour beaucoup que celui de la privation ou du report sous une qualité moindre, et les premières concessions les premiers produits auxquels nos concitoyens école citoyenne renonce, ce sont les produits issus de l'alimentation locale et des circuits courts, ce sont donc des ventes en moins pour notre agriculture locale pourtant déjà en grande difficulté, monsieur le Ministre, d'un bout à l'autre de la chaîne de production alimentaire, vous le savez, la situation est grave, elle est avant tout pour nos agriculteurs agricultrices, dont beaucoup sont toujours exclus du bouclier tarifaire et du guichet d'aide quant à l'amortisseur d'électricité prévue pour 2023, nous parlons d'une compensation de 25 % de la facture d'énergie, mais 25 % d'une facture qui prend 400 % en un an, c'est une facture toujours insoutenable et je reprendrai d'ailleurs ici les mots très juste de mes collègues rapporteurs la mission Agriculture c'est tout l'impensé de ce budget agricole ce le ministre nous parlons du quotidien de centaines de milliers d'hommes et de femmes qui font vivre l'économie la plus créatrice d'emplois et de valeurs ajoutées dans le pays pour elle et eux, l'urgence est là et elle également pour les générations de demain, une agriculture national local qui dépose le bilan, c'est une catastrophe sociale, mais aussi écologique et climatique après plus d'un an de hausse des prix des intrants et de l'énergie, il est plus que jamais temps de soutenir tout notre tissu agricole pourtant en lieu et place de cela, la présidence française de l'Union européenne a servi cette même année à entériner un nouvel accord de libre-échange conclu avec la Nouvelle-Zélande et le Parlement national ne sera même pas consulté, c'est insupportable dans la période à nos agriculteurs qui se demandent si leur exploitation tiendra une année de plus, vous avez envoyé le message suivant des produits venus de Nouvelle-Zélande opère des produits interdits, rappelons-le, dans l'Union européenne viendront parcourir 20000 kilomètres pour concurrencer l'agriculture locale dans nos assiettes, peu importe la conjoncture, peu importe la crise écologique, peu importe les conséquences sur nos filières agricoles ce modèle économique ravageurs poursuit ses passages en force jusqu'à s'extraire du contrôle du Parlement, j'en profite d'ailleurs Monsieur le Ministre pour vous redire qu'une résolution a été adoptée à l'unanimité pour que le CETA soit inscrit à l'Ordre du jour du Sénat et que nous n'avons toujours aucune réponse concrète ni de votre part, ni d'aucun autre membre du gouvernement, pourquoi est-ce que vous avez peur du débat, pourtant il y a le débat sur le modèle alimentaire vers lequel la France s'engage sur cette course au traité et sur leur empreinte écologique, ce débat est nécessaire, car nous n'avons plus le temps m'attendre chaque cataclysme qui climatiques que nous vivons est une preuve supplémentaire qui interrogent nos choix économiques, il y a quelques mois encore, nous vivions un été caniculaire d'une ampleur sans précédent, les sécheresses, les pénuries d'eau, les incendies qui ont ravagé le ouest de la France sont hein, Sylvianne au total c'est une surface de forêts 6 fois supérieur à la moyenne décennale qui a péri dans les flammes, c'est un sinistre record qui doit être considérée avec sérieux, en renforçant les moyens de l'Office national des forêts, et c'est tout l'inverse de ce que propose ce projet de loi des finances qui poursuit l'assaut sur les effectifs de l'ONF, avec cette année encore 80 suppressions d'emplois et c'est donc pour toutes ces raisons, pour faire plaisir à mon collègue Bernard buis en grande responsabilité que nous voterons contre les crédits de cette mission, je vous remercie. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Ce projet de loi de finances sur la mission Agriculture et l'objet d'un certain nombre d'interrogations, et pourtant c'est un budget qui apporte un certain nombre de réponses positives, l'assurance récolte dont on parlait depuis un certain nombre d'années, est enfin mise en oeuvre, les clés de répartition sur leur financement est clairement établies dans la loi, parti agriculteur partie compagnies d'assurance parti État. Simplement, aujourd'hui, certains ne sont pas d'accord sur les 560 millions d'euros inscrits au projet de loi de finances, tout simplement parce que ça ne serait pas suffisant alors que, honnêtement, aujourd'hui, personne n'est capable de dire combien d'agriculteurs souscriront cette assurance et combien cela coûtera à l'État et je voudrais avoir en preuve au cours des 2 dernières années, pour le gel de l'année dernière et pour la sécheresse de cette année et pour la grippe aviaire, le gouvernement a su répondre favorablement aux demandes que qu'il n'était pas supportable par l'agriculture, seul, alors pourquoi le gouvernement et c'était l'engagement du ministre de l'agriculture ne sera pas augmenté ses 560 millions est nécessaire, alors qu'il ne serait pas prudent de bloquer 100 ou 120 millions de plus aux dépens de certains nombres d'opération. Le TO-DE est inscrit au budget de ce ministère alors que précédemment il était ailleurs, sans garantie de durabilité, je crois que cette inscription nous donne l'espoir qu'il soit maintenu définitivement l'agriculteur, l'agriculture saisonnières notamment, qui en a grand besoin. Par contre, c'est vrai, il y a un certain nombre de points qui sont insuffisants et je voterai favorablement pour un certain nombre d'amendements, c'est vrai qu'il est pas normal que le casse d'art soit amputée de 10 ou 15 millions d'euros tous les ans, alors que c'est une recette qui vient de l'agriculture et que Bercy aime toujours se mettre 10 ou 15 % sous le coude et les récupérer sans rien dire. Il y a également des points positifs à travers la transition agroécologique je crois que les crédits de recherche, notamment sur la vaccination pour éviter notamment les crises sanitaires influenza aviaire notamment de perdurer, je crois qu'il serait mieux de mettre davantage dans la recherche sur les vaccins, plutôt que de payer cette année pratiquement un milliard d'euros pour payer les pertes. De même, il est positif d'avoir soutenu les 5 millions d'euros à l'agriculture biologique alors que ils étaient financés l'année dernière à travers le plan de relance, c'est également un point positif. Par contre l'absence de bouclier tarifaire, notamment pour les engrais n'est pas normal, les agriculteurs se sentent plutôt rassuré aujourd'hui pour ce qui est les carburants par contre pour les engrais, c'est une vraie difficulté, et tant qu'on aura la chance, la chance ou la malchance pour les consommateurs d'avoir des cours mondiaux qui feront favorable l'agriculture pourra tenir le choc, par contre, imaginons, et ça n'est peut-être pas très loin, que des récoltes mondiales, notamment venant de la Russie. Envahissent le marché du monde, hé bien, dans ce cas-là, on aura un effondrement des prix agricoles, avec une agriculture qui se font entrera en même temps. 5 millions de plans de relance pour le Dieu bio, je l'ai dit il faudra pérenniser, il ne faut pas pousser plus en avant une agriculture bio qui ne trouve pas ses consommateurs, mais il faut maintenir cette cette production agricole qui a une certaine légalité. Catherine Noizier parlera du bois énergie tout à l'heure, maintenant je vous direz, monsieur le président, que je compte beaucoup sur la la loi d'orientation et de son financement sur la transmission formation installation sur la recherche développement, sur la modernisation et sur la redynamisation des productions qui ont perdu leur compétitivité. Merci, cher collègue. La parole est donc maintenant à Henri Cabanel pour le RDSE.

Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Quelle agriculture voulons-nous et quels moyens, sommes-nous prêts à lui accorder depuis que je suis là, cet hémicycle j'essaie inlassablement de sensibiliser aux enjeux du secteur agricole et de la méthode à adopter ensemble pour une efficience et des résultats des enjeux externes de santé publique d'indépendance alimentaire d'adaptation au réchauffement climatique, de préservation de l'environnement et de la ressource anneaux d'emplois non délocalisables de préservation du foncier, de recherche et d'innovation des enjeux internes de revenu d'emploi rémunérateur de bien-être, de transmission avec une méthode que nous n'appliquons pas suffisamment une évaluation des impacts de nos décisions, car les chiffres cynique signifie peu au regard des enjeux, ce budget par exemple angoisse de 15 % mais les membres des différentes commissions ont quasi unanimement indiqué qu'il n'était pas à la hauteur des questions se posent quelle vision du bien-être de nos agriculteurs, avant de nous quand ouvriront nous le chantier du prix rémunérateurs et du revenu au, delà de Ghalib hein et de quelles actions pour favoriser la transmission des exploitations, quelle image positive pour nous offrir aux jeunes : quid de la loi foncière depuis des années, je propose des moyens supplémentaires aux affaires via les établissements plus foncier pour qu'elles assument pleinement leur rôle dans l'installation et le portage foncier et hein, et ce en toute transparence concernant la prédation du loup 11 pays européens se sont réunis hier à l'innovation du cercle 12 pour demander une régulation quelle posture avez-vous Monsieur le Ministre, face à la demande une une évolution des accords de Berne quelles mesure de simplification : Pouvons-nous encore initié comment dans un contexte de concurrence exacerbée d'enjeux climatiques que pouvez-vous plafonner le budget destiné à la recherche, rien que pour l'année 2022 la prévision des recettes de la taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles qui alimente le casse d'art se re-situer entre 143 et 148 millions d'euros et l'eau, alors qu'elle se raréfient, il faudrait anticiper par les vrais le partage de cette ressource est fondamental et ses usages, doivent être raisonné la piste de la réutilisation des eaux d'assainissement, par exemple, doit être véritablement étudié comme nous l'a montré, d'ailleurs, l'INRA et à Pech Rouge dans l'Aude, il faut simplifier les procédures, nous sommes retard sur ce sujet, concernant la gestion des risques, le dossier n'est pas nouveau, il aura fallu des millions d'euros dépensés après les épisodes de gel de grêle de sécheresse, inondations pourra en faire répondre à la détresse des agriculteurs avec la mise en place d'un dispositif universel de couverture de risques, cependant, où en est-on de la moyenne olympique Monsieur le Ministre : quelles sont les avancées avec l'Europe puisqu'inopiné, la décision a ne dépend autant de questions et de réponses à apporter pour passer le bien-être nos agriculteurs 1 septembre 2019 la MSA a communiqué l'effroyable si suicide pour la seule année 2015 depuis silence radio sur les chiffres, car la grosse machine, c'est un fait, mise en route et c'est très bien, le film au nom de la terre d'Édouard Bergeon a mis des images et des prénoms sur l'innommable le débat là cet hémicycle pour égaliser oui examiner ma proposition de loi, le rapport de ma collègue Françoise Férat et moi-même, ainsi que celui du député Damaisin ont sorti de l'oubli des milliers de femmes et d'hommes qui a choisi de mettre fin à leur vie, nous avons collectivement porter leur voix et ouvert la voie. le plan de prévention du ma lettre a ainsi été annoncé à novembre 2021 un coordinateur monsieur Daniel Lenoir a été nommé avec ma collègue Françoise Férat, nous l'avons longue a rencontré hier il nous a assuré sur votre volonté d'avancer sa mission s'achève en février 2023 et après Monsieur le Ministre, il est absolument nécessaire de prévoir une évaluation, de mesures commun aider un délégué interministériel une mission ministérielle ou un groupement d'intérêt public qui aurait l'Avantage de réunir tous les acteurs autour de la table, je pense aussi aux associations comme Solidarité paysans ou comme demain pour demain, qui oeuvre au quotidien pour aider les agriculteurs en difficulté ou des familles endeuillées, quels moyens à leur apporte le main je regrette, comme tous les rapporteurs une confusion ne ce budget concernant les sommes dédiées à ces mesures. Tout comme j'aurais souhaité un document unique qui détaille les financements par actions, comme par exemple la réa dans le budget prévu est à la baisse, il s'agit pourtant d'un dispositif d'aide à la relance d'exploitations en difficulté mais, et c'est le mal français, il est trop méconnue et complexe, pourrait être utilisé, malgré cela, Monsieur le Ministre, mon groupe RDSE ne votera pas contre ce budget Amos, même s'il n'est pas à la hauteur des enjeux, il s'abstiendra, très symboliquement, j'ai déposé à la main de qui reprend la première proposition de notre rapport CAN 2023 l'agriculture devienne une cause nationale, les paysans nous nourrissent leur dédier une année d'action serait à la hauteur de leurs missions et de nos ambitions. Je vous remercie, merci, cher collègue. Et la parole est maintenant à Daniel Gremillet pour les républicains. Monsieur Monsieur le président, Monsieur le Ministre Madame messieurs les rapporteurs, madame la présidente, chers collègues. Effectivement, c'est un budget qui va rentrer dans l'histoire, Monsieur le Ministre, ça fait pratiquement 60 ans. Que un pacte avait été passé entre les agriculteurs français. Et la nation Et la nation avec les différents gouvernements qui se sont succédé sur la création du fonds des calamités. Si en 1964 ce fonds a été créé, c'était pas pour faire plaisir aux paysans. C'est parce qu'on avait compris, déjà à cette époque, pour que l'assiette sont remplies, l'État avait aussi sa propre responsabilité, pour permettre aux agriculteurs d'affronter les différents aléas. Mon propos n'est pas de remettre en cause, on souhaitait tous c'est très fort Monsieur le Ministre, mon propos à cet instant, au-delà du budget, c'est votre engagement. Votre engagement parce que, en soixante-quatre. Il n'y avait pas de choix c'était systématiquement assis sur les assurances, incendie des agriculteurs, donc tout le monde par définition contribuer du principe de un pour un. Aujourd'hui, on est parti sur le volontariat et l'enjeu, monsieur le Ministre, il est terrible parce qu'effectivement, personne ne peut, à cet instant, notamment dans des productions très spécifique : l'élevage avec l'herbe et peut dire le nombre d'agriculteurs qui vont effectivement souscrire ces contrats d'assurance, la responsabilité est énorme, tant pour l'avenir des agriculteurs mettant aussi pour l'assiette des Français tant pour l'économie de notre pays que pour les entreprises agroalimentaires, on a du mal à le mesurer et je souhaiterais tout à l'heure dans vos réponses Monsieur le ministe qu'au-delà de l'assurantiel le gouvernement sans qu'un s'engage effectivement d'être aux côtés de l'agriculture pour garantir effectivement cette alimentation, temps nécessaire et permettre aux agriculteurs d'avoir des perspectives d'avenir. En 2ème sujet : Monsieur le Ministre, concerne. Les conséquences de la loi Egalim. Là encore mon propos n'est pas de de dire de faire un retour en arrière, mais ne vous alerter. Il ne reste pratiquement un an Monsieur le Ministre, nous avons 300000 exploitations agricoles qui vont devoir faire leur conseil stratégique pour pouvoir, dans un an, continuer d'acheter de pouvoir exister à travers des achats des produits phytopharmaceutiques sur les 300000 je pense que vous avez les chiffres comme moi, vous savez qu'on ait, avec un taux d'agriculteurs d'exploitation qui ont fait effectivement ce conseil stratégique très faible et qu'aujourd'hui je ne vois pas à travers ce budget, ça a été évoqué sur le casse d'art, on avait des moyens de de donner un souffle nouveau pour effectivement dans cette année qui qui reste à courir pour qu'au 31 décembre 2000 23 ans, soit en capacité de continuer, que la ferme France puisse continuer d'être performante, donc là ça fait partie des défilés, là aussi, Monsieur le Ministre, l'autre sujet concerne ce qui se passe aujourd'hui.

Quelques chiffres. Avant. La loi Egalim. La France était largement sur le je prends l'exemple du prix du lait, largement au-dessus de la moyenne de cours du lait payé aux paysans européens au jour d'aujourd'hui, monsieur le ministre, et vous le savez, on est pratiquement les derniers de la classe, il y a que 2 pays derrière nous et quand je prends le différentiel entre l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, on est entre 60 et 100 euros les de différence alors que nous avons les mêmes charges, là encore, Monsieur le Ministre, le problème de la compétitivité, le problème du revenu pour permettre aux éditeurs d'affronter cette situation très particulière et devant nous et nous n'avons pas de réponse à l'intérieur de ce projet de budget en dernier point Monsieur le Ministre, concerne la forêt vous avez effectivement c'est assez historique, là aussi, depuis un an on a jamais eu mis autant de moyens pour accompagner les agriculteurs accompagner les forestiers accompagner les communes, les territoires sur la reforme la reforestation sur la plantation. Mais vous le savez, monsieur le Ministre, planter un arbre n'apporte pas la certitude que cet arbre va pouvoir grandir pour planter un arbre, il nous faut ensuite des moyens humains, essentiellement pour l'accompagner et on sait aujourd'hui, Monsieur le Ministre, que nous avons un grand déficit aujourd'hui dans le secteur forestier d'accompagnement au niveau de ce secteur, quand je vois le travail qui a été réalisé au niveau de l'assise de des assises de la forêt et du bois, là aussi il y a une certaine déception, nous avions proposé que le TO-DE puisse être élargie aux forestiers qui en avait tant besoin, nous n'avons pas obtenu je terminerai mon propos en me disant : Monsieur le Ministre, où est l'ambition française de reconquête de l'indépendance alimentaire et de l'indépendance stratégique de notre forêt en France donc pour cette raison, nous allons voter contre ce budget 2023. Merci, cher collègue, la parole est maintenant à Franck Menonville pour les indépendants. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le monde agricole a connu une année 2022 particulièrement complexe, la volatilité des cours, la hausse des coûts de l'énergie, la hausse des prix des intrants des fourrages, la hausse des coûts de production et des charges et des conditions de climatiques difficiles mais également le retour de l'épidémie d'influenza aviaire dans un tel contexte le con le soutien de l'État est absolument essentielle pour surmonter la crise et adapter notre agriculture dans ce budget, donc les crédits de la mission Agriculture alimentation forêt et affaires rurales sont en hausse de 30 % cette année soit 900 millions d'euros induites notamment par le financement de l'assurance climatique pour sa première année de lancement le soutien public pour le financement de cette réforme, ça ça s'élève donc à 560 millions d'euros dans 255 millions d'euros sont portés par la mission fort, force est de constater, donc qu'il pourrait manquer 122 millions d'euros sur les 680 pourtant annoncé par le président de la République en septembre dernier, l'État doit absolument tenir ses engagements, pourriez-vous nous rassurer sur ce sujet, il en va de la crédibilité du dispositif et surtout au travers cette crédibilité, cette sécurisation l'adhésion des agriculteurs. Très attendu sur le terrain, donc, cette réforme doit permettre une diffusion beaucoup plus fort de l'assurance-récolte ainsi que des conditions d'indemnisation améliorée plus équitable et plus protectrice, nous devons maintenant faire en sorte que de nombreux agriculteurs donc s'inscrivent dans ce mouvement dans cette démarche, l'attractivité le l'offre assurantiel, il est essentiel, il faudra également avancer sur d'autres volets comme l'évolution des pratiques et des techniques agricoles, la recherche et l'innovation et une meilleure gestion de l'eau autre levier absolument essentiel en matière de gestion des risques en agriculture, c'est pour quoi je voudrais vous faire partager nos interrogations concernant les crédits dévolus au d'art et leur plafonnement à 126 millions d'euros, en effet, le Qatar finance l'accompagnement à la recherche du développement en agriculture, c'est un outil essentiel pour permettre aux aux exploitations agricoles d'innover pour répondre aux enjeux multiples que sont notamment l'adaptation l'atténuation du changement climatique au changement climatique, le renouvellement des générations, ces moyens doivent donc y être renforcée. je voudrais aussi ce soir évoquer notre élevage et nos éleveurs, les aléas climatiques, là les sécheresses Arese répétition la hausse des coûts de production comme, entre autres, l'énergie et les prix de la des aliments,

auquel je rajouterai la pression sociétale, la pénibilité du travail et l'agri-bashing tous ces phénomènes se traduisent par une décapitalisation du du cheptel français sans précédent, en effet, les effectifs de bovins viande décroise 3 % et ceux de des bovins lait de un virgule 5 pour 100 la fragilisation de la couverture vétérinaire, maillon essentiel des filières d'élevage vient encore ajouter sur nos territoires aux difficultés à ce titre, il me semble absolument nécessaire que le maintien des stages tutoré soit soutenu quelle initiative comptez prendre-vous prendre Monsieur le Ministre, sur ce sujet au travers, cela se joue bien évidemment la la la filière élevage en tant que telle, la compétitivité de l'élevage doit absolument être réarmer, elle doit être accompagnée par une car derrière l'élevage, c'est bien évidemment toute une filière de transformation qui ont qui en découle et notre souveraineté alimentaire, à ce titre, je voudrais saluer donc le travail qui est effectué par nos collègues sur le service de de remplacement et notamment la peine la pérennisation des crédits d'impôts et le relèvement de son taux, qui contribuent à l'amélioration et l'attractivité du métier aussi l'enseignement agricole est un autre levier important de la transition de notre agriculture soutenue dans ce budget, c'est indispensable pour répondre aux défis du renouvellement, notamment des générations enfin concernant l'ONF je veux saluer l'annulation donc des baisses qui étaient prévues, donc à hauteur de 80 ETP, même si vingt demeure encore à la charge de l'ONF et c'est pourquoi je soutiens pleinement les amendement des rapporteurs sur le financement de ces 20 ETP on est fait, nous avons ce besoin sur le, sur le terrain de de beaucoup et de plus de compétences et d'effectifs face aux défis immenses qui de du renouvellement Forestier dans nos territoires,

l'agriculture française est porteuse de nombreuses solutions pour relever le défi climatique du stockage du carbone du captage du carbone, assurer la souveraineté alimentaire et notre collectivité énergétique, je vous remercie. Merci et je passe maintenant la parole à Joël Labbé pour le groupe écologiste solidarité territoires.

notre agriculture, on l'a dit à plusieurs reprises déjà, se trouve au coeur de problématiques multiple est crucial pour notre avenir, l'augmentation des coûts de l'énergie et celui des matières premières, l'effondrement de la biodiversité et le dérèglement climatique. La faiblesse des revenus payé aux producteurs le mal-être agricole, on l'a évoqué également la montée de la précarité alimentaire au niveau de la société, la question du renouvellement des générations, autant de sujets de défi qui nécessite une politique ambitieuse pour accompagner la transition agricole et alimentaire vers plus de résilience vers aussi plus de justice sociale. Dans ce contexte de gouvernement propose un budget qui pour nous est insatisfaisant, il ne soutient pas suffisamment les systèmes vecteurs d'alternative d'innovation et de résilience en 1er lieu je voudrais parler ici de l'agriculture biologique. ça ne surprendra personne, qui est la grande oubliée de ce projet de loi de finances, la grande oubliée, une nouvelle fois, alors même qu'elle est porteuse de nombreuses solutions d'avenir. Entretien de la vie des sols, ce qui permet de limiter les consommations d'eau et d'un, et ce qui permet aussi de préserver la qualité de l'eau, la diversification des productions pour mieux faire face aux aléas. Elle provoque également une économie territorialisée moins sensible au contexte géopolitique. Ses atouts sont donc multiples, et c'est aussi sans compter sur les externalités positives que que génère ce mode de production à mettre en face des exerce des externalités négatives pas produite par une autre forme d'agriculture, il se trouve qu'à une étude a été publiée la semaine dernière. Concernant les coûts cachés des pesticides, hé bien la fourchette basse, c'est 370 millions d'euros. L'impact des pesticides sur la santé, sur l'environnement 370 millions d'euros, fourchette basse, je ne sais pas si vous avez ces chiffres, Monsieur le Ministre, vous pouvez me répondre tout à l'heure peut-être madame la présidente, je ne sais pas si vous avez ces chiffres, chers collègues, je ne sais pas si vous les avez c'est une étude franco-belge, dans le cas-là a participé le le professeur Philippe Barret, qui était intervenue à un colloque que j'avais organisé sur l'agroécologie, ce sont des scientifiques et qui mettent les chiffre sur la table, on en a besoin, il serait intéressant d'ailleurs d'organiser un débat de les inviter et pourquoi pas un débat contradictoire pour que, véritablement, on ait un débat sur ces sujets. c'est con ça semble ne semble toujours pas avoir été saisi par le gouvernement, la prolongation du crédit d'impôt HVE pour nous c'est une certification qui brouille le message aux consommateurs et n'apporte que peu de garanties environnementales. Au-delà de l'agriculture biologique, ce sont l'ensemble des solutions de transition agroécologique et paysanne qui sont insuffisamment soutenues par ce but Pour ce qui est de la grippe aviaire, les mesures de biosécurité sentent inadaptés et pénalise très fortement les systèmes plein air et les petits élevages pourtant ces modèles limite bien souvent les risques sanitaires via des densités et des déplacements d'animaux moindre, il devrait donc bénéficier de mesures et d'un accompagnement spécifique face à ces problématiques sur le volet alimentation alors que la précarité alimentaire augmente, nous regrettons le manque de soutien aux collectivités pour maintenir une restauration collective accessible à tous et qui atteignent aussi les objectifs de la loi Egalim en terme de qualité, des repas et de proportion de de produits bio, c'est la loi, je le rappelle et on est loin des 20 % de plus, il est essentiel pour nous d'aller vers une sécurité sociale de l'alimentation et dans un 1er temps peut être une allocation pour une alimentation durable construite en lien avec les usagers et les acteurs agricoles ainsi que ceux de la solidarité, enfin je voudrais moi aussi Abou aborder le sujet de la forêt, alors que les incendies ont révélé l'importance d'une politique cultivant la résilience de nos forêts, ce budget ne comporte pas d'augmentation des moyens de l'ONF, institution pourtant crucial pour notre pays, nous espérons que le gouvernement se décidera enfin à amorcer une hausse de ses effectifs. Alors, par rapport à ce budget, nous serions prêts à le voter si l'essentiel de notre de nos amendements étaient retenus, je vous remercie. Merci, cher collègue et et je vais maintenant passer la parole à Sébastien Pla pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Monsieur le président, madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, peut-on affirmer sérieusement que le budget agricole au progresse en 2023 si l'on intègre la prochaine programmation de la PAC ou le transfert du dispositif TODE est entré en vigueur du système d'assurance-récolte pour laquelle j'aimerais obtenir des réponses sur l'épineuse question de la moyenne olympique il serait appréciable de savoir si les démarches ont déjà été engagés auprès de l'Organisation mondiale du commerce afin de faire évoluer ce dispositif ça ne quoi cette belle idée d'assurance universelle sera voué à l'échec. Peut-on, en outre, espérer un renouvellement des générations, quand on sait qu'il manque encore 7000 agriculteurs par rapport chaque année pour compenser les départs à la retraite et que d'ici 10 ans, 20 % des Terres agricoles françaises risquent de disparaître, peut-on enfin croire que la forêt retrouve sa place centrale d'un autre modèle agro-écologique quand la progression des crédits destinés à la politique forestière et d'à peine 4 % et que l'ONF a perdu 40 % de ses effectifs en 20 ans Monsieur le Ministre, rarement l'ONF remettons des agents sur le terrain, pas dans les bureaux, ce ne sont pas 80 mais 478 postes que nous allons vous proposer de créer non pas un par département, mais eux n'un chaque unité territoriale mais à y regarder de plus près cette euros ça ne trompe l'oeil de 30 % des crédits de la mission Agriculture et de l'arbre qui cache la forêt d'un manque d'audace et d'ambition, au moment même où la ferme France et en 20 ans, nous sommes passés du second 5ème O-RAN des exportateurs mondiaux de production agricole Le monde de paysans est en grande souffrance, il ne se passe pas une semaine sans que je ne rencontre dans mon département céréalier préoccupé par l'impact de la sécheresse, le coût des intrants les difficultés à mobiliser la ressource eau ou un éleveur inquiet par le manque de vétérinaires et qui ne comprend pas que le PSN écarte les surfaces année Steve collective de la mise en oeuvre de l'éco-régime ou un pêcheur qui s'interrogent, de voir la ressource diminuer non pas par la surpêche mais par la pollution ou un vigneron qui prennent de plein fouet les aléas climatiques qui éprouvent des difficultés de recrutement et qui croule sous le poids des sur-transposition des règles et des normes, je pense en particulier au durcissement des critères de labellisation HVE sachant qu'plus de 30 pour 100 de nos exploitants pourraient perdent leur certification en 2030, du fait du durcissement du référentiel, ou encore des signes adressés négatif à ces exploitants qui exercent sous le Label Nature et Progrès, à qui l'État réclament aujourd'hui le remboursement de 4 années d'exonération fiscale alors qu'ils remplissent des cahiers des charges qui interdisent les OGM, l'utilisation des engrais chimiques et des pesticides et que penser, enfin de la valeur ajoutée créée par la ferme France quand les aides PAC deviennent pour bien des fermes, la majeure partie du revenu : est-il normal qu'un agriculteur sur scène n'est pas de revenus que des jeunes se désintéressent de plus en plus aux métiers agricoles et que les retraités vivant avec des pensions honteuse ou bien que la loi Egalim que que ce soit la une, ou la deux censé garantir une plus juste rémunération aussi décevante, alors même que la souveraineté alimentaire de la France est mise à mal et que la moitié de ce que nous mangeons est emporté le monde de paysans est aujourd'hui en première ligne face aux conflits géopolitiques touchant de plein fouet, touché de plein fouet par l'inflation incontrôlée du prix de l'énergie et des intrants, remettant en question la viabilité de leurs exploitations, déjà précaire face à ce terrible constat : comment voulez-vous infléchir la situation en employant les mêmes recettes, ce budget est en réalité un copié-collé des Budgets passés alors qu'un véritable plan Marshall agricoles permettrait d'inverser la tendance, je suppose que vous allez me répondre qu'une loi d'orientation pour l'agriculture est en cours de préparation, hé bien, c'est très bien, sachez que, ici, sur l'ensemble de ces bancs, nous sommes prêts à vous accompagner dans l'écriture de cette loi, mais comment pourrons-nous voter une loi de programmation agricole ambitieuse, une évolution conséquente des moyens d'âge, un contexte de dégradation des comptes publics, organisé par le désarmement fiscal de l'État, Monsieur le Ministre, je ne perçois rien de novateur dans ce budget, et tant que nous ne considère auront pas l'agriculture comme un secteur d'utilité publique et je dirais même plus vital nous ce rejet, incapables de répondre efficacement aux défis posés à la ferme France merci. Merci, cher collègue, et la parole est maintenant à Anne-Catherine Loisier pour le groupe Union centriste. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je me concentrerai sur le volet forestier et plus précisément sur les moyens humains mis au service d'une plus grande résilience de nos forêts, la stratégie d'adaptation, nous ferons changement climatique est aujourd'hui une urgence : si nous ne voulons pas revivre à l'avenir, ce que nous avons connu cet été en ce sens, je salue Monsieur le Ministre, les efforts du gouvernement en faveur des investissements en forêt et en soutien aux acteurs économiques de la filière je salue également la tenue des assises de la forêt Dubois qui ont mobilisé l'amont et l'aval au printemps dernier qui ont tracé des perspectives et se sont traduites par des enveloppes inédite prévues au plan France 2030 mais le paradoxe, Monsieur le Ministre, c'est que vous pensez que nous pourrons mieux protégés et renouveler nos massifs, plus vulnérables avec moins d'hommes et de femmes en forêt et c'est pourquoi l'ensemble des groupes politiques du Sénat vous demande de revenir sur ses positions concernant les ressources humaines en forêt, les agents de l'ONF, tout comme ceux du CNPF doivent être plus nombreux sur le terrain pour mailler le territoire pour identifier les peuplements dépérissant à traiter au plus vite les dessertes à ouvrir les accès au point d'eau aménagé avec les SDIS les nouveaux plans de gestion a élaboré pour les 900000 hectares de forêts publiques et les quelques millions d'hectares de forêts privées qui sont aujourd'hui sans documents de gestion j'durable pour planter un milliard d'arbres en 10 ans, comme nous y engage le président de la République, nous allons devoir quasiment doubler nos efforts, quel autre établissement public a connu une baisse de 40 % de ses effectifs en 15 ans alors même que ses missions d'intérêt général et que sa charge de travail augmentait, année après année, comment expliquez, monsieur le Ministre que l'ONF, piliers de la stratégie d'adaptation au changement climatique soit le seul des établissements publics, oeuvrant pour la préservation de l'environnement à rendre des emplois avec mes collègues rapporteurs de la mission de lutte contre les incendies et ceux de la commission des affaires économiques, nous vous demandons de stopper le programme de suppression des emplois inscrits au contrat ONF à 2020, 2025 et de revoir ce contrat dès le PLF 2023, nous vous demandons, a minima, compte tenu des contraintes budgétaires que chacun mesure ici de refinancer la totalité des 80 emplois supprimés en 2 villes, 23 et nous concédons de ne pas revenir sur les 190 ETP supprimés en 2021 et 2022, au-delà des 60 ETP fait chier sur la DFCI, il s'agit aussi, Monsieur le Ministre de refinancer des ETP pour l'adaptation des forêts, incluant le reboisement, il va de soi que nous devrons faire le point fin 2003 pour constater notre capacité ou non à relever les défis de l'adaptation de nos forêts avec les effectifs actuels, sachant que l'ONF connaît une double peine, à savoir une baisse des schémas d'emplois depuis un certain nombre d'années et des difficultés de recrutement liées aux nombreux départs à la retraite et aux tensions qui ont nui à l'attractivité de l'établissement, aussi, aujourd'hui, beaucoup d'unités territoriales ne sont pas au complet il conviendra d'être attentif à ce que ces postes soient pourvus au plus vite pour permettre à nos agences d'assumer leurs missions de terrain nous proposons en conséquence un abondement des crédits de l'ONF à hauteur de 1 mis en parallèle, nous proposons de créer 20 postes supplémentaires pour le CNPF et les 12 millions d'hectares de forêts privées, durement touchée par les incendies de ces derniers mois, je rappelle que 90 % des parcelles qui ont brûlé étaient des propriétés privées, avec seulement 350 ETP pour 3,3 millions de propriétaires, le CNPF n'est pas aujourd'hui en capacité d'assumer des missions renforcées d'animation de conseils et de contrôle des plans de gestion un amendement proposera donc un abondement de 1 virgule 3 millions pour le CNPF nous proposons ainsi, Monsieur le Ministre, d'ajuster les ressources attribuées aux 2 établissements publics pilier aménageur de la forêt française, à raison de 20 postes chacun 40 postes et de 4 millions d'euros pour être enfin en capacité de relever les défis de la DFCI et de la mise en gestion durable de l'ensemble de nos forêts, c'est nous le pensons, monsieur le ministre, un effort nécessaire et maîtrisé que vous soutiendrez pour un certain nombre de mes collègues centristes, c'est votre proposition qui conditionnera le vote final, je vous remercie.

Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. L'été 2022 s'est caractérisée comme l'année précédente, par une aggravation des feux de forêt et de végétation illustrant ce qui était encore, c'est qu'il y avait encore quelques sceptiques les conséquences dramatiques du réchauffement climatique sur l'intensification et l'extension du risque incendie on prend rapport enfin mission feu adoptée le 3 août 2022, par la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable et la commission des affaires économiques du Sénat, nous avons pu illustrer l'impérieuse nécessité de renforcer les moyens de lutte, certes, mais encore plus. Le niveau des actions de prévention son allocation de son allocution, le 28 octobre lors de la réception des acteurs engagés dans la campagne 2022 de lutte contre les feux de forêt, monsieur le président de la République à structure à structurer sa stratégie nouvelle face aux feux de forêt, en s'appuyant sur 3 piliers qui l'a nommé mieux contenir les incendies réussir à lutter plus efficacement et reboiser et gérer les forêts ses orientations s'inscrivent pleinement dans les indications de nos travaux et si nous pouvons saluer l'intention de prendre en considération les impacts des évolutions climatiques sur les risques qu'encourent les forêts, nous sommes déçus par la traduction budgétaire car, de fait, nous restons du côté de la déclaration d'intention nous convenons du besoin de renforcement et de multiplication des actions, le président de la République. On une cartographie des risques déjà existantes, les outils dessus le surveillance de météo France, déployés en région Sud-Est le rôle de vigie de l'ONF compétence que l'ONF exerce déjà l'application, la simplification des ALD l'inventaire des forêts, la modélisation de sa structuration, or l'ensemble de ces dispositions relèvent du bon sens, mais il n'y a aucune mesure nouvelle, ni du côté des dispositions ni insuffisamment du côté du budget : elles ne coûtent pour ainsi dire rien à l'État le PLF 2023 n'est pas le reflet des engagements de notre président, Monsieur le Ministre, le compte n'y est lorsqu'on parle des obligations légales de débroussaillement je m'inquiète même dans le temps, nous notre président de la République Anne appeler à la puissance publique pour se substituer aux propriétaires défaillants, craignant de devoir encore s'alourdir l'engagement des dépenses de nos communes, intercommunalités et département, même s'ils sont parfois soutenus par certaines régions qui se sentent concernés. C'est par exemple le cas de la région sud dont le budget annuel dédié aux actions de prévention s'élève à 5 millions d'euros abondé par du financement MCA vers nous avons n'ont pas répondu à la problématique du financement d'épitaphe DFCI qui sont les pierres angulaires sur lesquels se bâtit la stratégie de prévention, nous pourrions presque dire que ce sont nos collectivités territoriales qui se substitue à un état sinon défaillant pour le moins insuffisant. Le principe de la valeur du sauvé n'a. Pas été intégrés pire avec la refonte du FCTVA à financement constant, nous ferons 17 % de travaux en moins alors qu'il faudrait les démultiplier je rappelle pour mémoire que certaines forêts comme la forêt méditerranéenne ne sont pas productives et qu'il est illusoire de penser trouver là le financement de sa propre des femmes habilité quant à la mission devait de réussir à lutter plus efficace ma, il convient de souligner, comme l'appelle le rappelle l'Assemblée des départements de France, que le financement du SDIS repose essentiellement sur la fraction de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance. Mais que la forme contribution des départements ont buggé des SDIS et de 2 fois plus élevé que le montant de cette taxe pour armer les SDIS face aux conséquences des dérèglements climatiques, il semble donc indispensable d'en revoir son augmentation sans pour autant fragiliser la fraction au titre de la décentralisation de la fiscalité locale si le programme 161 incorpore effectivement l'annonce d'une ligne de 150 millions d'euros au titre du renforcement du Pacte capacitaire qui ne sont pas pour autant des crédits supplémentaires mais une fraction de la compensation de la CVAE l'inventaire réalisé par les préfets de zone ne manquera pas de souligner, entre autres, la disparité la vétusté et le sous-dimensionnement de nos moyens de lutte, il en va de même pour notre flotte aérienne dans le renouvellement annoncé à partir de 2000 trente-cinq qui ne fasse partie d'objet d'autorisations d'engagement au PLF 2023 aurait nécessité dans l'intervalle. Quelques dispositions compensatoires, enfin, dans la perspective de mieux gérer et reboiser les forêts nous convenons de la menace contribuent les feux et le dépérissement néanmoins les crédits de l'action vingt-six du programme 149 reste à niveau constant en termes d'autorisations d'engagement, nous pouvons parler de double contrainte lorsqu'on souhaite effectivement renforcer le rôle de vigie de l'ONF, tout en continuant de rationaliser à l'extrême son organigramme est-il nécessaire de vous alerter à nouveau sur l'importance des investissements à réaliser au bénéfice de l'entretien de la surveillance et des travaux sylvicoles nécessaires à la protection de la forêt sa régénération, ils sont d'enveloppements non, je vais en faire l'économie définitivement monsieur le Ministre, le compte n'y est pas, je regrette à nouveau que l'on passe à la forêt lorsqu'elle est en flammes, mais que l'on oublie de penser à elle pour éviter qu'elle ne bol.

Monsieur le président, Monsieur le Ministre, madame la présidente, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, au titre de la mission Agriculture alimentation forêt et affaires rurales, le gouvernement demande pour 2023, à l'ouverture de 3 4 84 milliards d'euros en crédits de paiement, soit 30 % de plus que l'enveloppe initiale pour l'exercice 2022, toutefois, une fois pris en compte l'ensemble du contexte de l'inflation et des changements de périmètre, la hausse n'est que de 9 % par rapport à 2022 cet écart entre l'affichage et la réalité du budget de la mission Agriculture pourrait prêter à sourire si le concernait pas un secteur primordial du budget de l'État, c'est pourquoi je soulignerai déjà qu'il ne s'agit pas d'un investissement massif en faveur de l'agriculture de demain, mais d'un budget à mi-parcours, au regard des enjeux actuels et futurs du monde agricole, le débat sur les crédits, agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales n'a pas pu avoir lieu à l'Assemblée nationale, cela a été rappelé en raison de l'activation de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, ça tenue ici au Sénat, pardon permet donc d'identifier comme ont déjà commencé à le faire, les différents rapporteurs, dont je salue le travail les manques, mais aussi les améliorations nécessaires au budget de cette mission, il faudra que le gouvernement en tienne compte, ce budget comporte une forte orientation en faveur de la du programme 149 Compétitivité et durabilité, de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, avec un soutien en faveur de la structuration des filières de la modernisation des exploitations et de la transition écologique, il s'agit là d'un enjeu d'enjeu structurant pour l'agriculture dans le cadre de la PAC 2023 2027 conformément aux objectifs du Pacte Vert pour l'Europe et cela a été rappelé par mail prédécesseurs mais s'il faut verdir la PAC, comme disent les technocrates de Bruxelles cet je ne doit pas faire oublier d'autres thématiques plus délaissée dans ce budget, ni occulter des engagements non respectés en ce sens, je déplore avec les rapporteurs le manquement important concernant les financements des objectifs de la loi d'orientation relative à l'assurance-récolte et aux outils de gestion des risques climatiques à l'agriculture, les carences du budget sur ce point sont éminemment regrettable et mettent en péril la réussite de cette réforme, de plus la crise énergétique touche pleinement l'agriculture et l'élevage et ses conséquences se font durement ressentir dans l'ensemble des filières pourtant rien ou si peu, a été préparée dans le budget de cette émission pour tenter d'atténuer les effets négatifs de l'augmentation des coûts de production agricole et agroalimentaire, or la crise actuelle, poursuit la déstabilisation de l'écosystème agricole déjà fragilisée par la crise sanitaire et les et les aléas climatiques exceptionnelles de l'été passé, il est nécessaire d'apporter l'aide nécessaire pour pérenniser et renforcer l'agriculture française et améliorer et améliorer celle-ci ne peut se faire sans un soutien renforcé aux agriculteurs en souffrance et en particulier au secteur de l'élevage, il connaît une période de crise que l'on ne peut passer sous silence, plus largement, le renouvellement des générations et la rémunération de l'activité agricole sont des anges qui auraient mérité plus attention il y a urgence à à agir dès ce budget, et c'est ce que proposent les différents amendements des rapporteurs pour améliorer le budget de cette mission je voudrais souligner que le compte d'affectation spéciale Développement agricole et rural, voit son enveloppe reconduite à 100 millions ça 26 millions d'euros, cela été rappelée aussi cela est dommageable, tant les besoins d'innovation sont forts étant les instituts les chameaux, les cultures et les autres bénéficiaires sont porteurs de projets, il est symptomatique de ce budget, qui ne prévoit qu'il ne prévoit pas l'accompagner plus l'innovation agricole dont la France a plus que jamais besoin pour terminer Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je voudrais que nous puissions affirmer ensemble que nous croyons qu'il ne peut y avoir de pays sans paysans dans la France de demain, je vous remercie.

Merci monsieur le président, monsieur le président, madame la présidente, messieurs les rapporteurs, mesdames et messieurs les sénateurs. Le Sénat examine donc ce soir, les crédits de la mission dans un contexte particulier qui a été rappelé par un certain nombre d'entre vous et inédit qui est celui du drame qui se joue en Ukraine et la guerre en Ukraine, qui a des conséquences assez lourdes, ça été rappelé sur notre agriculture et sur un certain nombre de d'autres sujets, en particulier l'inflation, le caractère stratégique de notre capacité à produire pour nous nourrir et fortifier plus encore et ce. Qu'il avait oublié ont découvert que l'alimentation pouvait devenir une arme et donc nous avons besoin d'y travailler, y compris en termes de souveraineté les conséquences quotidiennes de cette guerre pour notre secteur agricole et alimentaire sont patentes. Je vais vous le dire d'emblée sur ces sujets là nous sommes pleinement mobilisés pour soutenir les filières concernées, c'est de passer le cap, je pense au cap énergétique, les accompagner et faire en sorte qu'aucune difficulté ne reste sans réponse : la crise que nous traversons, doit nous appeler d'ailleurs collectivement à l'humidité, la souveraineté alimentaire agricole ne se décrétera pas, nous devons y travailler collectivement et pas à pas. Ce que vous avez décrit d'ailleurs pour un certain nombre d'entre vous d'une lente dégradation sur 15, 20 ou 30 ans, montre bien que c'est une oeuvre et si vous me permettez cette expression collective et que nous devons devant donc essayer collectivement de relever le défi de la souveraineté, à cet égard l'augmentation d'un milliard d'euros, des crédits de cette mission par rapport à l'est un signal pour ce 1er budget du quinquennat je voudrais d'emblée le préciser, en réponse à vos interventions, la réponse que nous apportons aux défis immenses que traverse notre secteur agricole ne se limite pas aux crédits de cette mission, tout d'abord parce que le ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire et l'un des rares ministères qui voit souvent ses moyens augmenter au cours de l'année, cela vient souvent se traduire le soutien de l'État aux femmes, des hommes qui nous nourrissent. Chaque fois qu'une crise les frappes et pour ne citer que quelques exemples, la crise qui a été lié au gel, la crise de la l'influenza aviaire, j'y reviendrai tout à l'heure, la crise porcine, la crise sur l'alimentation et autant d'éléments qui ont permis, je crois, d'essayer d'être en soutien des agriculteurs et qui continueront à se déployer, on le verra aussi d'ailleurs sur le sujet des calamités agricoles. Deuxièmement parce que nous sommes dans une période charnière et que notre action est globale, au-delà des crédits budgétaires que vous êtes appelés à examiner les aussi 26 milliards d'euros qui sont globalement louer pour cette année, si l'on compte la PAC, les exonérations fiscales qui ne sont pas examinés dans ce budget, les exonérations sociales et qui permet de regarder la complétude assez crédit il faut ajouter aussi les les crédits de France relance et les crédits de France 2030, qui sont des éléments évidemment important de structuration de nos filières et de notre agriculture, elle peut pas non plus se résumer à la seule question, la perte de compétitivité constatée depuis 90 à être ça fait écho d'ailleurs aux travaux qui ont été menées au Sénat récemment, même si pour moi, cette question est essentielle : il s'agit d'ailleurs de la raison pour laquelle nous avons d'ores et déjà réalisé des investissements massifs avec France relance et France 2030 pour plus de 4 milliards d'euros, ce que nous vivons est un changement de paradigme avec le réchauffement climatique comme accélérateur et perturbateur parfois des transitions et de l'urgence d'accompagner les fermes France dans toute leur diversité, pour les aider à sortir plus forte de cette 3ème révolution agricole et bâtir la souveraineté alimentaire et agricole de demain, en s'appuyant sur une méthode de planification, porté par la première ministre, comme vous le savez, cela passe d'abord, ça a été évoqué par plusieurs d'entre vous par là juste rémunère isolation des agriculteurs qui on est, pour moi la clé de voûte, avec le combat que nous menons collectivement pour l'application et le développement de la loi Egalim alors, j'entends les remarques qui ont été faites par un certain nombre d'entre vous. égal M2 était le produit d'une modification des hein, je crois que si nous n'avions pas égal de nous serions dans une situation catastrophique, en revanche, on a besoin de travailler sur un certain nombre de filières, je pense en particulier à la filière laitière sur lequel nous ne sommes pas au rendez-vous mais vous l'avez rappelé monsieur le rapporteur, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels je crois qu'avec elle Egalim et les agriculteurs et les organisations agricoles reconnaissent, nous avons pu progresser, on a un secteur particulier de risque qui est le secteur laitier sur lequel il nous faut travailler avec les 2 distributeurs avec les transformateurs pour faire ou en sorte que la rémunération soit un rendez-vous cela passe aussi par le principe de réciprocité d'normes actuelles avec la présidence française désormais qu'il est acté, il faut le mettre en oeuvre et le faire vivre au sein des différents accords internationaux pour conclure des accords internationaux qui permettent de développer des clause de réciprocité qui me mettent pas en concurrence déloyale, un certain nombre de nos productions, nos producteurs, je l'ai dit quand j'ai été auditionné par votre commission, la question de la souveraineté alimentaire, pour moi, c'est pas une question de repli sur soi ou d'autarcie, la question de la souveraineté alimentaire, c'est que les règles de concurrence soient plus équitable, mais ça n'est pas le la fermeture sur nos propres marchés parce que je rappelle que sur le lait, sur les céréales sur le port. évidemment, sur les vins et spiritueux, mais je ne veux pas résumer l'agriculture française à cela, nous sommes puissamment une puissance, une puissance exportatrice et donc il ne faut pas se priver de la capacité que nous avons le fer et par ailleurs dans un monde de dérèglement climatique, il me semble que plus que jamais nous avons besoin de sécuriser nos approvisionnements au niveau mondial et donc, de coopération et d'échanges plutôt que de fermeture sur nos frontières, je tiens à le rappeler, quand même, sans que c'est un un, un élément essentiel, évidemment la question de la rémunération, c'est un élément essentiel pour le renouvellement des générations, je n'évoque pas ce soir longuement parce qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais j'en ai parlé en commission, ça je lancerai dès la semaine prochaine la concertation sur le projet de loi d'orientation et d'avenir agricole un pacte et une loi qui permettra d'essayer d'éclairer le chemin sur un certain nombre de sujets divers et variés, avec un seul objectif : assurer le renouvellement des générations. Pour assurer la souveraineté de la ferme France cela passe aussi notre stratégie par la production de masse tout autant que par la montée en gamme selon les spécificités des filières et des productions car il ne faut pas opposer les de l'excellence, une marque et l'une des marques de fabrique de notre agriculture, y compris à l'extérieur de nos frontières, sa diversité fait sa richesse et sa compétitivité, cela passe aussi par produire plus, tout en produisant mieux et nous sommes engagés dans cette voie pour des pratiques plus résilientes en phase avec les attentes de la société en matière de bien-être et avec Londres, d'assurer au plus grand nombre de nos tu mens plus modestes l'accès à une alimentation de qualité, j'y reviendrai sans doute dans les amendements qui seront présentés et puis le dire aussi, il faut que l'on. Produits et ça a été dit par plusieurs d'entre vous, ce que les consommateurs réclament c'est pour ça qu'on a besoin de travailler sur les films de qualité, on a besoin de travailler aussi sur des productions qui ne sont pas sous ces signes là pour faire en sorte qu'on réponde aux besoins des consommateurs, c'est en particulier le cas on rencontre sur la volaille, pour ne citer que cet exemple, on voit bien que là on a une distorsion entre ce que nous produisons et ce qui est réellement consommé et donc on a besoin de travailler sur ces stratégiquement, filière par filière. Et les crédits de cette mission viennent enfin il en outre nous donner les moyens d'agir en ce sens avec l'entrée en vigueur de la réforme de l'assurance-récolte le TO-DE le maintien des financements dédiés à l'indemnité compensatoire de handicaps naturels, c'était quelque chose qui était très attendue par les zones défavorisées ou les zones à handicap, le soutien à l'enseignement agricole ou la feuille de route sur la forêt, j'ai présenté, pour ne parler que de la forêt, cette feuille de route, le 19 novembre dernier notre ambition pour la forêt se traduit concrètement dans ce budget dès ce budget avec la suspension de la réduction des emplois de l'Office national des forêts qui ait eu une réduction qui dure depuis 15 ans et et des moyens qui seront alloués et puis on a porté à 20 millions d'euros après les 10 millions d'euros supplémentaires votée à l'Assemblée nationale, des crédits qui seront allouées en supplément à l'Office national des forêts, les nombreux amendements déposés sur le sujet me permettront sans doute. De l'approfondir, j'ajoute que, il y a les crédits qu'on met pour l'ONF pour rétablir et stopper l'érosion des des effectifs et de les crédits qu'on met par ailleurs et c'était réclamé par les filières forestière sur France 2030 et dans d'autres dispositifs pour assurer le renouvellement forestier, les moyens humains, les moyens en investissement pour faire en sorte qu'on rompe avec ce qui avait été malheureusement acté il y a plus de 25 ans, c'est-à-dire la fin du Fonds forestier national. Je voudrais maintenant évoquer le soutien aux filières et aux exploitations agricoles, première éléments l'assurance-récolte élément structurant de ce budget afin de financer ce nouveau système assurantiel qui permettra de mieux protéger nos agriculteurs l'effort de l'État ne fait que, plus que doublé, alors j'ai bien d'autres. C'était votre interrogation, alors je vais essayer d'y répondre une une fois de plus, en espérant que je sois plus performatif ma capacité de vous convaincre le budget qui vous a été présenté un budget à 560 millions d'euros parce que les simulations qui ont été travaillé d'ailleurs avec la profession agricole dans la progressivité de la et la montée en puissance de l'outil de l'assurance-récolte fait qu'on est à 560 sur cette année 2023 puis une progression qui nous amène sur le triennal à 600 millions d'euros pour au enfin si jamais il y avait un débordement aller jusqu'à 680 millions d'euros, mais la vérité c'est que si nous allions plus vite dans le déploiement du dispositif, nous prolongerons les crédits, c'est l'engagement du gouvernement, c'est mon engagement, c'est l'engagement du 1er ministre du président de la République, il me semble que les engagements ont été suffisamment fort pour aller assez loin, les débats ont été suffisamment nourri d'ailleurs avec la profession pour que nous puissions porter sereinement la conviction que le budget répond à ce qui est la progression du budget d'assurance récolte et pas autre chose

par les pratiques par le matériel de notre agriculture aux enjeux du dérèglement climatique et puis enfin, c'est la question de l'accès à l'eau, on y reviendra peut-être tout à l'heure au travers des amendements qui sont portées, mais ces 3 piliers qui compte et c'est la combinaison de ces 3 piliers qui permettront à l'agriculture, d'être plus résilientes et pas autre chose, sinon nous serions défaut à la réalité qui est la nôtre, ce n'est pas l'assurance qui va régler tous les sujets de résilience et le sujet du dérèglement climatique, il nous faut par ailleurs nous adapter, même si l'assurance permet de résoudre à répondre à un certain nombre de choses permettrait de dire un mot d'ailleurs sur la question de la moyenne olympique personne ne découvre en tout cas je crois pas ce soir, que ce soit un débat qui soit long et que une personne n'a jamais pensé dans les débats de bonne foi que au 1er janvier 2023, nous aurions réglé cette question, c'est une question qui n'est pas une question européenne, c'est une question qui dépend des accords internationaux, des accords de Marrakech, nous y travaillons avec des collègues européens pour y répondre, pour essayer de faire en sorte que nous ayons une position commune dans ces accords, j'ajoute et je serais assez preneur qu'on nous arrivions à y travailler ensemble, il faut savoir le modèle que nous défendons. C'est-à-dire sortir de la moyenne olympique, c'est bien l'objectif que nous pouvons partager mais pour pour sortent pour aller à quelle moyenne et pour aller à quels objectif et il me semble que le travail que nous devons faire en terme de recherche et d'innovation et tout autant important pour faire en sorte que les que les des cultures soient plus résilientes à eau la la sélection variétale le travail qu'on peut faire sur les embêter et tout autant important que de simplement se battre sur la question de la moyenne olympique, il me semble que c'est plutôt là que nous trouverons les voies du succès que seulement en rénovant une moyenne olympique dont on ne sait pas à quoi on va la la confrontés au modèle alternatif, mais ça n'empêche pas que nous disons. évidemment dû travailler 2ème élément que je voulais évoquer le le sujet de la politique agricole commune, je ne serai pas long là-dessus parce que ça n'est pas l'objet principal, mais en tout cas, évidemment, c'est un élément important, je crois qu'on a pu sauvegarder le budget, on a pu aussi stratégique un plan stratégique national dans des délais qui. Permettent et qui sont compatibles avec la réalité des agriculteurs, c'est-à-dire qui leur permettent d'avoir les conditions dans lesquelles ils vont exercer leur profession suffisamment en avant je ne liste pas les hein, l'essentiel des choses, j'essaie de répondre sur la bio, où on a des crédits qui vont en augmentation sur la bio-je le dis, la question n'est pas d'avoir un choc d'offre la question, c'est d'avoir une chance de demandes et le sujet sur la bio en France comme ailleurs d'ailleurs, c'est un sujet de au-delà d'ailleurs de la question de l'inflation et du contexte particulier pour un certain nombre de nos concitoyens la la la croissance à de chiffre que nous avions connu depuis 5 ans ou depuis 10 ans, est une croissance qui, depuis 2020 était déjà réduite et donc on a besoin de travailler sur le la mobilisation des consommateurs pour faire en sorte que une consommation plus et important, parce que rien n'est pire que d'engager quelqu'un sur la voie du bio pour lui expliquer après qu'il va toujours avoir une rémunération je pense qui va être parfois inférieurs. Dans certains cas à ce qui est du lait conventionnel donc on plus plutôt que de de seulement s'opérer sur la route, la conversion bio, faire en sorte qu'il y ait pas des conversions, ça me paraît un élément essentiel, je rappelle en août que dans les 5 ans, et ça, c'est bien à mettre au à notre bilan collectif et pas seulement du gouvernement. On a doublé les surfaces en bio, ce qui fait que la France et la plus maire surfaces en bio et puis 2ème élément, dire que, évidemment, on a travaillé sur l'ICHN pour les zones de montagne, je le disais, et puis un point qui me paraît important, même si c'est pas un point budgétaire, on se voit, qu'on a besoin de travailler, ça fait écho à ce que a dit le sénateur du plomb sur les questions de. Tracasseries administratives et parfois la sur administration c'est le droit à l'erreur à l'intérieur de la PAC pour faire en sorte que nous viennent pas pénaliser des agriculteurs parce qu'ils auront oublié de cocher telle ou telle casse et nous sommes en train de travailler avec la profession pour mettre en oeuvre un droit à l'erreur qu'il soit effectif. Dans ces professions pour lesquels c'est assez compliqué, je ne reviens pas sur la prolongation du thé deux pour 3 ans, ça donne de la visibilité, c'est un point important, c'est un travail que nous faisons avec l'ensemble des filières, c'est un travail que nous ferons et que nous prolongerons aussi sur les questions du plan de souveraineté en fruits et légumes, puisque c'est un sujet qui est éminemment important pour leurs, pour leurs éléments stabilisation du TO-DE mais d'autres éléments sur lesquels nous devons travailler, je ne peux pas ne pas évoquer devant vous les crédits pour l'Outre-mer, les crédits du comité interministériel des Outre-Mer ont été maintenus tout comme l'aide européenne pour l'agriculture ultramarine le poser, il a faim gros tampon notamment aux enjeux de ne d'autonomie alimentaire j'en viens et, pour finir à la question de la sécurité sanitaire, ça a été évoqué plus 7 % d'augmentation des moyens par rapport à 2002 le évoquez 3 éléments possibles principaux : la mise en oeuvre de la loi santé animale pour poser les jalons d'une sécurité sanitaire, le renforcement de nos contrôles et la surveillance des dangers sanitaires l'influenza aviaire la peste porcine, la tuberculose, les salmonelles, la brucellose, la mise en place de la polyclinique en charge de la sécurité sanitaire dans mon ministère sera responsable, il s'agit d'une réponse forte aux préoccupations légitimes de nos qu'on situation de con, nos concitoyens à la suite d'un certain nombre de scandales samedi. Mais rappelons-le, nous sommes un pays qui en terme de sécurité sanitaire le plus haut degré d'exigence et qu'on vient comparé avec d'autres pays européens et même outre-Atlantique, faut arrêter de se vilipender là-dessus et dire que quand même, nous avons les deux alors il peut avoir à y avoir des des crises sanitaires, mais globalement, nous sommes un pays où la sécurité sanitaire pour nos concitoyens est assurée dans les plus les meilleures conditions, c'est quand même pas mal de le rappeler, il me semble que c'est un élément important. Nous reviendrons dans les amendements sur la question de de la restauration collective, comme je vois le montant va être bientôt terminé et dire qu'on avait quand même déployé un certain nombre de choses dans le plan France relance sur les investissements dans les collectivités, des projets alimentaires territoriaux, le tout pour 130 millions d'euros, et nous allons la circulaire du Premier ministre de de la première ministre du vingt-neuf dès septembre 2022 qui permettra d'aider tous les établissements à renégocier leurs contrats et a su ajuster au juste prix, ces négociations, il me semble que nous avons un travail à faire, nous avons aussi, je sais que nous sommes attendus sur la question du chèque alimentaire je ne saurais que trop partagé ce dit récemment le ministre de l'économie sur la question de la nécessité de travailler sur le chèque alimentaire, nous y reviendrons dans les amendements, il y a un 1er, dispositif qui a été fait avec le ministère des solidarités avec un fonds de 60 millions d'euros pour les personnes les plus défavorisées voudrais concluons simplement intervention en en disant et et vous, et je l'ai dit tout à l'heure que nous sommes évidemment travaille aussi sur la loi de préparation de l'avenir et de la loi, le Pacte d'avenir avec les agriculteurs et avec vous tous pour faire en sorte que nous puissions installer les agriculteurs, dire 2 éléments : le 1er. Sur la question du mal-être des agriculteurs, je ne veux pas laisser sans réponse, je ne crois pas qu'il y ait des d'amendements là-dessus, nous sommes particulièrement vigilants, la mission sera prolongée et donc nous continuerons à développer une mission au travers du mal-être agricole parce que c'est un élément essentiel, ce n'est pas ce que j'ai entendu d'ailleurs ce soir au Sénat, mais je pense qu'il faut que nous fassions collectivement attention aux mots qu'on emploie sur l'agriculture et sur les agriculteurs, beaucoup d'entre le vivent comme une violence et donc on a besoin de faire attention aux mots et on a besoin d'être auprès de, et c'est bien le sens. De la mission qui sera prolongée, je reviendrai sur les questions d'eau toute toute toute à l'heure et donc simplement sur la puisque ça fait écho à la à la sollicitation du sénateur Cabanel les crédits et les autorisations d'engagement sont stables, on a ajusté simplement les crédits de paiement à la réalité de la consommation et donc les, les, les autorisations d'engagement sont là et s'il y a besoin de crédits de paiement supplémentaires seront développés, mais on a plutôt ajuster à la réalité budgétaire, il me paraissait important de le dire madame la présidente, messieurs les rares. Porteur mesdames et messieurs les sénateurs, ce que je voulais vous dire, je sais que nous avons un certain nombre d'amendements qui nous permettront d'évoquer ou évoque un certain nombre de questions sur lesquelles je n'ai pas encore pu vous répond merci beaucoup. Merci, monsieur le Ministre. Donc nous allons maintenant attaquer les les la discussion des amendements, je vous rappelle que pour cette mission, le gouvernement, la conférence des présidents, pardon à fixer la durée maximum de la discussion discussion générale compris à quatre heures, ce qui veut dire que si nous n'avions pas terminé l'examen de cette mission à une celle-ci se poursuivrait samedi prochain. Nous allons procéder donc pour commencer à l'examen des amendements portant sur les crédits de la mission Agriculture alimentation forêt et affaires rurales figurant à l'état B. Avant d'entrer dans le détail des amendements, je veux dire que nous allons commencer. Par l'examen de 76 amendements en discussion commune. L'article 46 bis alinéa 2 de notre règlement prévoit une discussion commune en cas d'incompatibilité, or cette discussion commune est justement lié d'une part à des incompatibilités de fond, d'autre part, au fait que l'adoption cumulé de certains de ses amendements aurait pour effet de vider certaines actions des programmes de la mission. Alors au sein de cette discussion commune qui va donc être longue certains amendements ont été regroupés à la suite de la demande de priorité de la commission des finances. Cela permettra l'examen de 2 blocs thématiques cohérent l'un relatif à la restauration collective. D'une part, et l'autre au moyen de l'ONF, enfin, l'Office national des forêts, d'autre part, donc nous allons exposer les 76 amendements. Il y aura l'avis de la commission, la vie de du ministre. Puis, pour les explications de vote nous regrouperont les amendements. Autour des des 2 thématique que je viens d'évoquer plus quelques petites thématiques en plus de ses 2 principales voilà comment vont s'organiser les débats, donc nous entrons dans la présentation des 76 à mon

mode soit en mode ou sous contrat nourrit quand même plusieurs millions de personnes par jour, que ce soit dans les cantines scolaires, les hôpitaux, les EPHAD ou les administrations son rôle donc sociale n'est plus à démontrer, malheureusement, dans le contexte actuel d'inflation que nous connaissions et d'application des dispositions Egalim les Budgets alloués n'ont pas été réévalué depuis des années et sont désormais trop faible face aux enjeux auxquels les acteurs doivent faire face, selon les estimations de la filière restauration hors domicile, il manque déjà au 15 juin dernier 40 centimes d'Euro par assiette pour assurer des repas

rupture d'approvisionnement, échec d'appels d'offres, baisse des achats de produits bio, baisse des achats d'origine française au bénéfice souvent des produits étrangers, et de même que augmenter les prix payés pour porter l'effort sur les familles déjà fortement fragilisé s'avère impossible, je rappelle que le repas à la cantine et pour beaucoup d'enfants au demeurant le seul équilibré de la journée, un outre les règles de la commande publique ne permettent pas aux entreprises qui approvisionne ma restauration collective de récupérer de manière satisfaisante les évolutions de prix ne serait-ce qu'en raison de égal de du coût de l'énergie, du coup, le transport ou des matières premières cela a pour effet de détourner certains producteurs, transformateurs de la restauration collective au profit d'autres débouchés, il a donc un vrai risque de désengagement de cette filière, c'est au final la souveraineté de la filière française d'approvisionnement des restaurations active qui est en jeu, c'est pourquoi il est proposé de créer un programme spécifique dédié à la restauration collective avec une eau revalorisation navire en 40 centimes par repas, soit un budget complémentaire estimé quand même à 880 millions d'euros, après, pour des raisons de recevabilité financière, il y a les transferts entre les actions, vous avez compris et donc je demande naturellement au gouvernement de lever le gage. Ensuite l'amendement présenté par Nathalie Delattre la présidente Nathalie Delattre. C'est un amendement identique, il a été excellemment défendu par notre collègue François Bonhomme. Si l'amendement défendu par Daniel Gremillet. Oui, monsieur le président, Monsieur le Ministre, monsieur le rapporteur, c'est la même chose, il a été très bien présenté, je juge très juste un point, c'est vous alerter sur la situation aujourd'hui des appels d'offres infructueux, puisqu'on est passé à moins de 10 % on est pratiquement à un quart, on a 25 % des appels d'offres aujourd'hui qui sont infructueux, donc il y a eu une sensibilisation très forte dans le cadre du Salon des maires de la semaine dernière, je voulais pas en rajouter, plus le reste d'autres collègues, François l'a très bien dit. Amendements suivant Monsieur. C'est monsieur le président, Monsieur le Ministre, même amendement nous c'est vingt centimes, il a été excellent moment là aussi défendu, je rajoute et j'insiste sur un point. La cantine scolaire. Il l'a dit. Mais c'est souvent le seul repas équilibré dans la journée pour les enfants et, dans mon département, c'est encore plus vrai. Et aujourd'hui. Les cantines, notamment scolaires sont en train d'avoir un choix extrêmement contraint. Soit moins. Soit en réalité couper l'entrée ou le dessert. C'est ça la réalité qui est en train de se passer C'est pas que pour les cantines scolaires, mais particulièrement pour les cantines scolaires. Pour un certain nombre d'enfants, il en va aujourd'hui de leur alimentation seul repas équilibré, donc je pense que, puisqu'il y a des amendements de tous les groupes. On pourrait en adopter, hein, il faut regarder, lequel et je suis d'accord sur le ministre, il faudra que vous leviez le gage sur cette question. Merci amendement présenté par Joël Labbé. merci monsieur le président Monsieur 1000, chers collègues, un amendement dans le dans le même esprit, visant à atteint des objectifs de qualité des repas de la loi de la loi Egalim et faire en sorte qu'il y ait égalité des enfants devant la devant il est bon de rappeler que les 20 % l'objectif de 20 pour 100 de la loi Egalim 20 % de produits bio, actuellement on est à 6 % il y a beaucoup mieux à faire, au moment où les producteurs bio sont en recherche de débouchés et de débouchés locaux, je vous remercie.

pour Athènes nos nos objectifs légaux en matière d'approvisionnement de restauration collective, un produit alimentaire durable et de qualité les, les, les 2 textes qui qui nous sont auquel on, on doit se conformer, c'est la loi Egalim d'une part, et la loi climat et résilience, d'autre part, Merci ensuite le même amendement défendu par monsieur l'abbé. Le 800 46. Oui bien défendu, juste un petit complément, il s'agit de financer de la formation pour les agents, mener un travail de sensibilisation des des des convives d'achat de matériel également et la mise en place d'actions sur le gaspillage alimentaire et d'action territorial pour la construction de circuits courts merci.

il est important de mobiliser, donc la restauration publique comme cela a déjà été rappelé et par conséquent, cet amendement vise à étendre et à renforcer la prime pour les cantines afin de prolonger l'action engagée lors du plan de relance, ce sera la bonne manière, à nos yeux pour développer donc une alimentation saine et durable dans les cantines des petites communes et donc, l'objectif est aussi d'élargir l'assiette des bénéficiaires merci. Si le le le suivant Monsieur Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, cet amendement vise à prolonger l'action engagée dans le cadre du plan de relance en faveur du soutien d'investissement pour les cantines scolaires à hauteur de 100 millions d'euros pour valoriser les produits frais de locaux durable et de qualité, il s'inscrit dans la continuité des autres amendements déposés par le groupe mon groupe socialiste sur la nécessité d'apporter un soutien financier aux acteurs de la restauration collective pour atteindre les objectifs de produits durables et de qualité, inscrit dans la loi cette aide à l'investissement est en effet indispensable car pour cuisiner des produits frais, réduire le gaspillage ou supprimer les contenants en plastique par exemple, il est nécessaire d'avoir des équipements de transformation des espaces de stockage de fruits et légumes frais ou du matériel de cuisine et de conservation des aliments adaptés, or cette année, cet investissement coûteux peut être un frein, particulièrement pour les petites communes, 2 ans après le lancement, dans la mesure du plan de relance le bilan apparaît bien mitigé car seulement 15 % des communes ciblées, ils ont fait appel pour la restauration scolaire, par ailleurs, dans le contexte actuel d'inflation et d'augmentation du coût de l'approvisionnement des moyens alloués à la restauration collective semble aujourd'hui inadaptée, d'après l'Insee, entre août 2021 et 22 les coûts de production agricole ont explosé avec les répercussions que nous connaissons plus 23 7 % % de charges agricole, plus 29,6 pour les aliments pour animaux puissent 42 4 pour l'énergie ou encore plus 85 et demi pour les engrais cet amendement cherche à remédier en partie à cette situation en amplifiant la faible dynamique actuelle en l'élargissant aux grandes villes, aux départements et aux régions, aux hôpitaux, universités et pas ou autre encore prison c'est l'objet du présent amendement qui propose d'augmenter les crédits de 100 millions d'euros, merci monsieur le président.

qui serait initiée par le gouvernement pour que le curage des retenues existante, fasse l'objet d'un accompagnement des agriculteurs Amnesty seulement à hauteur de 125 de 250 millions d'euros et que la réglementation afférente à ces opérations de curage qui est assez complexe soit simplifiée pour gagner en rapidité de mise en oeuvre, parce que sur ce sujet également, comme d'autres, il faut aller vite. Merci monsieur ce temps Yonne pour le suivant. suivant. Le président, Monsieur le Ministre le présente amendement vise à créer un fonds dédié à la distillation des stocks accumulés de vin rouge, l'objectif est clair : éviter le gaspillage et de très nombreuses faillites, il est impératif que ce vin plutôt que d'être perdu soit distillait aujourd'hui près de 3 millions d'Actos sont sont aujourd'hui en cuve et les revenus de la profession s'effondre, entraînant des difficultés de trésorerie et des cours de vente de vin de vin en vrac en chute libre, la consommation de vin rouge a chuté en France ces dernières années, les mesures de rétorsion américaines, les effets de la crise Covid auxquels se rajoutent les conséquences de la crise ukrainienne, coût de l'énergie et et notamment l'inflation bouleverse la filière, il faut à tout prix assainir la situation envisager dès maintenant un fonds dédié à la distillation des stocks accumulés tout en incitant la profession à réorienter la production vers les vins rosés et blancs pour financer cette opération, il est proposé de prélever 240 millions d'euros sur le programme Compétitivité et durabilité, de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, il y a des des affecté à un fonds Didier à la distillation des stocks accumulés : le vin rouge. Merci, présidente de Latran. Merci monsieur le président, il s'agit là par cet amendement, de créer un fonds de compensation de 200 millions d'euros à destination des des entreprises vinicoles qui sont touchés par la crise, alors on le sait, il y a eu différentes crises, on a commencé par l'attaque ce train, puis la crise Covid avec les bars, les restaurants fermés les crises climatiques avec le gel, les grêle le stress hydrique, nous allons de crise en crise, simplement, effectivement, nous avons peu d'aide en en compensation l'attaque se trompe est aujourd'hui évalué à plus de 400 millions de de dommages et d'où la demande de de ce fonds de compensation de 200 millions parce que c'est une fuite en avant, il faut bien qu'à un moment donné on commence par traiter sur cette crise structurelle les problèmes un par un et c'est vrai que l'attaque je souhaiterais que le ministre-nous disent aussi s'il a des nouvelles de de ce de cet accord que l'on avait plus ou moins eu en 2021, je ne crois pas que je Joey Biden nous nous arrange les boulons, entre guillemets, comment va évoluer ce dossier de dommage collatéral aéronautique sur la filière viticole merci. Merci donc on continue, on entre maintenant dans la série d'amendements qui concerne les enjeux forestiers monsieur Guey, le 830. Alors si monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, c'est mon 5ème budget déjà 4. Quatre, Quatre, ministre de l'Agriculture et chaque année qu'on arrive sur l'ONF. Le ministre-nous dit, on peut faire mieux avec moins d'effectifs. Oui ça. Et je pense que nous sommes arrivés au bout. Et on l'a vu cet été. Depuis 20 ans, vous connaissez les chiffres. 4 1000 1, jambes une privatisation rampante. Parce que, entre les ceux sous statut de fonctionnaire et statut de droit privé, un non, on est à égalité un dialogue social, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça entre les syndicats et une direction qui a été très malmenée depuis des années. Et on voit malheureusement qu'avec le dérèglement climatique. Les enjeux sont nombreux et c'est pas ma collègue Anne-Catherine Loisier qui me dira la forêt c'est pas que Dubois il y a toute une gestion. Bien d'autres. Et donc il a besoin à un moment, d'hommes et de femmes qui sont sur le terrain et effectue ses missions. Et donc il faut absolument arrêter. La casse et nous, nous pensons, nous aurons plusieurs amendements le premier il est ambitieux se redonner 231 millions pour revenir aux effectifs de 99 et donc aux 4000 agents assermentés. Et nous pensons pas que ces 3 messieurs nous pensons en réalité que c'est ce qu'il faut aujourd'hui pour effectuer ces missions et on ne confond pas tout, moi je connais bien la forêt d'Aquitaine qui a malheureusement brûlé chez quel est le droit privé mais ça a brûlé partout.

Ces dernières années, donc nous nous le demandons et j'espère que cette année nous allons Richard nous mettent d'accord façon commune que nous redonner ont les moyens. à l'ONF de fonctionner avec des hommes et des femmes qui sont bien formés, d'ailleurs, le Centre de formation autour de Nancy, il aurait aussi beaucoup à en dire, je vous remercie. Merci le suivant Madame Cukierman. Oui, merci Monsieur le président, Monsieur le Ministre finalement en amendement de repli de l'amendement précédent présenté par mon collègue Fabien guerre j'oserais dire, sans vouloir le plagié que j'en suis à mon onzième budget et que, effectivement, cette question de la situation de l'ONF revient, année après année et force est de constater, et nous l'avons vu y compris ces 2 derniers jours avec des représentants de la, de l'ONF, de l'autre côté de l'autre côté de la rue que sa gestion devient de plus en plus préoccupante, elle devient de plus en plus préoccupante, notamment pour la raison suivante c'est que le contrat d'objectifs entre l'État et l'ONF et de plus en plus exigeants et mais de plus en plus en pression la gestion salariale et du personnel de l'ONF, avec des exigences liées au réchauffement climatique lié à la gestion de la forêt domaniale et de notre pays qui font qu'il devient impossible aujourd'hui de concilier l'un ni l'autre le bien-être au travail et de concilier une bonne gestion forestière, et d'ailleurs un un rapport de la mission de contrôle sénatoriale a été rendue ici même le 3 août 2002 2022. Qui me demandaient de revenir à minima sur la suppression des 475 postes et vous dans ce budget, vous consacrez la suppression de 80 postes supplémentaires à un moment donné, sans mauvais jeu de mots, il y a urgence parce que oui, la forêt brûle mais au-delà de la forêt, c'est finalement toute sa gestion, c'est aussi parce que. Les personnels de l'ONF on cette cette mission-là qui est fondamental, le rapport avec les élus, avec les différents organismes qui font que, au quotidien, ils sont, outre de bons gestionnaires et aménageurs des espaces forestiers aussi de bons conseillers auprès des élus, sur ce qu'il y a à faire ou ne pas faire les fragiliser, remettent en cause toute sa gestion de la forêt publique dans notre pays.

autant de de de budget mais en tout cas, effectivement ce sujet revient et revient sans cesse, année après année, on est quand même, enfin je veux dire faut faut se mettent peut être déchiffré derrière ces chiffres, il y a des femmes et des hommes, et ses 6000 postes en moins depuis la création de l'ONF 1000 postes en moins pas il y a pas si longtemps, comment on peut faire fonctionner un service public en enlevant comme ça, les hommes et les femmes qui le font vivre, c'est totalement impossible, donc, il faut d'abord revenir sur ce contrat d'objectifs, ce contrat d'objectifs qui je pense a qu'un seul objectif, c'est de casser le service public de la forêt, donc je pense qu'il faut très vite revenir sur cet aspect dans ce que vous proposez, on ne reviens même pas à je dirais une stagnation des effectifs puisqu'on en perd encore, donc ça c'est totalement inacceptable, donc nous à travers ces ces amendements et effectivement on en a plusieurs, et je pense que dans le débat, il faudra qu'on trouve, hein, un terrain d'entente, mais en tout cas à minima, il faut au moins 200 200 effectifs en plus pour cette année, ça me paraît totalement indispensable l'amendement que je présente, on en propose mis tout simplement pour revenir à l'État 2017 qui ne paraît pas totalement, totalement dingue et puis je voudrais quand même rappeler que ces hommes et ces femmes, ce sont des fonctionnaires et ce statut de fonctionnaire, il est particulièrement important, parce que la dérive qu'on a eues avec des contrats, des contrats courts, non, on a besoin de fonctionnaires, pourquoi, parce que c'est une garantie de l'indépendance et on fait de la gestion forestière, c'est-à-dire qu'à la fois il y a de la vente de bois qui est à la fois il y a de la gestion de la biodiversité qui à la fois il y a le lien avec les élus locaux directement sur leur territoire, on a besoin de cette indépendance et on a besoin ce statut de fonctionnaire, c'est c'est des postes de fonctionnaires dont on demande et dont on a besoin aujourd'hui, merci. nous assistons ébahis et ce depuis quelques années au démantèlement organisé de l'ONF, nous ne sommes pas sidéré, puisque chaque année, nous déposerons des amendements et nous sommes nombreux à le faire, les bouleversements liés au changement climatique sont sans précédent, la forêt est notre allié, plus que jamais nous n'aurons pas d'avenir sont nos forêts qui qui doivent rester vivantes qui contiennent des écosystèmes absolument indispensable le rôle de l'ONF dans la gestion durable de la forêt est essentiel : l'ONF gère 17 millions d'hectares de forêts publiques, 30 pour 100 de la surface nationale forestière en dépit de son importance stratégique, l'État se désengage progressivement de sa mission et se défausse en partie sur les communes forestières, en effet, comme le disait mon collègue, le conseil d'administration de l'ONF a adopté un nouveau contrat d'objectifs et de performance qui le lie à l'État pour la période 2021 et 2025 et ce qui se profile, c'est la suppression sur ces années là de 475 postes déjà depuis 2000 17000 postes ont été supprimés, c'est absolument incroyable et impossible dans la situation dans laquelle nous sommes, nous devons absolument faire face à des adaptations sans précédent et répondre aux urgences écologiques de la fièvre et économique de la filière bois d'un politique que nous devons mener doit être une politique à vision publique à long terme et consacrer les moyens nécessaires, donc par mon amendement qui n'est pas au même niveau puisque on je pense qu'on descend au fur et à mesure des amendements qui est de 50 millions d'euros, propose de mettre un coup d'arrêt à cette hémorragie de ressources humaines en abondant le budget de l'ONF pour permettre la sauvegarde des 475 emplois menacés d'ici le nouveau contrat d'objectifs et de performance mais également en octroyant les fonds nécessaires pour recréer 500 postes, soit 10 % des postes supprimés ces 20 dernières années. Merci, cher collègue Monsieur Cabanel. Merci monsieur le président, cet amendement vise à augmenter les moyens de l'Office de 28 millions d'euros, le schéma d'emplois de l'Office de ce contrat depuis 3 ans pour 2023, ce sera encore 82 TP qui seront supprimés cette tendance n'est pas la bonne face à l'élargissement des missions de l'ONF en attendant si les dotations prévues dans le cadre du PLF 2 2023 sont conformes aux engagements pris par l'État dans le cadre du contrat 2021 2025, l'extension des incendies à des territoires jusque là épargnées nécessite l'ajustement des moyens de l'ONF. Merci madame la trique, contrat. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, donc, à l'instar de nombreux collègues issus de nombreux bancs, cet amendement vise à apporter un soutien à l'ONF, mon collègue Sébastien Pla l'évoquer d'autres amendements propose de créer 478 postes afin de redonner des moyens humains à l'office pour mener à bien ses missions à l'heure du changement climatique à l'heure où les incendies touchent sont nombreux partout en France et à des endroits où nous n'avions pas l'habitude de les voir et à l'heure où la gestion durable de nos forêt devient impérative en 20 ans, l'ONF a perdu près de 38 % de ses effectifs, alors même que ses missions non seulement demeure mais sont renforcés du fait des conséquences du réchauffement climatique, pourtant le PLF prévoyait initialement la suppression de 80 postes, il a fallu la mobilisation des députés pour que le gouvernement renonce en partie à ce projet destructeur néanmoins le déficit de moyens humains au sein de l'ONF demeure, il apparaît urgent de renforcer ses effectifs, donc c'est l'objet de notre amendement de créer 478 postes, soit l'équivalent de la crise de la création d'un poste supplémentaire dans chaque service de l'ONF, nous avons aujourd'hui besoin de renforcer ce service public de la forêt si essentiel je vous me. Merci Monsieur Salmon. c'est, c'est le symbole de la forêt française, cette forêt qui est mise à mal par tous les aléas climatiques par les bouleversements ces 410000 420000 personnes qui vivent de la filière bois, mais la forêt, c'est bien d'autre chose, c'est tout un tas d'aménité c'est une une capacité à réguler le climat, on en a absolument besoin aujourd'hui autant pour le bois matière que pour toutes ces autres que je viens de de présenter. cet amendement propose 500 500 ETP, effectivement, c'est une base je pense une base très raisonnables, j'ai entendu 475 on est à quelques dizaines près, c'est parce qu'il y a 320 unités territoriales, on a des hommes qui souffrent, qui sont en sous-effectifs qui n'arrivent plus à faire leur mission correctement et donc 500 semble une bonne base pour repartir sur une vraie dynamique pour aider toutes ces ce personnel à faire son travail, un travail qui ne peut pas être fait par des contractuels, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, ce sont des fonctionnaires, et lorsque l'on doit, hé bien, à la fois servir un client mais aussi être garant de la pérennité de la forêt, être capable de sanctionner, hé bien il n'a que les fonctionnaires pour pouvoir le faire, donc voilà je je plaide vraiment en faveur de ces 500 emplois qui sont nécessaires. Merci madame Préville le suivant. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, donc c'est un amendement de repli par rapport à celui que j'ai défendu tout à l'heure, il s'agit d'enrayer les baisses d'effectifs, et donc je propose cet amendement à 22 millions d'euros pour l'ONF pour c'était stopper le l'hémorragie des 475 emplois menacés d'ici 2025.

face à cela, les crédits de gestion durable de la forêt de développement de la filière bois progresse de 3,11 % s'agissant des moyens Directs de l'ONF, ils augmentent de 9 millions de 1 autorisations d'engagement et de 8 8 millions d'euros en crédits de paiement si ce sont les bienvenues, mais je n'oublie pas la contraction du schéma d'emplois de l'ONF depuis les 3 ans aussi, cet amendement vise à augmenter de 15 millions d'euros, les moyens de l'office. Merci madame DeMarco. Merci le dérèglement climatique affaibli nos forêts qui sont de plus en plus confronté aussi aux attaques parasitaires, au risque d'incendie aux tempêtes ou ça serait-ce ce que nous avons subi de plus en plus en Gironde, les agents de l'ONF sont en première ligne pour surveiller et protéger la forêt et occuper des espaces naturels alerter des départs de feu et les combattre, conformément aux recommandations du rapport sénatorial, cet amendement vise à renforcer les effectifs de l'ONF et créer 200 postes. merci monsieur le président, en 2000 à près de 808000 actuellement chargé de gérer 11 millions d'hectares des forêts publiques françaises, le nouveau contrat d'objectifs de performance 2021 2025 prévoit la suppression de 475 postes supplémentaires alors que le gouvernement a promis le maintien des effectifs pour l'année 2023, dans ce contexte et à l'heure où les forêts françaises sont au coeur de multiples enjeux écologiques et économiques le présent amendement vise à louer et plus de moyens financiers à l'office, en recréant 200 postes et en créant un programme financement de l'Office national des forêts, l'entretien et la valorisation des milieux forestiers doivent être un pilier de la transition écologique, notamment dans les territoires ruraux, je vous remercie. Merci monsieur Cabanel vous. Oui, merci Monsieur le Président, c'est un amendement de repli par rapport au précédent qui propose donc une hausse de budget de à hauteur de 11 millions d'euros. Ensuite, 2 amendements identiques, le 1er présenté par Monsieur du plomb. Madame Serra, monsieur le président, bon, cet amendement vise à mettre le gouvernement face à ses responsabilités en l'invitant à assumer le financement de l'annulation du schéma d'emplois de l'ONF, qui l'annonce effectif avec l'enveloppe de 10 millions d'euros ouverte dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité alors qu'elle n'est que partiel, si en effet 3 3 millions d'euros traduisent partiellement l'engagement du gouvernement de l'annulation du schéma d'emplois de moins quatre-vingts ETP de l'ONF en finançant 60 ETP seulement cela nous laisse pas moins 20 ETP à la chance de l'ONF aussi les rapporteurs pour avis, appelle le gouvernement conjointement avec monsieur Jean avec Madame Anne-Catherine Loisier monsieur Pascal Martin et monsieur Olivier Reitmans, rapporteur de la mission conjointe de contrôle sur la prévention des feux de forêt un ETP est estimé en moyenne à 65000 euros, ce qui nécessite un 1000000 d'euros de hausse financé via la subvention pour charges de service public, et Madame Ferrat, Madame Loisier. et donc également par nos, nos collègues de la commission des affaires économiques, moi je voudrais vraiment insister, Monsieur le Ministre, je crois que c'est l'investissement minimum nécessaire et maîtrisé pour en fait revenir sur les suppressions de postes qui était prévu au contrat ONF 2023 suppressions pour un montant global de 95 postes pour la contractualisation, financé par l'ONF et 80 postes qui sont absolument essentiels, vous en avez refinancer déjà 60 fléché sur la DFCI, c'est, c'est mais ce n'est pas suffisant et il faut absolument aussi que nous puissions compter sur davantage de postes disponible dans The ni nos unités territoriales monsieur le mythe, vous avez parlé tout à l'heure du plan France 2030, mais le plan ce 1er jour France 2030 pour le mettre en oeuvre, il va falloir des gens sur le terrain et il nous faut absolument dans une nos unités territoriales sur l'ensemble du territoire que nous préservions ces postes pour assurer ses missions absolument capital j'ajoute que nous le savons, l'ONF et comme beaucoup d'établissements confrontés à des difficultés de recrutement donc dans bon nombre de nos unités territoriales les effectifs n'y sont pas, donc si on rajoute cette difficulté de recrutement par rapport à des postes qui ne sont pas pourvus à ce jour, plus des suppressions de postes supplémentaires, autant vous dire que nous n'y y arriveront jamais, donc, vraiment, Monsieur le Ministre, le minimum que nous puissions faire c'est de revenir sur l'ensemble des suppressions qui était prévu en 2000 23 au contrat ONF étape.

de cet amendement pour être pour être cohérent, même si c'est quatre-vingts postes sont, on l'a dit, pas à la hauteur des des besoins. Merci donc voilà pour les amendements qui concernait l'ONF on continue avec la présentation de de tous les autres amendements, monsieur l'abbé. monsieur l'abbé. Le président monsieur mise sur collègue cet amendement vise à abonder les financements liés à la gestion des aléas afin de proposer des indemnisations aux producteurs exclus du système d'indemnisation actuelle et victime de la sécheresse en effet de nombreux agriculteurs restent en dehors, reste en dehors du système et sont insuffisamment soutenues par le nouveau système de gestion des risques et ne seront donc pas suffisamment, voire pas du tout soutenu face à l'impact des épisodes de sécheresse notamment les exploitations très diversifié, les maraîchers sur de petites surfaces ou des éleveurs ayant décapage capitaliser ou compenser la sécheresse par un fort accroissement de leur quantité de travail, nous souhaitons alerter sur la situation de ces producteurs et proposant donc une aide forfaitaire pour les accompagner, plus globalement, plus globalement, nous souhaitons attirer l'attention du gouvernement sur la nécessité de porter un système de gestion des risques équitable et efficace, capable d'accompagner l'ensemble des producteurs à l'image du projet de fonds mutuels et solidaire que nous avions défendu en février lors des débats sur la loi sur l'assurance-récolte. Merci et le suivant, c'est vous-même aussi, le 800 Le secteur de l'agriculture biologique fait aujourd'hui face à un ralentissement de la demande qui, dans un contexte d'augmentation de l'offre génère des difficultés conjoncturelles pourtant aucun budget permettant de déclencher les outils de gestion de crise n'a été mobilisé, la baisse de la demande à générer des mécanismes dits de réduction volontaire de la production, c'est notamment le cas dans la filière lait et dans la filière porc ce mécanisme de régulation des flux en période de crise ouvrent normalement droit à indemnisation encadrés par la réglementation européenne, ils sont régulièrement pratiqués lors de crises touchant des productions conventionnelles, mais malheureusement pour l'agriculture biologique, alors que les difficultés sont présentes depuis des mois, rien n'est fait pour aider les producteurs en Direct notre amendement propose donc de dégager une enveloppe pour la mobilisation d'outils de gestion de crise et d'aides financières pour les secteurs et exploitations biologiques en difficulté. Merci et et le suivant : 850. En un an, entre septembre 2021 et septembre 2022 le prix des engrais azotés a augmenté de 100 de plus, nous le savons, ces produits on a ont un impact majeur sur le réchauffement climatique et sur la pollution des eaux, il est donc aujourd'hui plus que nécessaire d'accompagner les agriculteurs pour se passer au plus vite de ces produits à la fois pour la résilience de notre agriculture, et pour la protection de notre environnement à l'initiative du Sénat la loi climat et résilience avait abouti à la création d'un plan azote ce plan n'est, malheureusement, à notre connaissance, toujours pas publié et n'est pas non plus financer cet amendement vise donc à lieu à lui alloué une somme de 71 millions d'euros les alternatives existent pour se passer de ces substances, notamment le travail sur la vie du sol, les engrais organique ou le développement des légumes, une des d'enclencher ce processus de transition. Merci et puis continuer sur votre lancée le 847. Cet amendement vise à soutenir davantage les projets alimentaires territoriaux, la question de souveraineté alimentaire et de résilience se pose de manière de plus en plus urgente, à nos sociétés dans ce contexte, il est urgent de reterritorialisation de relocaliser notre alimentation les projets alimentaires territoriaux sont des outils efficaces pour atteindre cet objectif, ils ont certes bénéficié de financement du plan de relance, mais il convient aujourd'hui d'accélérer encore leur déploiement les circuits courts et territorialisées sont également des outils pour construire des prix, des prix juste au producteur, les protégés de la concurrence déloyale des produits importés et ne respectant pas nos normes sanitaires, sociales et environnementales et répondre aussi aux attentes sociétales en terme de qualité de l'alimentation, ils sont également à même de participer à la construction de filières agro-écologique durable et résilientes l'ensemble de ces facteurs, appelle à la généralisation des projets alimentaires alimentaires territoriaux sur l'ensemble du territoire, nous proposons de de financer par cet amendement. Oui, monsieur le président, Monsieur le ministre et je voudrais profiter de cette prise de parole. Non pas que pour présenter cet amendement, mais surtout pour rappeler deux 3 choses la première pour répondre à Bernard buis tout à l'heure, il peut paraître cocasse de faire des amendements après avoir demandé de rejeter le budget, il n'a reste pas moins vrai Bernard que dans le même temps, nous savons pertinemment parce que ça a été le cas, et ça le sera sûrement cette fois-ci que nous sommes frappés du couvert du 49 3 ce qui veut dire que vu que le gouvernement ne va pas spécialement écoutez ce qu'on a à lui dire, il nous semble important, même si d'un côté nous rejetons les crédits que d'apporter des éléments qui puissent lui permettent d'avoir quelques éléments supplémentaires dans le cas où il viendrait la bonne idée de prendre des bonnes idées que nous pouvons lui donner, à l'intérieur du 49 3 c'est d'ailleurs pour ça que nous demanderons de voter certains amendements maintenant, monsieur le président de séance, il y a des choses que je ne comprends pas du tout, je ne vois pas comment ce mélange des amendements peut être véritablement retrouver à travers une certaine forme de logique, alors on me dit que ça vient des crédits, la façon dont les crédits sont imputés, ce qui voudrait dire que le premier qui sera adoptée, ferait tomber tous les autres, ce qu'il faut dire que je pense que ce soir on va voter des choses dans un brouillard total sans savoir exactement ce qu'il va se passer, parce que du moment où il y en a un qui va être votée si il fait tomber tous les autres qui sont sur la même ligne, ou le même ou les comment pouvoir organiser le vote, donc j'espère avoir quelques éléments là-dessus et en fin de seconde pour présenter mon amendement il Marest vingt-trois c'est 20 millions d'euros pour véritablement traiter la problématique de la de la recherche appliquée dans l'agroalimentaire, je pense que notre pays a besoin de se munir d'une mission de recherche pour l'agroalimentaire, qui n'est pas aujourd'hui à la hauteur des enjeux. Monsieur du plongée expliqué au départ, pourquoi le règlement nous conduisait à cette discussion commune mais quand nous allons passer aux explications de vote après les réponses. Des rapporteurs et du ministre nous procéderons par groupe thématique d'amendements, ce qui je pense rendra les choses plus plus clair en tout cas. C'est le règlement et je suis chargé de l'appliquer. Monsieur Tissot pour le 742. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, cet amendement pour but a pour objectif d'assurer le financement d'un plan interministériel de communication grand public, telle que souhaitée par la Cour des comptes dans son dernier rapport sur le soutien à l'agriculture biologique, nous proposons de consacrer 20 millions d'euros à cet effet, soit le montant annuel à louer à la campagne de communication des produits laitiers qui a prouvé son impact sur la consommation dans un contexte difficile pour la filière, il s'agit de renforcer les campagnes de promotion pour l'agriculture bio en donnant tous les moyens d'action à leurs acteurs, par ailleurs, nous tenons à rappeler que la Cour des comptes, encourage la création d'un poste de coordinateur ou déléguée interministériel permettant l'étude holistique des impacts et besoin pour le développement de l'agriculture biologique, nous souhaiterions, Monsieur le Ministre vous entendre à ce sujet, merci.

Il a défendu le le 820 monsieur Cabanel, ah non pardon c'était celui-là. C'était moi 841 pardon. Merci Henri alors que l'on constate un ralentissement de la demande en bio et une augmentation de l'offre, il est nécessaire de lui de lui allouer un budget, notamment via l'Agence Bio pour communiquer auprès des consommateurs, une enveloppe de 400000 euros avaient été débloqués au printemps, avec des effets très positifs qui avait contribué à stimuler la demande, malgré un montant faible, il faut donc réitérer l'expérience avec un budget plus conséquent, l'amendement propose 20 millions d'euros, nous nous sommes inspirés des montants de campagne pour la consommation de produits laitiers qui permettent plus d'efficacité, via notamment la possibilité de communiquer par la télévision aujourd'hui, l'État met des moyens sur la conversion en bio et fixe des objectifs d'accroissement des surfaces en parallèle de plus en plus de producteurs sont désireux d'adopter ce mode de production mais aujourd'hui sont découragés par le contexte, les politiques publiques se doivent d'être cohérente, il faut donc apporter un message clair aux consommateurs sur les atouts et l'intérêt des produits biologiques pour la santé et l'environnement. Merci le 820 monsieur Cabanel. Oui, merci Monsieur le Président, les agriculteurs sont de plus en plus engagé dans la transition écologique pour répondre à une demande sociétale dans son rapport publié en juin dernier sur le soutien à l'agriculture biologique, la Cour des comptes de préconiser, je cite, d'établir un plan interministériel de communication grand public sur les bénéfices de l'agriculture biologique en s'appuyant sur les évaluations scientifiques de son n'aime pas que sanitaire c'est l'objet de cet amendement qui prévoit une enveloppe de 20 millions d'euros pour ce plan de communication. pour objectif d'assurer le financement d'un plan interministériel de communication grand public, telle que souhaitée par la Cour des comptes dans son dernier rapport sur l'agriculture biologique, l'agriculture est en train de se transformer, nous devons accompagner cette transformation, l'agriculture biologique, l'agroforesterie la permaculture sont les solutions d'avenir, elles existent déjà, elles ont prouvé leur bons effets et, à vrai dire, nous n'avons pas le choix, l'espoir est là, l'espoir, comme le disait Verlaine lui comme un brin de paille dans l'étable et nous devons absolument convaincre nos concitoyens de d'avoir recours à l'agriculture biologique, d'une part mais d'autre part, nous devons aussi avoir les arguments pour leur faire adopter ces pratiques et, notamment, nous devons aussi rendre les choses accessible à tous nos concitoyens, c'est est absolument essentiel pour notre santé, juste au passage je je voudrais dire que les pesticides peuvent se retrouver dans nos corps jusque dans nos cheveux et je ne saurais que vous conseiller de faire des tests pour savoir quels sont les polluants que vous avez dans vos cours et qui ne sont pas évidemment des choses souhaitable parce que nos corps ne sont pas faits pour contenir ces produits chimiques. Monsieur Montaugé. parce que la problématique de l'accès à l'eau de son partage et de sa protection provoque trop souvent, on le sait, des incompréhensions, voire des crispations qui mène en réalité à déblocage définitif malgré les besoins divers avéré, donc nous proposons de consacrer au déploiement de ces pété, GE 20 millions d'euros, un autorisations d'engagement sur 2 ans et 10 millions d'euros en crédits de de paiement et et je rappelle, je l'évoquais à me direz hein discussion générale que le Conseil général à la grippe à l'agriculture vient de produire un rapport très intéressant de de assorti de préconisations qui vont dans ce sens du déploiement de péter Merci ensuite 2 amendements identiques, le 1er madame Préville. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, en septembre 2017, le gouvernement avait annoncé l'arrêt du financement par l'état de l'aide au maintien en agriculture biologique ainsi la ou les régions n'ont pas pris le relais, les agriculteurs bio n'ont plus accès à cette aide, ce qui pénalise fortement le développement de la filière, dans un contexte de la hausse du coût de la vie qui pénalisent la demande en produits bio et de baisse des prix payés aux producteurs dans certaines filières, comme le lait, le sous-financement du soutien au développement de cette agriculture et donc problématique puisque les services éco-écosystémique qu'elle génère, ne sont pas rémunérés à leur juste valeur cet amendement propose ainsi d'affecter 20 millions d'euros à un nouveau programme, aide au maintien en agriculture biologique destiné à rétablir le financement par l'état de l'aide au maintien.

la question des des aménité positive portée par l'agriculture bio biologique et l'ensemble des agricultures dites vertueuses les choses, monsieur le Ministre, madame la présidente, ont été chiffrés, alors j'ai parlé de 370 millions tout à l'heure, c'était la fourchette basse, la fourchette haute va plusieurs milliards alors aujourd'hui c'est pour ça que je vous interpeller, monsieur le Ministre, il va bien falloir mettre les chiffres sur la table et si en amont on va aider l'agriculture biologique qui n'a pas d'impact négatif sur le, sur la qualité de l'eau, par exemple, au contraire, elle préserve la qualité de l'eau, si ça c'est pris en compte, hé bien, à cette agriculture-là les prix des produits agricoles ne la différence n'est plus la même les les produits biologiques rattrape les produits conventionnels en étant de qualité et en jouant un rôle de préservation des déséquilibres environnementaux des pollinisateurs de la qualité de l'eau de la qualité de l'air de la qualité du sol de la santé humaine, merci. Merci l'amendement suivant Monsieur Merci monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, cet amendement est la manne d'appel qui vise à attirer l'attention du gouvernement sur la nécessité de relever le plafond des recettes du Qatar qui a, on le sait, un rôle central dans la recherche appliquée dans le domaine agricole, les, les prévisions de rendement de de cette taxe sont de lors de 140 millions d'euros, donc on est l'amendement que nous proposons vise à augmenter de 14 millions d'euros les moyens donc alloués à la recherche, par l'intermédiaire du Casa. Merci et le suivant Monsieur Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, cet amendement vise à élargir au cumin, le bénéfice du dispositif TODE il vient faire écho à l'amendement déposé par les membres de mon groupe et adopté dans le cadre du Plfss pour 2023 par le Sénat mais non retenu à l'Assemblée Nationale aujourd'hui, un agriculteur sur 2 états des du document avec 11510 en France et 23 moyenne c'est 240000 exploitants ces coopératives ont permis de développer diverses formes de mutualisation et ont été pionnière sur le développement des groupements d'employeurs dans la coopération agricole mais si employeurs ne peuvent pas appliquer l'exonération dédié à l'embauche de travailleurs saisonniers, or cette exonération TO-DE concerne et des tâches liées au cycle de la production animale et végétale ou aux actes de conditionnement des produits agricoles directement accomplie sous l'autorité d'un exploitant agricole, les Pumas sont dirigées par des exploitants agricoles aussi elle répondent à cette exigence, donc cette exclusion et donc d'autant plus contexte à tout contestable que les cubains sont les employeurs agricoles qu'elles embauchent des saisonniers et qu'elle constitue le prolongement de l'exploitation de leurs adhérents, elle est donc un obstacle au développement de l'emploi partagé en agriculture et constitue une rupture d'égalité avec les groupements d'employeurs associatifs en agriculture qui bénéficient

Oui, monsieur le président, Monsieur le Ministre, en juin 2022, la commission nationale paritaire présidée par le ministère de l'Agriculture a accepté une augmentation du point d'indice de 2,75 concernant les réseaux des chambres d'agriculture et donc l'augmentation de la du, du coût de la masse salariale, par définition, il faut que ces chambres et la capacité de pouvoir payer ce montant là qui correspond à 11 millions d'euros, il faut trouver la compensation parce que sinon ça veut dire que, par défaut, il faudrait le prendre sur la gestion courante des chambres qui veut dire que, par définition, elle le prendrait sur des actions qu'elle conduit pour les agriculteurs, donc soit soit il y a la possibilité d'augmenter la taxe, ce qui n'a pas été pris comme choix : soit il y a la possibilité d'augmenter la subvention de charges de service public ou la possibilité de donner une subvention exceptionnelle du montant de 11 millions donc c'est à vous de choisir Monsieur le Ministre, mais je pense que c'est un sujet qui est extrêmement important dans la discussion actuelle et pour l'avenir de l'activité des gens dans l'agriculture sur la totalité du pays et en particulier par rapport à la souveraineté alimentaire que nous souhaitons.

que j'évoquais ni hein discussion générale cet amendement donc vise à apporter un soutien spécifique à l'élevage extensif, il s'agit également de alliées un lien avec les l'INRA E et la des études scientifiques d'évaluations des externalités des élevages de type extensif au regard de leurs aime pas que sur la dimension économique, social, environnemental et culturel des territoires concernés cet amendement propose de consacrer pour cela 10 millions d'euros au financement d'un plan spécifique d'accompagnement qui reposerait notamment sur des études scientifiques démontrant les nombreuses qualités de ce type d'élevage et le leurs externalités positives nombreuses.

de développement agricole et rural, je comprends monsieur le ministre, il faut bien entendu comprendre pourquoi on observe une sous-consommation des crédits alors que les instituts techniques ont des projets à mettre en oeuvre, en attendant l'amendement vise à doter le compte, ça fait tache spéciale de 10 millions d'euros supplémentaires.

d'atteindre nos objectifs en matière d'agriculture biologique, et notamment celui de 18 % de la SAU d'ici 2000 27 au niveau français, avec en toile de fond celui atteint 25 %, sur le plan européen, il vise ainsi augmenter les moyens alloués à la recherche et à l'innovation en agri-bio le budget actuel n'est pas à la hauteur des enjeux et de plus n'est pas en adéquation avec la place occupée par le but aujourd'hui dans l'agriculture française le présent amendement propose de débloquer un budget de 5 millions permettant de financer 10 sujet de recherche à hauteur de 500000 euros pour 3 ans, un investissement qui soutiendra certains acteurs publics de recherche, comme l'institut de l'agriculture et l'alimentation biologique les étape qui gère actuellement coordination 60 projets, c'est l'objet du présent amendement. Et amendements suivants : Madame 13 villes. Si Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, cet amendement a pour objectif d'augmenter les moyens financiers et humains des acteurs de la crise de l'agriculture biologique par une mobilisation financière les interprofessions agricoles et la et par l'accroissement des subventions pour charges de service public, c'est une préconisation préconisations faites par la Cour des comptes dans son rapport de juin 2022 le présent amendement vise donc à permettre à l'Agence Bio d'atteindre ses objectifs en rehaussant son budget de 9 millions d'euros permettant de doubler son plafond ETP, 40 au total et de financer ses actions de communication et de soutien au développement territorial de l'agriculture biologique, je voudrais revenir très rapidement sur l'intervention de mon collègue Joël Habay tout à l'heure effectivement une des aménité positive par excellence de l'agriculture biologique, c'est la qualité de l'eau, les micro-polluants de l'eau, c'est un sujet qui émerge, qui est un impensé jusqu'à maintenant mais qui a surgi cet été à cause de la sécheresse puisque sécheresse implique concentration encore plus importante des micro-polluants de l'eau, nous devons nous y pencher et savoir que l'agriculture biologique permet de limiter l'arrivée des micros polluants dans l'eau, merci. Monsieur le Président, malgré une progression en France et des surfaces cultivées en bio, entre 2010 et 2021 sans aucune augmentation des moyens dédiés à cette politique, nous ne rempliront pas pas l'objectif fixé par l'Union européenne, hein, 2020 dans le cadre de son pacte vers la stratégie de la ferme à la fourchette, je le rappelle, il s'agit de consacrer 25 % des Terres agricoles à l'agriculture biologique d'ici à 2030, l'amendement se concentre sur le rôle de l'Agence Bio dans les moyens restent stables, nous souhaitons qu'il soit abondé de 9 millions d'euros, ce qui permettrait l'agence de doubler ses moyens humains actuellement réduit à

les pesticides sont partout, sont partout dans l'environnement, ils sont dans les soldes dans l'air dans les corps de tous les être vivants et tout ceci amène tout un tas de problématiques de santé problématique sanitaire avec des retards mentaux une érosion des capacités cognitives tout cela éprouvé et pourtant nous faisons comme si cela n'existait pas, c'est assez dramatique, et en ce moment, nous assistons à une perte de vitesse du développement de la bio alors que le gouvernement, du moins dans ses paroles dit qui veut placer l'écologie au coeur de sa feuille de route et la promotion de l'agriculture biologique doit donc être renforcée, c'est ce que nous défendons tous sur ces bancs, plutôt à gauche, ici, la Cour des comptes elles-mêmes dans son rapport de juin 2022 sur le soutien d'agriculture biologique, préconise d'augmenter les moyens financiers et humains des acteurs de cette agriculture par une mobilisation financière des interprofessions agricoles et par l'accroissement des subventions pour charges de service public, c'est pourquoi il est nécessaire de donner tous les moyens d'action aux acteurs du bio afin qu'ils puissent remplir leur mission transition des modes alimentaires, on a ici un mode un choix de société qui est devant nous, par sa position de fer de lance du développement de l'agriculture biologique, l'Agence Bio, et l'un des principal acteur son plafond de TP et les subventions pour charges de service public prévues sont restés stables, soit 19 TP et de 88 millions d'euros en 2023, mais ces moyens, c'est très clair, reste très insuffisant pour répondez efficacement à toutes ses missions. Le présent amendement vise à permettre à l'Agence Bio d'atteindre ses objectifs en rehaussant son budget de 9 millions d'euros permettant de doubler son plafond de TP, je dis bien 9 millions d'euros, à comparer au 8 milliards. Qui sont des coûts externalisés, des pesticides, donc il faut faire des choix et je compte sur vous pour les faire merci. le 1000000 d'euros dédié à la recherche de vaccins contre les épizooties afin d'anticiper d'éventuelles crise similaire à celle de l'influenza aviaire quand les maladies évidemment peuvent être traitées par vaccin à cette fin, nous procès nous souhaitons procéder à une augmentation de crédit de 9 millions d'euros, l'influenza aviaire n'est ni la première ni la dernière épizootie à laquelle neutre élevage est ou sera confronté, malheureusement et la recherche dans ce domaine, il me semble indispensable, comparé aux milliards d'euros de la Damned station depuis l'an dernier, cette hausse ne paraît pas exagéré, pardonnez-moi d'insister : un milliard d'euros d'indemnisation et dans ce budget, on propose un million j'ai envie dire un tout petit millions

Oui, monsieur le président, Monsieur le Ministre, oui, cet amendement est identique, mais je je tiens vraiment à appuyer face aux multiples épisodes si, comme la grippe aviaire, entre autres, il faut anticiper, il faut prévoir et cela passe par la recherche et tout particulièrement la recherche pour la vaccination, les crédits engagés en l'état, dans le cadre de l'action de santé et protection des animaux ne sont clairement pas à la hauteur des enjeux pour faire face aux risques sanitaires présent et ou à venir : l'agriculture doit être soutenu et sécurisé par la recherche et la science, la recherche prend du temps, il faut lui donner les moyens nécessaires, dès maintenant, telle est l'objet de cet amendement consigné par un certain nombre de mes collègues du groupe d'étude élevage et qui rejoint donc l'amendement précédent présenté par les 3 co-rapporteur, il vise à multiplier par 10 le 1000000, dédié à la recherche sur les vaccins, c'est du bon sens, car certes il vaut mieux prévenir que guérir. merci Monsieur le le président, cet amendement vise à accompagner le développement d'une filière industrielle de production de chambre en France je ne reviendrai pas sur l'ensemble des qualités les qualités du du chanvre et d'ailleurs un un de nos collègues le disait très bien, en rappelant que tout était bon dans le dans le chanvre et on voit bien que le renforcement de son développement agricole est indispensable sur de nombreux secteurs, que ce soit sur l'alimentation, la construction, le textile, le bio plastiques la papeterie et donc on a besoin de l'accompagner cette filière, c'était d'ailleurs l'objet de d'une résolution que nous avons voté largement ici, il y a quelques quelques semaines et donc la la le le besoin que on ait une politique publique et un accompagnement des pouvoirs publics, justement sur cette filière et on sait que pour mettre en place cette filière sur l'ensemble des départements, on a besoin, il y a besoin, notamment pour récolter le Champ de machines spécifiques, et donc on propose à un amendement qui prévoit un abondement programme d'adaptation des filières à l'évolution des marchés de 8 millions d'euros pour justement accompagner ce développement et permettre l'équipement des agriculteurs pour pouvoir justement mettre en place cette filière merci. Ensuite, l'amendement 278 qui le défend. Il est défendu, défendu. Monsieur du plomb ou Madame Ferrat, le 369 monsieur du plomb. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, le système d'information national d'enregistrement des moments d'animaux été va être modernisé, ça demande un effort financier qui aujourd'hui n'est pas véritablement mis sur la table et il semblerait qu'il manque 6 millions d'euros pour garantir le maintien des services réglementaire performant pour les opérateurs pour les tout ceci dans le cadre de la traçabilité de l'élevage français puisqu'on est en train de parler de la Base nationale des opérateurs ainsi que la bande à la base, dédié au moment des bovins donc ce cet amendement permet de pouvoir éclaircir la problématique du manque des 6 millions d'euros, en les mettant dans le budget de façon à ce que les opérateurs puissent véritablement faire les efforts nécessaires et être sûr que la totalité de leurs efforts sera financé.

un moment où, disait à traduire une préconisation faite par la Cour des comptes dans son rapport de juin 2022 sur le soutien de l'agriculture bio, il vise à augmenter les moyens financiers et humains des acteurs de l'agriculture bio, et plus particulièrement de l'Agence Bio, dont le rôle est central en matière de développement. De la promotion et la structuration de l'agriculture biologique français, il s'agit plus concrètement sur la base des préconisations de la Cour des comptes, d'augmenter le financement des actions de communication et de soutien au développement territorial de l'agriculture bio et de créer 40 équivalents temps plein, car le plafond d'emplois de l'agence reste stable, à hauteur de 19 équivalents temps plein, il faut rappeler que l'Agence Bio, à de nombreuses missions, en terme de communication de production et d'analyses de tests de statistiques de soutien des projets collectifs des agriculteurs mais constitue également une instance de dialogue entre l'amont agricole et l'aval industriel, son rôle est donc crucial, il apparaît aujourd'hui nécessaire de lui donner des réels moyens de remplir ses nombreuses missions. Ensuite amendements identiques, monsieur, monsieur l'abbé. Et Monsieur le président Monsieur Ministre, chers collègues, cet amendement vise à soutenir la recherche et l'innovation en agriculture biologique, le budget actuellement accordés à la recherche et au développement en agriculture biologique n'est pas à la hauteur des enjeux agricoles environnementaux ni du poids qu'occupe aujourd'hui l'agriculture bio dans l'agriculture française notamment tab l'Institut technique de l'agriculture biologique est largement sous-financé, c'est véritablement le parent pauvre des instituts techniques avec parfois même des difficultés pour exercer ses missions pourtant les enjeux sont majeurs pour améliorer la recherche de l'agriculture biologique et appuyer les agriculteurs dans le développement d'innovations agronomiques, social et durable tab est ainsi un outil formidable porteur d'une approche systémique multi-filières et transversale de l'agriculture biologique en lien étroit avec les agriculteurs de terrain, il a largement reconnu au niveau national, européen et international et mérite aujourd'hui d'être soutenus par l'État, comme le souligne le récent rapport de la Cour des comptes, publié en juin dernier. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, c'est un amendement qui vise à augmenter, a augmenté, pardon, les moyens alloués à la recherche, à l'innovation en agriculture biologique et de renforcer la coordination des travaux conduits pour mieux répondre aux attentes des professionnels et des agriculteurs, une demande faite par la Cour des comptes dans son rapport de juin 2022 sur le soutien de l'agriculture biologique, le budget actuellement accordés à la recherche et au développement de l'agriculture biologique n'est pas à la hauteur des enjeux agricoles environnementaux et climatiques que cela représente, ni du poids qu'occupe le bio dans l'agriculture française le présent amendement propose de débloquer un budget de 5 millions permettant de financer 10 sujet de recherche à hauteur de 500000 euros pour 3 ans, un investissement qui donnera de la force à des acteurs publics, de la recherche comme tape qui gère actuellement en coordination 60 projets cela permettra notamment d'inciter les autres instituts techniques agricoles ils interprofession qui les financent, à s'investir davantage dans les projets spécifiques à l'agriculture bio, de mettre en place un réseau d'établissements d'enseignement agricole exclusivement consacré à l'agriculture biologique, par exemple, merci. Le suivant monsieur Cabanel. Oui, merci Monsieur le le président cette un amendement identique à celui de ma collègue Préville le donc il a été défendu. Merci le 753 Madame Préville à nouveau.

l'agroforesterie est une technique qui associe les arbres à la production agricole, culture et élevage au sein d'une parcelle agricole cette technique ancestrale se pratique par la plantation de haies autour de la parcelle ou de manière hein intra-parcellaire, c'est-à-dire par la plantation d'arbres en alignement, l'objectif est à la fois économique et écologique en effet l'agroforesterie permet d'améliorer les rendements agricoles de manière significative à la lutte contre l'érosion des sols, elle permet la production de bois et donc de diversifier les revenus d'une exploitation les arbres Servent également d'abri pour les animaux, limite le ruissellement et contribue à la préservation des paysages aujourd'hui l'importance de la présence des et des arbres au sein des systèmes agricoles et de plus en plus reconnue en témoigne par exemple le plan national de développement pour l'agro-foresterie ainsi que le programme planton des du plan de relance de la France, qui prévoit de replanter 7000 kilomètres de sur la période 2021 2022, le développement de l'agroforesterie sur le territoire français, ne peut se réaliser que par la formation des agricultures et des agriculteurs ainsi que grâce à l'aide des conseillers techniques cet amendement propose donc d'allouer des fonds pour permettre la gratuité de ce service de conseil à raison d'un conseiller technique en agroforesterie par département : le budget global pour l'État nécessaires au financement de ce service est de 5 millions d'euros.

leur faisaient face, c'est leur travail, qui a permis à la France d'avoir l'une des agricultures les plus durable au monde pour sensibiliser les Français à ces âges et ainsi que valoriser les métiers, cet amendement vise à déclarer l'agriculture comme grande, grande cause nationale en 2023, c'est ce que j'ai exprimé tout à l'heure dans la discussion générale, ça faisait partie donc de la première proposition de notre rapport sur le mal-être des des agriculteurs, c'est assez symbolique, mais c'est un message fort que l'on peut faire passer, donc j'espère que vous pourrez, tout, tout sur tous les bancs, vous soutiendrez demain merci. Merci, ensuite le 833 Madame Barilla. Merci monsieur le président. Début novembre, la France est passée du statut de risque modéré à celui d'avérer vis-à-vis de l'influenza aviaire mon département de la Dordogne n'est d'ailleurs pas du tout épargnées, bien sûr, face à la virulence croissante de cette maladie dans le but d'éviter un pic épidémique épidémique de nombreux arrêtés préfectoraux ont été pris dans les territoires concernés afin de rendre obligatoires les auto-contrôles hebdomadaires sur les volailles élevées en plein air, mesures de surveillance de mortalité un élevage pour les élevages de plein air et mesures de surveillance des mouvements vers un établissement d'abattage, hé bien la difficulté, c'est que le coût du matériel nécessaire à la réalisation des prélèvements, ainsi qu'à leur conditionnement l'acheminement et les analyses de laboratoire sont à la charge du propriétaire, l'État ne prenant pas en charge ces contrôles si les éleveurs plein air comprennent parfaitement et ont conscience de l'importance de la lutte contre la propagation, elle a un coût important pour eux, qui ne peut pas être absorbé et qui, mais qui ne peuvent pas absorber et qui met en difficulté un grand nombre d'entre eux, qui craignent de ne pas pouvoir continuer leur activité, nous considérons que la lutte contre cette maladie ne doit pas mener à la disparition des élevages de plein air qui participe grandement la transition vers une agriculture durable, qui produit une alimentation de meilleure qualité, répète respectueuse, pardon, du bien-être animal et de l'environnement, c'est donc le sens de notre amendement qui prévoit le remboursement des auto-contrôles. Merci ensuite un amendement de monsieur l'abbé, le 800. Oui, un amendement identique qui a été très bien défendu par ma collègue en complément, le rapport de l'Inde cesse le montre, ce sont les fortes densités et les multiplications des mouvements d'animaux qui font exploser l'épizootie phénomène auquel ne contribue pas les filières de plein air.

un mot devrait arriver, mais dans un hiver, donc il y a encore quand même une année, on l'espère la moins complexe possible pour l'ensemble de nos éleveurs, moi même j'ai été l'été dernier chez un ami, éleveur de de canetons produit froid gras. Par ailleurs. On a abattu tout son cheptel, enfin il est pas cheptel pour évidemment les quand on met tout son groupe à l'indemnisation pour tous les éleveurs. neuf euros neuf euros si les gaver, évidemment, on est loin de ce que peut ramener un canard, y compris avec les fêtes, où on va avoir des très grandes difficultés, notamment sur le foie gras, donc nous proposons de de créer un fonds d'indemnisation de l'abonné. à hauteur de 5 millions d'euros, ce qui nous paraît pas une somme. Insurmontable, parce que nous considérons que dans la période, et ils ont subi.

De racheter les cantons, donc la question. Pour un fonds exceptionnel, le temps que le vaccin arrive de 5 millions d'abord parce que tout le monde n'a pas un ta indemniser et vous le savez, de 2022 ça traîne un peu et pour préparer, mais non, mais c'est une réalité, comme vous avez pas été indemnisés de 2000 22 et que vous attendez encore ça devient complexe sur le ministre faut entendre ça, donc nous proposons que d'abonder ce fonds exceptionnel de 5 millions d'euros, je vous remercie. Merci, ensuite le 740 monsieur Montaugé. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, chers collègues, cet amendement, toujours sur le même sujet, vise à créer une ligne budgétaire spécifique de 3 millions d'euros pour financer un plan d'accompagnement exceptionnelles de la filière pas Mickey palmipèdes gras mais un élevage extensif, voilà je je rappelle mes collègues l'ont fait, mais je voudrais le citer que dans un rapport qui a été rendu en juin 2022 c'est récent cesse fait bien une corrélation entre la densité des élevages et la survenance de crises, et je cite ce rapport à propos des des facteurs de surveillance là l'ANC s'écrit la densité des élevages de palmipèdes le Sud-Ouest et la grande diversité des espèces de volailles produite sur une même zone dans le Grand-Ouest avec le croisement de l'ensemble des activités d'élevage des intervenants et des mouvements de tous les maillons de ces, de ces filières, constituent des facteurs de survenance et il rajoute, il donc, en conséquence, je cite, une diminution durable de la densité des élevages de canards dans certaines zones, et un objectif structurel à moyen long terme, qui doit s'inscrire dans la révision des stratégies de développement et d'organisation des filières, il me semble qu'il y a là monsieur le le ministre de quoi, de quoi travailler mais je terminerai en vous disant, et vous le savez, je le sais que les la claustration obligatoire pour ce type de de petits élevages de petite taille et de faible densité est vraiment une une

par des pesticides dont les produits sont détruits déclassé ou qui se voient décertifier dans le cas de producteurs en agriculture biologique, particulièrement touchée par cet enjeu en effet quand ces contaminations sont constatées, il est bien souvent impossible de retrouver l'auteur des faits et son origine, ce qui empêche toute indemnisation au producteur. Le seul système existant à ce jour, et celui de la responsabilité civile du responsable de la contamination, cet amendement vise donc à proposer une indemnisation de ses producteurs afin de répondre à cette problématique qui génèrent des situations économiques et humaines très difficiles, il appelle aussi le gouvernement à mettre en place un outil pérenne qui pourrait être un fonds d'indemnisation s'inspirant du modèle FM est-ce nous ne pouvons laisser ces paysans sans solution, nous nous devons de sortir des pesticides, le plus rapidement possible et nous nous devons, dans l'attente de réponses à cette à ces situations. Un exemple, c'est le le sulfoxaflor ce pesticide très volatile, j'ai encore moins vite, madame la présidente, si vous me calmer très très volatile et qui contamine jusqu'à 2 hectares au moins dans ce dans son environnement, l'exemple d'un producteur de pommes bio qui s'est retrouvé déclassé et alors qu'il avait aucune responsabilité, mais il a pu, a rejeté sur qui que ce soit, d'où l'importance de ce type d'indemnisation, je vous remercie. Merci, cher collègue, je ne veux pas brider la présentation des amendements mais je vous rappelle qu'il reste une heure pour conclure la mission ce soir, à cette heure-là. Enfin, si vous voulez la conclure ce soir. Mais si vous voulez.

merci Monsieur le Président de 3ème, rapporteur. Voilà une 3ème larron voilà, vous avez raison, cet amendement vise à donner les moyens au Centre national de la propriété forestière d'assurer sa mission de dynamisation de la gestion de la forêt privée nous les rapporteurs, nous tenons à rappeler que c'est la forêt privée qui a brûlé à plus de 90 % cet été et nous appelons à renforcer les moyens du Centre national de la propriété forestière à hauteur de vingt équivalents temps plein pour déployer un réseau de référence de référent DFCI et accroître l'animation territoriale pour dynamiser la gestion de la gestion de la forêt privée aussi, nous appelons le gouvernement conjointement avec le sujet, bah si Madame Anne-Catherine Loisier monsieur Pascal Martin et monsieur Olivier Rickman, rapporteur de la mission conjointe de contrôle sur la prévention des feux de forêt a donné à la politique forestière, les moyens de ses ambitions un ETP est estimé en moyenne à 65000 euros, ce qui nécessite un 1000000 d'euros de hausse financé via la subvention pour charges de service public, montant de cet amendement, merci monsieur le président. Merci Madame Loisy amendements identiques. Oui, c'est un amendement identique, donc de la Mission de lutte contre les incendies, je, je soulignerai juste qu'il s'agit donc de soutenir l'autre grand Établissement public aménageur de la forêt privée française, donc on a 2 2 piliers qui compte seulement 350 ETP pour 12 millions d'hectares à gérer avec trop, plus de 3 millions de propriétaires donc un effort n'est vraiment nécessaire pour soutenir les forestiers privés. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, donc, cet amendement est proche des 2 précédents il vise également à renforcer les moyens humains du Centre national de la propriété forestière afin qu'il puisse mener à bien sa mission 75 % de la forêt et privée et représentent environ 23 % du territoire, or cette forêt est très morcelée, c'est un vrai une vraie problématique pour sa gestion et donc la mission du CNPF est absolument centrale les effectifs permanents ne sont que de 337 ETP le PLF 2023 prévoit 11 ETP supplémentaires mais qui ne sont pas financées dans le budget de l'état, donc nous proposons de financer ces 11 postes, ce qui correspond à un montant de 715000 euros, je vous remercie.

Merci monsieur le président, monsieur le ministre, il vise donc à à prévoir le financement des dès 11 postes déjà précédemment présentés voilà.

Merci, si si c'est la même somme dans les trois amendements, ensuite le 772. Ce qui pas. Il y a personne pour le défendre monsieur Tissot, le 743. Oui, monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, toujours pour la bio, cet amendement vise également à traduire l'une des recommandations de la Cour des comptes dans son rapport de juin 2022 sur le soutien de la grippe bio, il s'agit d'augmenter les moyens alloués à l'appareil statistique en matière d'agriculture biologique moyen qui sont actuellement insuffisants au vu des besoins, en effet, nous estimons que pour permettre un développement efficace de ce secteur, il est essentiel et nécessaire d'évaluer les politiques publiques mises en oeuvre et d'engager un appareil statistique plus performant pour les politiques publiques, futur de plus ces données devront être publiés afin d'éclairer le consommateur dans ses choix les données de l'agglo sont encore trop opaque et n'encourage pas le consommateur à la consommation de produits bio, le présent amendement propose ainsi d'allouer une enveloppe supplémentaire de 1 1000000 d'euros afin de financer les les équivalents temps plein, nécessaire pour faire remonter et consolider les données économiques de l'agriculture biologique en lien avec l'Observatoire de formation des prix et des marges. Merci ensuite Monsieur Salmon le suivant. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, il s'agit du même amendement, je pense que la biodiversité s'effondre et pourtant beaucoup continuent de regarder ailleurs, il est grand temps d'examiner tout cela de près avec des vrais observatoire afin d'établir les responsabilités car il ce n'est pas dans 10 ans qu'il faudra s'étonner un peu comme pour le réchauffement climatique, que l'on a rien fait, merci. Merci monsieur Cabanel. Amendements identiques donc défendu. Monsieur Montaugé le suivant un an monsieur plat. cet amendement propose de financer la généralisation d'une prise en charge par l'État du remplacement d'exploitants agricoles en cas d'urgence, cette expérimentation concluante, a été mise en place dans l'Orne, il est proposé ici de la généraliser, afin de prendre en charge le financement du coup de l'adhésion au service de remplacement quand l'exploitant n'est pas des rats, ainsi que le coût du remplacement, selon le service de remplacement France sur le coût de cette généralisation sur l'ensemble du territoire s'élèverait à 735000 euros pour l'État pour une seule année dans le président tu amendement vise donc à le financer. Merci, et enfin le dernier de cette discussion commune Monsieur des plus élémentaires de la vie, c'est-à-dire essayer de manger à sa faim et par ailleurs permettre à nos compatriotes, par leurs achats de de produits agricoles français en vue de que nos agriculteurs vivent mieux, avant tout, je rappelle que nous nous sommes prononcés depuis très longtemps pour une revalorisation des salaires et en particulier pour une robe à la réalisation substantielle du SMIC, mais le gouvernement s'y oppose systématiquement, je vous rappelle que le président de la République avait promis en 2020 la mise en place d'une aide par chèque alimentaire mais, pour d'obscures raisons techniques, monsieur le ministre des Finances n'a pas trouvé les moyens de présenter de le présenter au PLF 2023 alors que madame la première ministre, on avait fait début de ses fonctions au début de ses fonctions, alors Monsieur le ministre, il s'agit d'un amendement d'appel bien entendu visant à vous inciter à aider nos agriculteurs en faisant en sorte que, pour un coût modique sur le projet, un chèque alimentaire soit créée par défaut, en vue d'inciter les futurs ayants droit à acheter les produits agricoles français, en attendant que vous puissiez convaincre la première ministre de décider une réalisation générale des salaires et des minima sociaux en faveur de nos concitoyens l'amendement semble avoir été entendu puisque, par anticipation, puisque tout à l'heure, vous nous avez annoncé une enveloppe de 60 millions d'euros pour ce projet. Merci donc je vais demander maintenant au rapporteur de nous donner leur avis sur ces 76 amendements. Bien.

c'est donc comme je vous l'ai dit, lors de la discussion générale, une demande de retrait sinon alors, ceci étant, on est absolument conscients y a un problème au niveau de des grossistes et de la restauration collective aujourd'hui sur l'application de la loi Egalim les hausses de charges, et Très bien, là je j'évoque le 829 848 736. C'est très particulier, comme cette manière d'examiner, je pense qu'il faudrait qu'on revoit les années prochaines, 846 il y a là 5 amendements concernant l'accompagnement des structures gérants des cantines scolaires pour pouvoir maîtriser les coûts de D. les familles, fixée pour les familles, c'est une démarche qui est légitime, bien évidemment, regarde notre rejet en commission des finances nous sommes appelés à vous demander le le retrait et j'appelle votre attention sur le fait qu'on a parmi ses amendements donc de qui sont à une accompagnement à 20 centimes et d'autres à 40 centimes si on ne veut pas siphonner certains programmes qui gage la mesure il vaudra mieux s'il y a vote favorable qu'il porte sur la le financement à 20 centimes, même si ça n'est pas nécessairement suffisant merci. Donc toujours pour continuer dans la restauration collective, le 832 rectifié le 737 rectifié le bis, donc ça c'est pour un plan d'et étendre le plan de relance aux cantines scolaires à l'ensemble des départements, régions et grandes villes, donc c'est un une demande de retrait. Sur le 783 concernant le curage des retenues d'eau, là aussi, on a affaire, un sujet majeur sur le plan à la fois agricole sur le plan écologique, avec un peu problématique d'acceptabilité et la nécessité de redéfinir un cadre légal de la même manière, le, le sujet est clairement légitime la demande est fondée, mais au regard de la position de la commission des finances, notre proposition et de rejet, Sur la question de la distillation pour prendre en compte les problèmes de stocks aujourd'hui en matière de vin il l'écoulement de ses de ses productions pour les raisons évoquées : c'est un retrait. Pour le 780 rectifié bis concernant le fonds de compensation pour les sociétés vitivinicole, touchée par la sur taxation c'est bien sûr une demande de retrait, compte tenu du montant. Nous avons 15 amendement concernant les effectifs de l'ONF et donc que les propositions de recrutement d'agents pour soit resté au niveau de l'année précédente de 2000 fin de l'année en cours plutôt 2022, soit pour redonner des moyens humains à à à l'ONF dont on sait que l'en charge de la forêt dans ses diverses fonctionnalités à la fois, production de bois mais aussi tout ce qui relève des services et éco-systémique et donc qui relèvent des missions de service public et qui par ailleurs nécessite effectivement pour exercer des pouvoirs de police donc de d'avoir la qualité de de fonctionnaires, j'ai une remarque à faire, c'est que les propositions vont de 1 1000000 à 300 et quelque 231 pardon millions pour pouvoir remettre à niveau l'ONF si d'aventure l'amendement retenu était le plus élevé, on s'il faudrait effectivement le programme enfin le programme concerné qui gagnerait cette mesure, ce qui conduirait à

Retrait et s'il y a un vote sont les remarques que j'ai évoqués. On est sur lequel 370 pour toute Pour tous les amendements ONF, vous avez bien compris ça, une demande de retrait. 852 rectifié bis, l'aide pour les paysans, victimes de la sécheresse et exclus du dispositif actuel d'indemnisation, c'est une demande de retrait puisqu'on a mis en place un système assurantiel et avec une participation de l'État sur le sujet longuement parlé. Sur la question de la à l'aide d'urgence au à l'agriculture biologique aux exploitations en difficulté, c'est le 844 la proposition est une proposition de retrait, même si, effectivement, aujourd'hui, il a besoin, c'est réel, compte tenu des difficultés qui ont été évoquées, compris par le ministre dans son propos liminaire. S'agissant des du plan national donc, le 850 à concernant le plan national, en vue de la réduction des émissions d'ammoniac notamment et de protoxyde d'azote, plutôt notre avis et tu as un avis de retrait pour les raisons évoquées sur le plan sur la position de la Commission, néanmoins, effectivement, le sujet est un sujet réel. 847 pardon les projets alimentaires territoriaux qui, aujourd'hui, effectivement, se développe sur le territoire national, qui permettent de d'avoir une approche une une territorialisation de, de, de l'agriculture en quelque sorte qui vient en complément d'approche filière qui était celle qui a été dominante au et prégnante au cours de ces dernières décennies et qui est à mon avis, utiles à la fois pour le l'agriculture est également pour le consommateur. 516 rectifié donc renforcement de la recherche appliquée en matière agroalimentaire a beaucoup parlé, c'est tout de même une demande de rentrer, compte tenu de la vie qui a été prononcée, même si nous sommes conscients que c'est indispensable. Le 742 et 3 autres avenants amendement pardon identique concernant l'un plan de communication à l'agriculture biologique, on a évoqué effectivement le fait que la culture biologique, en tout cas la consommation de produits biologiques est en baisse depuis 2000 vas question de savoir s'il s'agit de quelque chose de conjoncturel ou 2 structurelle et donc, là, là aussi, le sujet est devant nous, la communication nécessaires pour eux relancer la la demande, je lui dis, vous l'évoquiez, mais pour la raison, proposition de retrait au regard de la position de la commission.

donc c'est la création d'un programme, un plan de déploiement des PDG pour 20 millions d'euros, donc c'est une demande de retrait, bien sûr, même si la gestion de l'eau sera un sujet à suivre. Sur le 788 et également le 845 2 amendements identiques sur l'aide au maintien en agriculture biologique, effectivement, cette aide a a disparu et la Cour des comptes dans son rapport évoqué effectivement la nécessité d'accompagner l'agriculture biologique,

c'est aussi une demande de retrait, même si c'est indispensable, nous en sommes bien d'accord. C'est que enquête coopératives du du TO-DE aux coopératives d'utilisation du matériel agricole, c'est une demande de retrait, vous imaginez bien, si l'ensemble des entreprises demandent ça certes nous allons répondre à beaucoup d'attentes en terme de prestations et de coûts mais je ne suis pas sûr que le système tienne. le 367 portent sur l'augmentation de la situation pour service public de bénéficier enfin au profit des des chambres compenser la hausse du point de rémunération la demander et légitime et néanmoins demande de retrait pour les raisons. évoquer 741. Plan d'accompagnement durable de l'élevage extensif, le sujet est devant nous, sur le développement de d'une diversité en en matière de modalité de de production mais demande de retrait pour les mêmes raisons. 773 rectifié, c'est toujours un amendement de contournement du plafond du casse d'armes donc idem demande de retrait. Alors 4 amendements identiques à partir du 745 concernant une dotation de 9 millions en faveur de l'Agence Bio, pour augmenter ses effectifs et donc permettent de renforcer et d'accompagner l'agriculture biologique, dont on connaît les difficultés récentes de ces dernières années puisque l'évolution de la demande n'est plus là, celle qu'on a connu, il a la croissance s'est arrêtée et, donc, pour les mêmes raisons, pour ces quatre amendements demande de retrait. Amendement 368 9 millions d'euros pour la recherche de vaccins contre l'épizootie, donc c'est une demande de retrait, même si nous sommes complètement d'accord que c'est indispensable d'y penser 777 rectifié, même chose. Donc je continue 763 dotation de 8 millions pour la filière du chanvre idem demande de rentrer 278 rectifié bis, même chose 369 numérisation et adaptation des bases de gestion des informations d'identification demande de retrait. Il s'agit de le 744 concerne une dotation de 5 millions d'euros pour la recherche en agriculture biologique, c'est une préconisation de la Cour des comptes, l'amendement et est fondé, au moins sur c'est à travers cette cette préconisation mais demande de retrait au regard de la position de la commission des finances.

de sensibilisation au sujet de la, de l'agriculture pour en faire une grande cause nationale en 2023 la question de la reprise et la transmission des exploitations est un sujet qui est devant nous, avec près de 300000 exploitations perdus en 20 ans, et donc le sujet est réel, l'enjeu est important néanmoins retrait pour les raisons que vous connaissez. Donc je passe au 833 rectifié et le 849 le remboursement des auto-contrôles hebdomadaires des volailles, donc c'est une demande de retrait, la ville peut être déjà deviné. La prochaine fois. Le 835 rectifié fonds d'indemnisation de la grippe aviaire, auteur de 5 millions demande de retrait. Plan d'accompagnement exceptionnelles de la filière palmipèdes gras demande de retrait. Excusez-moi, c'était le 740 rectifier 851 rectifié, même chose. 371. Retrait Retrait on rejette la mission, hein, je ne sais pas si vous m'avez entendu au départ, mais comme on rejette ça sert à rien, malheureusement qu'on retienne des amendements hein 771 rectifié, même chose. C'est tous 731 rectifié, même chose, enfin vous avez compris, voilà, c'est sur l'ensemble des amendements, on est obligé de les retirer puisqu'on rejette la. Trois amendements identiques à partir du 743 806 et 822 il s'agit d'améliorer l'appareil statistique en matière d'agriculture biologique, les données sont nécessaires si on veut pouvoir faire un pilotage adéquate sérieux des politiques publiques menées c'est légitime mais demande de retraite pour les raisons que vous pouvez

Je vais essayer de faire une voix, ce qui a été fait à 2 voix, donc en essayant de donner des éléments sur un certain nombre de sujets, alors je les je les prends par quasiment identique, simplement j'ai parfois un peu rajouté des choses, je prends le le paquet alimentation donc cantine restauration collective les P hâter le chèque alimentaire ça me permettra de faire une réponse globale, c'est les amendements, monsieur le Président, 172 768 855, 829 848 736 846 832 737 et les amendements 847 et 720 sur les AT et le chèque alimentaire d'abord vous dire que c'est vrai que c'est un sujet de préoccupation pour nous tous, à la fois liée à l'inflation et la fois aussi ou lié à l'organisation d'abord vous dire que quand même on a, on ne part pas de rien, puisque le plan de relance 50 millions sur la partie investissement ou dans les cantines scolaires, c'est vrai que je ne sais plus quel sénateur a dit que ça avait pas été saisis par les collectivités, donc c'est pas la question forcément des moyens, il y a parfois une question de mobilisation qu'il faut qu'on accélère il disons que c'est un élément important, deuxièmement 80 millions pour les projets alimentaires territoriaux et puis par ailleurs, ce que j'ai dit dans le PLF 2023 60 millions pour une aide alimentaire durable voter avec le ministère des solidarités pour accompagner les plus démunis en attendant ce que ce soit, quoi, vous m'avez déjà interrogé à plusieurs reprises la question du chèque alimentaire, je l'ai dit tout à l'heure, il me semble qu'il faut qu'on réfléchisse différemment la question du chèque alimentaire par rapport à ce que on essaye de lui faire faire, on essaie de demander aux chèque alimentaire, de tout faire : produit de qualité produits de proximité commande publique modération du coup, organisation des filières ici le bio là le végétal, la, la, la, enfin bref, on ne peut pas tout faire avec un seul objet, donc il faut qu'on essaye de travailler sur un travail, un travail collectif dessus mais qui permettra de structurer quelque chose qui soit multi-peut être multi-entrées, il me semble que d'ailleurs on devrait pouvoir travailler dans la restauration hors domicile sur un certain nombre de sujets, puisqu'on sait que, principalement, c'est là qu'on peut orienter un certain nombre de choses pour faire en sorte que dans la commande publique, on puisse avancer, donc il me semble que là on a un travail à faire, je dis d'ailleurs sur la commande publique on que j'essaie de porter au niveau européen, une évolution de la réglementation des marchés publics sur ces sujets-là, comme sur d'autres, en tout cas sur ce sujet-là, parce que ce serait un élément qui permettrait de débloquer les choses enfin quelques éléments sur le pâté pour dire que

et par ailleurs dans France relance dans le volet agriculture le guichet agriculture de regarder si ça permettrait pas de prolonger les projets alimentaires territoriaux, on sait les freins Organisation des producteurs collecte logistique et donc on a besoin de travailler sur tous ces sujets, voilà sur l'ensemble des sujets disons qu'on a des dispositifs à l'oeuvre faut qu'on avance sur les AT mais on a des dispositifs et donc c'est pour toutes ces raisons, sur l'ensemble des sujets, j'ai oublié d'évoquer, pardon le que le gouvernement a mis en place un dispositif d'aide aux familles les plus démunies, je la je pense aux plus petites communes qui permet à l'objectif de répondre à l'objectif de l'accessibilité, c'est le dispositif cantine à un euros et disons que c'est un élément qui permet de pondérer de modérer le coût des tarifs à chacun de pouvoir s'en saisir, c'est aussi j'ai été maire, président de PCI c'est aussi à chaque collectivité de s'en saisir, on voit bien qu'il y a des choix qui sont de nature différente donc sur tous ces sujets-là. C'est une demande de retrait, sinon c'est un avis. Je prends pardon dans cet ordre là les questions de l'eau qui a été évoqué en particulier par le sénateur Montaugé si j'ai bonne mémoire 2 amendements, l'un sur le eu l'autre sur les les les curage des retenues d'eau sur les pété je on est déjà quelque chose qui se développe puisque la volonté, c'est bien de faire en sorte que les petites je puisse se développer, je vous dire quelque chose, jeux, on demande aux agriculteurs de les faire, ils le font souvent de bonne foi et avec la volonté de construire des, des, comment dirais-je, des compromis territoriaux, si c'est pour qu'à la fin, ils se retrouve au tribunal et on a quand même un sujet, je le dis très simplement, c'est une démarche dans lequel on a incité les agriculteurs à aller en disant : essayer de concerter, c'est dialoguer et essayer de mettre tout le monde autour de la table non mais on a besoin quand même on partage je crois d'ailleurs la vous la volonté mais la volonté, ça peut pas être simplement de dire : on se met autour de la ta pour qu'à la fin on dise finalement : je signe pas l'accord, il me semble que dans un certain nombre de cas et on l'a vu récemment sur les débats qu'on a eu plutôt dans la région Poitou-Charentes, non, non, mais il faut faire les PDG GE mais il faut inviter tout le monde quand même une fois qu'on se met dans la démarche et essayer d'avancer, et quand on a signé en bas d'une feuille. Qu'on était d'accord pour pas après, revenir au tribunal pour dire je suis plus d'accord, parce que ça c'est des sujets qui viennent un peu agacé la volonté souvent pragmatique des agriculteurs d'avancer sur la le curage des retenues existantes, on est d'abord c'est pas forcément une question de de financement c'est une question pour moi de réglementation qu'il faut qu'on assouplisse ou qu'on clarifie sur un certain nombre de sujets, notamment les autorisations versus les autres modalités et c'est là-dessus qu'on est en train de travailler pour essayer d'assouplir les choses, il y a une grande masse, c'est vrai, vous avez raison d'eau qui peuvent être mobilisés dans ce cadre-là. Sur la question des de des fonds dédiés à la distillation, ça c'était l'amendement 786. Retrait sinon défavorable 2ème sur la question de la distillation, c'était plus là pour J'en ai parlé non. J'espère que je suis clair. Mais. Sur la question là l'amendement 786 monsieur temps urnes sur la question du fonds dédié à la distillation de 140 millions d'euros d'abord, il me semble que, il faut qu'on regarde avec raison, quand même, c'est des Budgets qui sont immenses, par ailleurs, il me semble que dans une année où on a pu produire quand, en 2021 on a subi gel et que la question, c'était plutôt de ne pas avoir de stock, y compris pour couvrir des marchés intérieurs domestiques ou des calories à l'extérieur, je suis pas sûr que l'heure soit pour le coup à la distillation, il y a des outils de régulation par ailleurs qu'il faut qu'on essaye de développer, ne semble pas, donc ça c'est un avis défavorable la compensation sur les surtaxation portée par la sénatrice Delattre en particulier, impossible de vous dire, à cette heure, même si on est en décalé de six heures ce qui est en train de se passer, l'objectif c'est bien de prolonger

la sénatrice disait à juste titre, il faut qu'on traite l'ensemble des problèmes si on met 200 millions pour la distillation 200 millions parce qu'on a des pénalités, j'entends aussi les demandes pour certains d'arrachage, on va finir par arriver à des chiffrages qui va être compliqué, on a besoin, moi je pense, d'avoir une philosophie globale, en particulier sur le le les secteurs que connaît bien la sénatrice de l'autre, qui sont les secteurs du Bordelais, j'en viens à la série sur l'ONF. Alors d'abord pour saluer le travail, je le dis très simplement qu'il a fait l'ONF alors madame la la la la, sénatrice Préville c'est toujours intéressant de vilipender le gouvernement qui est en place, vous avez dit : je ne sais plus, je crois que c'est le président Gontard, qui a dit : 6000 postes supprimés 1000 depuis 2017 donc 5000 avant 2017, alors j'entends que tout le monde veut se racheter peut-être de ce qui n'a pas été fait avant 2017,

l'idée de : on va faire mieux avec moins, c'est intéressant, mais c'est un concept souvent donc la volonté du gouvernement, vous avez dit il faut arrêter l'hémorragie, ben, c'est ce qu'on fait dans le budget 2023 avec ce qu'on avait mis en première intention et ce qui a été votée à l'Assemblée nationale 10 plus 10 millions d'euros, ça va permettre de couvrir ses besoins là j'entends ce qui a été dit sur les vins, madame la sénatrice sur les les vins de restants, ils sont financés sur les ventes et la commerciale et la contractualisation ONF et donc il me semble que là nous avons fait une un 1er signal qui est un cinéma de stopper l'hémorragie, et c'est vrai qu'il y a eu une hémorragie et donc chacun doit prendre ses responsabilités sur le sujet, on essaye de le faire sur la DSI, il me semble d'ailleurs que dans le contrat d'objectifs que nous avons à retravailler avec l'ONF, il faudra que, après, on se dise quelles sont les missions qu'on veut conférer à l'ONF et après quels sont les moyens et pas à verser parfois la chose, mais moi je pense aux agents de l'ONF, qui pendant des années on à la fois vu la baisse des effectifs, et au fond, parfois le sentiment qu'on ne savait pas ce qu'on leur demander, il y avait un problème de sens et donc on a besoin de travailler sur les objectifs, le sens et le travail qu'a à faire, l'ONF, c'est d'ailleurs valable, je dirai tout à l'heure, et donc c'est des moyens, mais c'est aussi qu'est ce qu'on veut faire sur la défense de la forêt contre un incendie sur la replantation et la reforestation il y a des tas de choses, j'ajoute que dans France relance un certain nombre de missions, y compris sur la replantation qui vont être financés, y compris pour l'ONF, ça a été évoqué tout à l'heure donc, sur ces sujets-là, c'est une demande de retrait, sinon c'est un avis défavorable mais il sent qu'on ne on est dans une prise de conscience collective, reconnaissons-le, de la nécessité de stopper l'hémorragie trois de mettre en adéquation, ce qu'on demande l'ONF je, je le dis, les agents de l'ONF ont trop souffert de cette absence de vision pour qu'on on ne se préoccupe pas de cette question, c'est un premier élément, madame la sénatrice, j'entends bien, et vous connaissez bien ces sujets que vous ne soyez pas satisfaite de ma réponse,

donc ça c'est les amendements 838 131 762 790. 778 733 805 789 780 684 817 779 370 770 et 732. Comme on nous donne le temps restant je j'accélère les choses, les dispositifs d'indemnisation, monsieur le sénateur, la bé je crois que c'est vous qui l'avait porté pour le alors on a derrière on a un dispositif assurantiel, qui a été votée à l'Assemblée et au Sénat, qui me paraît solide, la question c'est de rentrer dans les critères quand on rentre dans les critères, c'est-à-dire celui d'avoir été pénalisé par un incident grave type une sécheresse ou autre, on rentre dans les dispositifs où on y rentre pas mais il y a pas besoin d'un dispositif parallèle, il me semble que les dispositifs qui sont posées, donc c'est un avis défavorable sur l'agriculture biologique simplement dire que, puisque là il y a une il y avait toute une série d'amendements, ne les voulais que leur Monsieur le Président, 844700. On les reprendra après dans les explications de vote, allez-y donnez vous explique. C'était un avis de du monde de retrait parce que d'abord on il y a beaucoup de choses qui sont faites, j'ai entendu ce qui était demandé sur le maintien, il y a le crédit d'impôt, c'est pas 20 millions c'est plus de 100 millions qui sont projetés, il y a là de la conversion, c'est plus de 35 % d'augmentation dans la PAC, donc il y a des éléments, il y a un besoin de communication, je le dis très simplement ici au Sénat, pour vous dire, je suis prêt à ce qu'on regarde, qu'on mette des moyens complémentaires à l'agence sur la communication, mais c'est pas 500000 euros, sans qu'on ait un plan de communication qu'il faut qu'on travaille ensemble. c'est pas comme avant cette affaire-là, on voit bien qu'on a un sujet aujourd'hui de de demande est plus un sujet d'offre et donc on a besoin aussi de se mettre en remettre en cause sur le plan de communication qu'il faut qu'il qu'on doit mettre à l'heure parce que, manifestement, la crise ne justifie pas seulement la question de la baisse ou du risque de demandes, donc c'est un avis d'une demande de retrait pour l'ensemble de ces amendements non c'est un avis défavorable, monsieur le sénateur Labbé, c'est un avis défavorable sur le 850 Monsieur le Sénateur de plomb sur le programme sur la l'article sur le casse d'art, j'ai déjà dit les éléments qui font que, on va bien récupérer, en 2000-là dans les là 2023 le restant de crédit 2022, il nous appartient, effectivement, de mieux mobiliser ces crédits j'ajoute qu'on vous avez beaucoup parlé du CASDAR, mais dans France 2030 je déploie tous les jours avec l'INRA et avec des des programmes d'investissement dans l'innovation et la recherche qui viendront compléter utilement les fonds de caisses défavorable sur le 739 défavorable sur le 367 sur les champs d'agriculture ce le sénateur du plomb, je crois que c'est vous qui en avait parlé, je connais bien les chambres d'agriculture pour les raisons que vous savez comme vous d'ailleurs, enfin, pour d'autres raisons, je suis très attentif aux besoins, je, je vais voir dans les jours qui viennent, le président des chambres d'agriculture, vous regardez la question d'émission, les missions de service public, qui a des missions près agriculteurs mais il y avait aussi des missions de service public, ils sont réinterrogé par le contexte particulier des, des, l'augmentation des salaires dans les chambres et c'était bien légitime, donc on va regarder dans les jours prochains, mais à date, c'est un avis défavorable défavorable et je regarderai avec le, le, je m'y engage sur la l'influenza aviaire simplement un élément sur les élevages de petite dimension, moi je m'appuie sur ne cesse et et pas à la carte Lanxess nous a donné des éléments, vous avez rappelé pour un certain nombre d'entre vous, moi, je suis assez favorable à ce qu'on regarde, j'ai demandé à l'ne cesse de nous faire des propositions pour regarder si dans les petits élevages y avait pas des choses nous posons pas non plus, c'est aussi dramatique pour un petit éleveur que pour un grand de perdre son élevage et de noirs abattu pour tout le monde, c'est la même cause : vous avez, vous m'avez interrogé sur la vaccination, on est en train de faire une expérimentation, j'espère avoir des résultats, c'est vous, monsieur le sénateur Guy et on espère avoir des résultats au mois de, au mois de décembre, janvier qui nous permettra de qualifier et mettre en place un plan de développement pour l'année suivante, il y a aussi la question de fabrication des vaccins et de quel type d'animaux, on pourra vacciner pour être bien sûrs de leur utilité, donc c'est une demande de retrait, sinon c'est un avis défavorable sur le chambre 763 278 ces 2 avis défavorable sur le 369 c'est une demande de retrait de Monsieur du plomb sinon défavorable sur l'agroforesterie, d'abord, on est dans des sujets c'est madame la sénatrice Préville on est dans des sujets qui sont soumis à concurrence d'ailleurs, il y a pas que les gens de l'agriculture qui interviennent sur l'agroforesterie

et pour cause, en en forêt privée 75 %, la forêt française simplement vous dire que le plafond d'emploi augmentera de 11 ETP, ce qui va permettre à l'opérateur de mettre en CDI, des gens qui étaient en CDD et par ailleurs, leur budget en 2023 va augmenter de 1 virgule 3 millions d'euros avec une subvention supplémentaire d'1 virgule 3 millions d'euros, sans doute, il faut faire des effets de rattrapage plus long mais on ne peut pas dire que nous ne faisons pas l'effort, donc c'est une demande de retrait sinon défavorable et enfin le 734 de monsieur Montaugé sur la génération la prise en charge du remplacement des exploitants, c'est un travail que nous aurons à mener, me semble-t-il, globalement, dans la loi d'orientation et donc c'est une demande de retrait sinon défavorable mais il me semble que c'est un sujet sur lequel nous pouvons travailler parce qu'on a besoin de regarder comment on essaye de stabiliser dans les exploitants, ça fait partie des sujets de bien-être au travail et et de mal-être, en corollaire retrait sinon défavorable voilà monsieur le président. Merci, monsieur le Ministre, donc sur l'ensemble des amendements, il y a des demandes de retrait ou des avis défavorable pour les raisons que la commission expliqué et avec les arguments qu'a donné le ministre madame la présidente, Prima avant qu'on ordonne la discussion sur les explications de vote. Si Monsieur le Président, je voudrais attirer l'attention de tous nos collègues qui sont encore là ce soir pour vous dire qu'il nous reste très peu de temps, d'ici la fin de la mission, donc nous avons 2 choix soit nous passons au vote sans explication de vote et nous allons peut-être avoir une chance de finir ce soir, soit on lance des explications de vote, on ne lancera que les premiers, c'est clair et je pense qu'il n'aura pas grand monde, samedi, pour entendre les explications de vote sur les autres amendements, donc évidemment c'est la liberté de chacun des parlementaires voilà si on pouvait ne pas faire d'explication de vote sur les avis peut être qu'on gagnerait on gagnerait du temps, je vous laisse libre de votre choix, mais évidemment il me semble que c'est plus raisonnable de finir ce soir. Alors Madame Cukierman rappel au règlement. Merci monsieur le président, monsieur Miss, mes chers collègues, pour un rappel au règlement, il n'y aura pas d'explication de vote s'il le faut, simplement pour vous rappeler tout de même ce qu'on pourrait en rire, mais en fait, là je crois que ce soir je suis mais nous sommes en colère, d'abord nous sommes et ce n'est pas pour être sic. Nous sommes au Parlement, le lieu où nous parlons, et où nous pouvons échanger nous examinons ce soir le la mission Agriculture ça te faire le France dont tout le monde sait se targuer quand il le faut, de ces femmes et de ces hommes agriculteurs qui, au quotidien, donnent de leur temps pour travailler et dont chacun sait ici sur tous les bancs, loués éventé leur travail au quotidien ce qu'ils font, par une discussion commune alors c'est la faute à personne, bien évidemment, j'ai même envie de saluer les rapporteurs, qui sont sont sortis comme ils ont pu, ce n'est pas la faute à la séance, ce n'est pas la faute à ceci, mais en tout cas, force est de constater que plus de 70 amendements qui vont des enjeux de la restauration à l'ONF à la gestion de l'eau, c'est vrai qu'on a eu un si bel été tellement pluvieux que il y a pas de souci, José voilà à la viticulture qui n'est qu'accessoire, puisqu'elle permet à notre agriculture d'être excédentaire à toutes les à tous les enjeux de l'ONF, c'est vrai qu'il y a pas de débat de la fourrure sur la forêt dans notre pays en ce moment et à tant d'autres que je ne vais même pas pouvoir énumérer ici, parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir finir tous ensemble et nous allons-y arriver, il n'y a pas de souci, c'est certainement la magie du Sénat, nous sommes dans une situation où, sur la les surtout ces armements notre groupe comme tous les autres ne peut même pas justifier ces votes, ce qui pose également. Un déni de démocratie, parce que oui, nous n'allons pas demander des scrutins publics mais nous avons un rendez compte sur un certain nombre d'amendements et sur ce que les uns et les autres peuvent voter pour, contre, nous avons un débat, c'est la démocratie, donc moi, très sincèrement, j'invite tous les collègues et nous le ferons à faire remonter à nos groupes et a interpellé pour que nous ayons une véritable réflexion et à avoir un véritable débat dans le cadre du projet de loi de finances digne de ce nom. bien, chers collègues, acte et donner de votre rappel au règlement, je pense qu'effectivement chacun est interpellé par la situation, donc il y aura peut-être des discussions à avoir sur la manière de, de, de, de faire je, je pense que chacun l'a dit à sa manière, alors ceci étant dit, il nous reste un peu de temps, donc je vous propose que par groupe d'amendements sur les mêmes thèmes on essaye quand même de dire 2, 3 choses : il peut y avoir des amendes et des explications de vote groupé, donc je vous propose d'abord pour les prendre dans l'ordre. Il y a les amendements qui vont de l'amendement numéro 172 à l'amendement 737, c'est-à-dire les amendements qui porte sur la restauration collective. Est-ce que sur ces amendements de manière groupée pour pas les prendre un par un, est ce qu'il y a des explications de vote.

alors je je comprends la proposition du du président effectivement de le faire par paquet, mais on sait très bien que si on engage une explication de vote sur des sujets dans lequel on a que ça soit sur la cantine scolaire, ce soit sur la question de l'ONF, on en a pour un peu plus de temps et que de toute façon, on n'y arrivera pas, donc c'est pas, c'est pas sérieux, mais ce que je voulais dire c'est que j'ai pris la parole et j'ai fait un rappel au règlement sur la sur la la mission juste d'avant pour la même problématique, c'est-à-dire qu'on a fini une mission où là, on avait même pas d'explication de vote quand même, hein, on a, on a balancé des amendements comme ça les uns après les autres, problème vraie problématique sur le temps qui est imparti par rapport à assez passe par rapport à ses missions, et le fait qu'on puisse les discuter correctement et franchement quand on voit les sujets, je ne vais pas redire ce qu'il a dit Cécile Cukierman, évidemment, elle a la question de l'agriculture, on a des agents de l'ONF, qui étaient devant les portes du Sénat pendant 2 jours, où là il y a un vrai enjeu où ils ont besoin d'explication et qui sont présents et que je salue, effectivement, je pense qu'ils avaient besoin qu'ils avaient envie d'écouter nos arguments de savoir pourquoi j'ai entendu ce qui a pu dire ce qui a pu dire, Monsieur le Ministre, d'ailleurs je lui rappelle quand même que le contrat d'objectifs et les 2021 2025 et que même si on arrête l'hémorragie, comme vous dites, ce ce contrat d'objectifs, il a été fait en accord avec le gouvernement et avec votre gouvernement, donc à un moment donné, OK, je comprends que vous avez compris que c'était peut-être pas dans ce sens-là qu'il fallait aller mais très bien, j'en prends acte, ça veut dire qu'on va revoir ce contrat d'objectifs qu'on va changer les choses et qu'on a enfin compris qu'on avait besoin d'un véritable service public de la forêt qu'on a besoin d'agents et qu'on avait besoin de fonctionnaires, c'est une bonne chose, voilà merci. Bonhomme et Monsieur Rémy.

Mais bon enfin on va. Pas entamer le débat là-dessus là, dans ces conditions là, mais il y a des possibilités d'y joindre le débat d'amendements, ça dépend aussi de la commission des finances n'a pas le choix qui a été fait, donc il y a un amant du donc on met en discussion commune tous les amendements qui pompe sur les mêmes missions parce que si on les adoptait un parrain, le premier amendement adopté fait tomber tous les autres alors que là, tous les amendements ont été présentées, donc les tous les systèmes ont des avantages et des inconvénients, mais on a ses inconvénients, parce qu'aussi on a un temps contraint. Daniel Gremillet oui monsieur le président je vais être très bref, vu les conditions, je retire mon amendement.

sur certaines d'entre eux parce que, parce que ce sont les nôtres, ça va aller sur d'autres, ça va être beaucoup plus compliqué, quoi, voilà donc c'est on est dans une situation ubuesque, ubuesque, je pensais pas un jour en tant que sénateur,

Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je vois qu'il y ait un peu d'énervement, c'est normal la nuit avance. Moi je pense qu'on est au bout du système voilà je, je vous le dis tranquillement, je vais prendre une minute, je pense qu'on est au bout du bout. 49 3 à l'Assemblée nationale ici. Première partie : moi j'ai pas fait beaucoup, enfin, j'ai assisté à un truc là sur la première partie où la majorité sénatoriale vote des amendements à juste raison gouvernement arrive dit bon voilà. C'est bien, mais on va faire une 2ème délibération c'est vous-même qui allait porter ça, moi j'ai vu des choses incroyables. Des gens se lever et dire : je suis d'accord avec l'amendement que j'ai défendu heureusement et je vais voter contre la deuxième débat et non mais voilà, on en est là pour équilibrer les comptes, puis après on passe à une deuxième partie. C'est l'humiliation du Parlement, je vous le dis comme ça quoi tranquillement où on n'a pas le temps de débattre, enfin bon on va pas se refaire dans ces conditions là, on va retirer tous nos amendements, ce qui est ce qui concerne notre groupe ce qu'on a même pas le temps de les voter, et puis bon, voilà, je retire ensuite celui sur la deuxième partie cinq six mais franchement, c'est pas une très belle image du Parlement qu'on donne ce soir et on vote quand la mission, voilà ce qui nous concerne, chacun faisant ce qu'il souhaite, après moi, je pense qu'il faut qu'on ait un vrai débat, là je pense que c'est le dernier budget qu'il faut qu'on fasse comme ça et je pense que c'est une urgence démocratique la démocratique parce que. Honnêtement, quand nous regarde, si les Françaises et Français nous regardent parce qu'ils sont outrés et chaque parlementaire qui est ici, quelle que soit 100 sensibilité, on ne peut pas être satisfait de ce qu'on vient de faire, franchement, je vous remercie, monsieur le président Je le président, Monsieur le Ministre, pour dire à peu près la même chose que mon ami Fabien. Je l'ai dit tout à l'heure, on était dans le brouillard, déjà au début donc ça pouvait pas être mieux à la fin, ça c'est le 1er point le 2ème, c'est que le but de ce que nous avons fait, c'est de faire entendre au ministre les positions qu'on a. Qu'on les prenne ou qu'on les prenne pas de toute façon on va rejeter la mission donc retirant la totalité de nos amendements, rejetant la mission, le ministre a entendu ce qu'on avait à dire sur les différentes propositions, vu qu'ils feront un 49 3 hé ben on leur remettra le singe sur l'épaule et il prendra les responsabilités de maître, ce qui voudront dans le 49 3. Monsieur Menonville ah non, pardon, madame Loisier. Même explication et même traitement avec beaucoup de déception sur ce que l'image que le Sénat donne ce soir mais nous retirons nos amendements.

ça me chagrine quand même beaucoup quoi ce sur sur ces, sur ces aspects-là, il y a des, des gens qui attendait des réponses et je sais bien que les sujets sont différents et qu'on a tous des sujets importants, je pense qu'on avait quand même un message envoyé, sur la question notamment de l'ONF, j'ai vu qu'il y avait des amendements, grosso modo, notamment un qui était partagée par l'ensemble des groupes qui avait une majorité et qu'qui pouvait en tout cas à trouver une majorité, il me semble que c'était un signal assez fort qu'on pouvait envoyer donc voilà, moi je, je regrette qu'on en qu'on a et c'est vrai que je regrette aussi l'image qui peut être donnée ce soir quoi. Madame Lienemann. Moi, je comprends bien l'attitude de colère, ce qui m'ennuie dans cette affaire, c'est qu'il a quand même Laurent Duplomb disait de toute façon, on va pas voter la mission et le gouvernement fera 49 3 c'est pas tout à fait la même chose de définir des avis et, sur certains sujets à voir un vote important du sénat parce que le message transmis n'est pas de même nature, je pense à la nécessité de consolider les postes de l'ONF, par exemple, voire de développer les choses, un vote n'a pas la même valeur et chers collègues, c'est pas la première fois, c'est pas un incident de séance j'ai présidé dans la même situation que Pierre Laurent, des débats du même ordre, où j'ai mis une demi-heure, a expliqué que le règlement du Sénat faisait que quand on avait un si on n'était pas en discussion commune le premier amendement faisait tomber tous les autres, parce que les chiffres de la mission était déjà complètement donc c'est structurel dans la manière de penser le le débat budgétaire, c'est donc un débat lourd à régler, mais la première des choses, c'est le temps, parce que ce qui nous a pas permis de travailler sérieusement, c'est le temps qui est trop limité, donc la première chose à revendiquer, c'est ça : je prends acte du fait que vous semblez tous d'accord sur l'idée qu'il vaut mieux retirer moi j'aurais aimé un vote du Sénat sur les créations de poste à l'ONF.

on avait voulu aller à au bout du débat, il fallait reporter à samedi. Vous vous décidez de ne pas reporter à samedi, donc nous allons être dans la situation effectivement de retirer les amendements et de procéder à un vote global sur la mission, madame la présidente. monsieur le président, moi je comprends la colère, je la partage parce qu'il y a beaucoup de travail derrière tout ça il y a énormément de travail de chacun de vous des administrateurs de la commission des finances de la commission des affaires économiques sur un sujet comme l'a dit Cécile qui est un sujet majeur, et Dieu sait si le sujet de l'agriculture ici au Sénat, et quelque chose que nous connaissons que nous travaillons et pour lequel nous avons tous dans nos diversités de penser un engagement extrêmement important parce que c'est la même de nos territoires, ceci étant dit, ce soir, on ne va pas évidemment pouvoir voter dans des conditions qui soient optimales, moi je voudrais dire, et notamment je voudrais m'adresser aux agents de l'ONF, qui sont ici ce soir, ne pensez pas que parce que ce soir on ne va pas pouvoir voter les crédits de la mission Agriculture que nous ne serons pas à vos côtés et je pense que, à la fois par les explications du ministre par l'engagement de tous les groupes politiques qui ont été ici nous montrons notre engagement à l'agriculture pour les chambres d'agriculture pour les projets territoriaux pour l'ONF pour le CNPF pour la forêt pour certains dans d'autres bancs pour l'agriculture biologique pour la transformation pour la restauration, qui représentent des enjeux économiques et des enjeux pour nos collectivités territoriales, les enjeux, ce soir, c'est des enjeux tant on est pressé par la discussion budgétaire générale par les autres missions que nous aurons de demain, après-demain, et donc nous sommes dans cette situation, mais je veux dire ici à tous les intervenants et à toutes les parties prenantes de l'ensemble de la mission agriculture que le Sénat continue et continuera à travailler sur toutes les problématiques. Bien donc je repose une dernière fois la question est-ce que tous les amendements sont retirés, est ce qu'on passe à un vote global sur la mission. Oui,

Par le groupe, les républicains sur les crédits de la mission. Je vous rappelle que l'avis de la commission est défavorable. évidemment, le gouvernement lui est favorable, il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement, le scrutin est ouvert.

Plus personne ne demande à voter.

votants 343 exprimés 293 pour 55 contre 238. Le Sénat n'a pas adopté. Nous avons encore quelques votes à émettre, donc je vous demande de rester, on va finir avant deux heures. Donc je mets aux voix déjà l'article. 41 c'est qui suit la mission que nous venons de voter. Qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté ensuite, il y avait plusieurs amendements articles additionnels, donc qu'est-ce que ces amendements sont maintenus.

Qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté. Et ensuite, nous procédons. Oui au vote, excusez-moi du des crédits du compte spécial développement agricole et rural.

Je vous rappelle que l'avis de la commission est défavorable. évidemment, le gouvernement lui est favorable, il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement, le scrutin est ouvert. Tout le monde est d'accord pour le même vote. Donc même votre. Ce qu'on a Que la demande de scrutin public et retiré oui voilà, donc même vote sur les crédits du compte spécial. Il est donc rejetée, mes chers collègues, je vais lever la séance, la prochaine séance aura lieu le jeudi 1er décembre à 10 heures 45 pour l'examen de la mission Immigration, asile et intégration du projet de loi de finances pour 2023 la séance est levée.